La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente Fuentès séance a été distribué, il n'y a pas d'observation, le procès verbal donc adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à d'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. La parole est d'abord à monsieur Daniel Gremillet rapporteur pour le Sénat de la CMP pour cinq minutes. Monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente chère Sophie. Mes chers collègues. La CMP sur le projet de loi sur le nouveau nucléaire est parvenu à un accord. Je me réjouis de la reprise de la plupart des apports sénatoriaux. En effet, la commission des affaires économiques avait souhaité compléter le texte selon 4 axes, premièrement. Notre commission a estimé indispensable d'actualiser la planification énergétique, c'est pourquoi le Sénat à l'article 1er a entendu abroger les 3 verrou à la relance du nucléaire issu de la loi, transition énergétique de 2015. L'objectif de réduction à 50% de l'énergie nucléaire le plafond des autorisations de 63 2 gigawatts et la trajectoire de fermeture des 14 réacteurs inscrite dans la PPE. C'est aussi le Sénat qui a introduit de nouveaux objectifs en matière de recherche et d'innovation. Et d'hydrogène nucléaire à l'article 1er bé c'est enfin un cinéma qui a inscrit la relance du nucléaire dans la prochaine loi quinquennale de l'énergie afin que cette loi fixe un objectif clair de construction pour les EPR de les SMR en précise les moyens à l'article 1er pour garantir la neutralité technologique à l'article 1er, nous avons obtenu que le SMR bénéficient des mesures de simplification. Et que les autres technologies dont les électrolyseurs et d'hydrogène fasse l'objet d'une clause de revoyure dans un délai de 5 ans et pour renforcer le contrôle parlementaire. Nous avons prévu une réédition des comptes du corps au gouvernement devant le Parlement dans un délai d'un an, puis tous les quatre ans. Deuxièmement notre commission a voulu renforcer la sûreté et la sécurité nucléaire à l'article 9 bis. Nous avons intégré la résilience au changement climatique, dont la démonstration de sûreté des réacteurs tant au stade de l'autorisation que du ré-examen et la cyber-résilience dans leur protection contre les actes de malveillance. C'est une première et c'est crucial à l'article 4. Nous avons prévu que les travaux pouvant être anticipée par l'exploitant soit défini par décret après avis de l'ASN. Je tiens à remercier ici le rapporteur pour avis Pascale Martin pour avoir défendu cette idée à mes côtés à l'article 9, nous avons prévu que le exploitant remette un rapport quinquennal sur la sûreté. Dans le cadre du ré-examen refusant une réorganisation mal évaluée et mal anticipé de l'ASN. IRSN que le Sénat n'avaient pu examiner nous avons supprimé toute référence à une éventuelle réorganisation aux articles 9 à 11 bis et en Laissons-nous le temps Madame le Ministre de l'expertise sur ce sujet majeur en parallèle nous avons consolidé les attributions et le fonctionnement de la commission des sanctions de l'ASN aux articles 11 11 bis et 15. Enfin nous avons alourdi et compléter les peines en cas d'intrusion dans les centrales nucléaires à l'article 13. Troisièmement, notre commission entendu. Des collectivités territoriales et le public soucieux du principe de participation duplique. Nous avons interdit la construction de nouveaux réacteurs avant l'achèvement du débat public ou de la concertation préalable à l'article 2. Attachée à la protection des compétences et des finances locales. Nous avons obtenu l'extinction des réacteurs Dusan pour les collectivités territoriales et le recueil. De. Et le de leur observation sur l'évolution de leurs documents d'urbanisme aux articles 2 et 3. Dans le même esprit nous avons garanti à ces collectivités territoriales, au bénéfice de la taxe d'aménagement à l'article 3. Dernier axe, notre commission a souhaité renforcer la sécurité juridique. Il s'est agi de mieux définir les procédures de en matière d'urbanisme ou d'expropriation notamment aux articles deux 3 et 7. L'autre enjeu a été de compléter ses procédures en proposant une régularisation de l'instance à l'article 7 bis pour accélérer le règlement contentieux sur les nouveaux réacteurs et on entend en introduisant une clause de revoyure à l'article 5 pour encourager l'enfouissement des infrastructures du réseau de transport d'électricité. Au total, notre commission entendu porter une vision résolument moderne de l'énergie nucléaire plus complexe et plus actuel intégrant pleinement les risques climatiques et numérique, qui sont les enjeux du sec. Ce faisant, et la donner un aboutissement législatif très concrète et très con concret et complet aux recommandations de sa mission d'information transpartisane sur NRJ et l'hydrogène nucléaire de juillet dernier que j'ai conduite avec mes collègues Jean-Pierre Moga et Jean-Jacques Michau. Je voudrais aussi remercier. Ma collègue rapporteur de l'Assemblée. Nationale Maud Bregeon et du travail qui a été fait et les concertations que nous avons ensemble pour effectivement arriver à ce compromis je invite à adopter ce texte de compromis et forme le voeu que la prochaine loi quinquennale sur NRJ qui doit être présenté d'ici. Mi-2023, acte véritablement la relance du nucléaire, je l'espère profondément Madame la Ministre d'avoir une stratégie énergétique pour notre pays. Je voudrais remercier particulièrement aussi toute l'équipe. Que s'soit Alexis Ambre Clément associé aussi Coralie qui était encore avec nous. Sébastien et madame la présidente, et tous les membres de la commission économique qui ont fait un travail formidable. À mes côtés, merci. Madame le Ministre, vous avez la parole. Madame la présidente, madame la présidente de commission. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Vous avez une nouvelle fois la responsabilité de vous prononcer sur un texte majeur pour bâtir l'indépendance énergétique de notre pays. La responsabilité de vous prononcer sur un texte qui contribuera au défi de ce siècle libérer notre pays de sa dépendance aux énergies fossiles. La responsabilité, enfin de vous prononcer sur un texte qui permettra à notre pays de produire une énergie abondante compétitive et décarboner. L'objectif du gouvernement est claire, atteindre la nuque la neutralité carbone d'ici 2050 en réduisant drastiquement notre consommation de pétrole et de gaz fossile qui pèsent encore pour près des 2 tiers de notre consommation d'énergies fossiles, pour réussir l'immense défi de long terme de se libérer des énergies fossiles nous devrons construire un consensus politique qui transcende les étiquettes partisanes car je vous le dis avec conviction. Notre politique énergétique ne peut pas se permettre de subir à nouveau les atermoiements et les décisions erratiques qui ne se fonde ni sur la science, ni sur la raison et qui parfois dépendent d'accord électoraliste de circonstances. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Je suis convaincue que nous posons depuis l'été dernier les fondations d'un pacte de renouveau énergétique un pacte qui permettra de faire face à l'urgence climatique. Il y a l'urgence énergétique. Un pacte qui repose sur des discussions nourries et approfondies entre le gouvernement et le Parlement mais également entre le gouvernement et les élus locaux. Les organisations environnementales, les entreprises et plus largement l'ensemble des Français. Je vais d'ailleurs en profiter pour saluer les milliers de nos concitoyens qui ont contribué à la grande concertation sur le futur mix énergétique de notre pays. Je me réjouis qu'ils s'emparent de ces sujets qui sont certes complexe mais déterminant pour notre avenir. L'énergie est aujourd'hui au coeur du débat public est au coeur de nombreux travaux parlementaires que vous avez initiée c'est donc essentiel que nous y travaillons ensemble car comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire, il n'y aura pas d'indépendance politique sans maîtrise énergétique. Après le vote des textes sur la sécurisation de nos approvisionnements énergétiques. L'été dernier sur l'accélération de la production des énergies renouvelables en début d'année je souhaite avec le projet de loi d'accélération des procédures administratives nucléaire poursuivre la relance de notre filière nucléaire. Je me réjouis de l'accord trouvé en commission mixte paritaire. Je tiens particulièrement à remercier les rapporteurs, le rapporteur présidente, Sophie Primas. Et les autres membres de la commission mixte pour leur investissement jusqu'à la dernière minute qui a permis ce succès c'est un signal fort envoyé à notre filière pour qu'elle se mobilise en vue du lancement du programme de construction de six EPR de et de la mise à l'étude de 8 complémentaires et ne nous interdiront pas d'aller plus loin en fonction de la réalité de nos capacités industrielles. Vous le savez également l'enjeu des compétences est au coeur de la transition énergétique. Cela est particulièrement vrai pour la filière nucléaire. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la filière de dresser un état des lieux précis des besoins en compétences pour réussir la relance les résultats de l'étude qu'ils ont réalisés sont limpides. 100.100 1000. Voilà le nombre d'emplois que la filière estime nécessaire de recruter au cours de la prochaine décennie, des soudeurs, des chaudronniers, des tuyauteurs, ou encore des ingénieurs autant d'opportunités au coeur des territoires pour les jeunes ou les travailleurs en reconversion de prendre part au plus grand projet industriel de notre pays depuis les années 70, ce seront les visages de cette France nation verte que nous appelons de nos voeux. Dans le prolongement de ce travail je également le point avec l'université des métiers du nucléaire début juin sur la stratégie de formation qu'elle mettra en oeuvre pour répondre à ses besoins de compétences. Ce projet de loi sur le nucléaire matérialise plus profondément le soutien du gouvernement et du Parlement et une politique énergétique ambitieuse et crédible. Je me félicite. À ce titre de notre fut tout au long de l'examen de cette loi d'opposer nucléaire et énergies renouvelables car notre urgence je le répète et de sortir des énergies fossiles et nous aurons autant besoin du nucléaire que des énergies renouvelables pour y parvenir. Avec ce projet de loi nous accélérons également le renforcement de l'ensemble de notre filière permise notamment par la montée au capital d'EDF, les investissements pour moderniser notre outil de production comme à Framatome, au Creusot. Dans la continuité du plan de France relance et avec le plan France 2030 pour investir dans les innovations en matière nucléaire. Cette ambition je la porte, au-delà de nos frontières je m'emploie en effet depuis plusieurs mois réunir nos partenaires européens au sein d'une alliance du nucléaire civil. Nous sommes désormais 14 membres à travailler aux côtés de la Commission européenne pour que l'énergie nucléaire trouve la place qui lui est dû, dans le mix énergétique européen. Je réunirai la semaine prochaine, mes homologues à Paris pour faire le point sur les projets européens de nouveaux investissements dans le nucléaire et on sera surpris d'en connaître le nombre. C'était également tout le sens de mon déplacement il y a quelques jours aux côtés du président directeur général d'EDF. Luc Rémont sur le chantier britannique de l'EPR d'Hinkley Point, pour défendre notre savoir-faire d'excellence à l'export. Mesdames, et messieurs les sénateurs voté définitivement ce texte et permettre à notre pays de réaliser une grande avancée écologique en mobilisant tous les leviers de décarbonation pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est aussi donner l'opportunité à notre pays de conjuguer. Réindustrialisation et maîtrise énergétique s'est lancé le chantier du siècle en matière industrielle et d'emploi. La prochaine loi de programmation énergie climat dont je vous détaillerait prochainement la préparation devrait être ambitieuse et réaliste, au regard de nos capacités, je serai la garante. Je vous invite donc à poursuivre, et je nous invite à poursuivre ce travail collectif initié pour bâtir la souveraineté énergétique de notre pays. Je vous remercie. Nous passons maintenant aux explications de vote, des groupes à raison d'un orateur par groupe et nous commençons avec Monsieur avec Jean-Pierre Corbisez pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. pas. La présidente madame un ministre monsieur le rapporteur, madame la présidente. Mes chers collègues. Une fois n'est pas coutume, c'est un texte largement amputé des modifications apportées par le Sénat qui nous est présenté aujourd'hui. Une situation que je trouve fort regrettable dans la mesure où je reste persuadé que nombre de ces ajouts avec toute leur pertinence. En 1er lieu il est dommageable à mon sens d'avoir retiré à l'article 1 l'ensemble des objectifs fixés par le Sénat en termes quantitatifs notamment sur nos ambitions concernant la part de matières recyclées dans la production de l'énergie nucléaire. Les intentions engage les objectifs oblige. Nous aurions même pu aller plus loin sur la question de la réutilisation du combustible au regard du contexte de tension que nous connaissons aujourd'hui dans l'acheminement de ce type de matériaux, tant en raison de la raréfaction de la ressource que du contexte géopolitique tendu. Certes le rapport prévue par l'article 1 des à l'horizon des 5 prochaines années est de bon ton et aborde ces questions. Mais toute cette évaluation n'aura-t-elle pas dû être fait en amont. Notamment pour éviter un débat dans la précipitation, comme c'est malheureusement souvent le cas avec le gouvernement qui a pris la mauvaise habitude de tordre le bras au Parlement en imposant des procédures d'urgence et des délais contraints. Le propos est le même, s'agissant du rapport prévue à l'article 1 F.. Ces études et ces analyses aurait dû être réalisé en amont et soumise aux parlementaires afin de leur permettre de se prononcer en étant parfaitement éclairée. À titre individuel est toujours à l'article 1. Je regrette le retrait de la mention des installations d'hydrogène bas carbone comme susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi. Nous passons d'un côté, je pense d'une possible accélération des procédures en la matière en contradiction selon moi avec des potentialités de cette énergie. Par ailleurs, sur le fond, nous sommes tous d'accord pour dire qu'en matière d'énergie, il nous faut conquérir notre autonomie qu'il nous faut travailler mieux et plus vite. Nous savons aussi que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Et la simplification et l'accélération de nos procédures de pas se faire au détriment du débat parlementaire, ni en enjambant la consultation des citoyens, ou encore en réduisant notre niveau de vigilance et d'exigence quant à la préservation de notre environnement et de la biodiversité. De ce point de vue la suppression des dispositifs nouvelles réunies sous le titre renforcer la transparence démocratique sur le nucléaire doit nous interroger. En outre la multiplication dans le texte de la CMP des rapports que devra produire le gouvernement ne souhaite remplacer les investigations que peuvent mener directement les parlementaires via une délégation. Une opportunité ratée de redonner plus de place aux députés et aux sénateurs. Si j'étais taquin, oserais-je dire que nous sommes encore étonné. Saluons malgré tout le maintien de l'information préalable du département et de la région sur les projets de création de nouvelles installations. Une attente forte de nos collectivités, en raison notamment des responsabilités du département en matière de route et de sécurité incendie ou des implications sensible pour les régions en termes d'équilibre territorial. À noter également une mise en cohérence du texte, suite au débat à l'Assemblée nationale avec la réécriture de l'article 9 pas l'adaptant à la décision de nos confrères député de retirer du texte intégration de l'IRSN à l'ASN. Au-delà des inquiétudes légitimes des personnels, cette fusion n'était pas opportune au regard des missions spécifiques de chacune des autorités et en raison de la sensibilité très particulière du domaine de l'énergie nucléaire qui justifie selon moi de maintenir séparés les missions de contrôle et celle d'expertise et de recherche. qu'on va enfin la nouvelle disposition intégré à l'article 3 concernant l'objectif de zéro artificialisation nette. Nous savons toutes et tous. C'est un sujet très sensible pour lequel d'ailleurs nous attendons toujours les propositions du ministre en charge des collectivités. Mais je pense que nos collègues élus locaux seront rassurés que les projets d'installations de réacteurs nucléaires ne sont pas comptabilisés dans les objectifs régionaux ou locaux de réduction de l'artificialisation des sols. Nous respectons la la logique de ne pas pénaliser le développement de nos collectivités territoriales pour des projets d'envergure ou l'intérêt national. Ah, bilan mitigé. Vous l'aurez compris, dressé par notre groupe dans le prolongement des avis émis lors des discussions préalables général et parce que le sujet est d'importance et parce qu'il nous faut collectivement prendre nos responsabilités pour faciliter l'autonomie énergétique de notre pays, notre groupe votera majoritairement en faveur de ce texte. Merci. Merci. La paroi les maintenant à la présidente, Sophie Primas. Pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur. Chers Daniel mes chers collègues. Le projet de loi nouveau nucléaire dont nous examinons les conclusions de CMP aujourd'hui est important, il est très important. Cela faisait bien longtemps que l'énergie nucléaire n'avait pas été placé au centre de l'attention publique. Je rappelle que la dernière autorisation de création remonte à 2007. L'énergie nucléaire dans notre pays, devenue était devenue un problème quand nous pensons ici depuis longtemps au Sénat que c'est une solution une solution pour notre indépendance énergétique afin de sortir des hydrocarbures russes, en particulier avant 2030 et de faire face à l'électrification. De tous nos usages une solution pour notre transition énergétique afin d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais Madame la Ministre que de temps perdu depuis 2007 du temps perdu pour servir des intérêts politiques plus que pour servir l'intérêt de notre pays. Politique d'attrition réacteurs existants. Programmation de l'arrêt de 14 réacteurs sur 20 arrêt du programme Astride fermeture de Fessenheim en 2020 des fautes qui nous ont privés de vision d'avance en matière de recherche qui nous ont privés de souveraineté technologique de compétences de capacités énergétiques et de performance climatique Fessenheim à elle seule, c'est une production manquant de 11 TWh, ce sont 10 millions de tonnes de CO2 en plus dans l'atmosphère. À cela s'ajoute une politique d'attentisme du gouvernement s'agissant des nouveaux réacteurs depuis 2017, aucune décision décisive n'a été prise ni lors de la planification énergétique par la loi énergie-climat de 2019 ni dans l'APP de 2020. Résultat notre système électrique est aujourd'hui en vigilance particulière sur le plan de la sécurité selon RTE et sans marge sur le plan de la sûreté selon l'ASN. À contrario, la commission des affaires et comme. Économique s'est mobilisée avec constance en faveur de l'énergie nucléaire dans la loi énergie-climat de 2019 nous avons décalé de 10 ans. Le calendrier de fermeture des réacteurs existants, sous réserve bien sûr de sûreté dans la loi climat résilience de 2021, nous avons conditionné tout autre fermeture à la prise en compte de la sûreté nucléaire, de la sécurité d'approvisionnement et des émissions de gaz à effet de serre. Daniel Gremillet son rappelle ce fut une bataille dans la loi énergie renouvelable de 2023 nous avons introduit des mesures de simplification pour l'hydrogène, quelle que soit sa source renouvelable comme nucléaire notre commission s'est aussi largement mobilisés dans ses travaux de contrôle dont la mission d'information transmet transpartisane évoqué tout à l'heure. Daniel Gremillet, a ainsi plaidé pour construire 14 EPR de SMR afin de maintenir un mixte majoritairement nucléaire à l'horizon 2050. Quelle clairvoyance. Mais quelle opiniâtreté. Instruite par l'expérience. Notre commission a reçu positivement le projet de loi est considérablement infléchi et enrichi le texte qui portera clairement la patte l'empreinte du Sénat. Elle a complété les procédures techniques par une vision politique en actualisant nos objectifs énergétiques nationaux et la future loi quinquennale sur l'énergie. Nous serons attentifs à ce que cette loi comporte des objectifs ambitieux, des moyens suffisants au au-delà à ce que le gouvernement clarifie sa stratégie acte les constructions des prochaines installations instruisent les autorisations, précise leur financement notre commission ainsi promue une vision moderne de l'énergie nucléaire intégrant de nouveaux risques climatiques numérique et de nouvelles technologies Les SMR les électrolyseurs d'hydrogène. Elle a ainsi encouragé une vision décentralisée de l'énergie nucléaire attentive aux compétences et en particulier d'urbanisme et aux finances locales. Je me félicite que Senna est obtenu l'exemption des réacteurs des objectifs locaux et régionaux Dusan ce fut Madame la Ministre vous le savez une longue et difficile bataille nous serons très vigilants à ce que le gouvernement ne réintroduise pas par voie législative voire réglementaire. L'objectif d'objectif national pour ses projets notre commission enfin soutenu une vision exigeante de l'énergie nucléaire. Soucieuse de la sûreté des réacteurs et la gestion des déchets. Et bien entendu je suis satisfaite que le Sénat est obtenu le retrait total de la réorganisation de l'ASN et de l'IRSN dans ce texte présenté à l'Assemblée nationale par amendements gouvernementaux improvisée sans étude d'opportunité d'impact sans concertation. Nous avons ici d'ailleurs initié une saisine de l'Opecst pour comprendre les objectifs qui était sous-jacent et évaluer la réponse idoine. Nous serons très attentifs à ce qu'une éventuelle réforme ne viennent pas confondre les responsabilités ou déstabiliser les compétences. C'est cette vision d'une énergie nucléaire fondée sur la science et la raison inscrite dans le monde actuel est ouverte sur les technologies futures que notre commission a poursuivi, c'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains votera les conclusions, cette CMP.

Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues si le rapporteur. moi j'ai pu le dire lors de l'examen en première lecture de ce projet de loi ici au Sénat, le nucléaire c'est l'histoire d'une ambition française qui s'est transformé en véritable stratégie. C'est une aventure industrielle qui a connu un sérieux ralentissement lors des 2 dernières décennies et à laquelle nous avons décidé de donner un souffle nouveau. Nous avons bâti notre stratégie nucléaire sous l'idée d'une sécurité d'approvisionnement et la recherche de notre indépendance énergétique. Après les chocs pétroliers des années 70, la guerre en Ukraine nous a rappelé notre dépendance aux énergies fossiles et les risques d'un abandon de cette filière. Pour autant notre souveraineté énergétique, il faudra couper le nucléaire au déploiement massif d'énergies renouvelables. L'engagement devra être franc et massif en conservant un cap constant. Madame la Ministre, nous devons absolument nous donner les moyens économiques et politiques de conserver cet engagement le programme paraît ambitieux des investissements lourds, mais le prix de notre indépendance. Par ailleurs, notre planète est également confronté à un dérèglement climatique que personne ne peut ignorer. Vous connaissez l'engagement de mon groupe. Pour une écologie pragmatique. Il est de plus en plus urgent d'abandonner les centrales à charbon et autres sources d'émissions de gaz à effet de serre. L'avenir c'est obligatoirement un mix énergétiques bas-carbone produire de manière indépendante. Oui. Produire proprement et de manière indépendante. 1000 fois oui. Il est donc essentiel d'investir massivement dans la maintenance, la rénovation et le renouvellement de notre parc nucléaire si malmenée depuis trop longtemps par des politiques contradictoires totalement inadapté. Je me félicite que le texte issu de la CMP entérine la suppression de l'objectif de réduction de 50% de la part du nucléaire dans notre bouquet énergétique à l'horizon 2035. Poursuivons nos investissements dans la recherche, l'innovation et la formation. Un secteur majeur pour l'avenir de la France. À ce titre le nucléaire nouvelle génération est une belle perspective, je pense bien sûr à tout ce qui est SMR ou EPR. Je suis également préoccupé par les lire nécessaire que nous devons créer afin d'harmoniser notre politique énergétique nationale. Avec les orientations politiques européennes. En ce 9 mai de l'Europe, cela a tout son sens. Je connais votre engagement Madame la Ministre sur ce sujet. Soyez assuré dans notre soutien. Il en va de même d'ailleurs sur le dossier de l'hydrogène bas-carbone qui est intrinsèquement lié à celui de la taxonomie. Ne passons pas à côté de la possibilité de décarbonation de notre économie pour laver plus Vert que Vert. Le GIEC nous exhorte à nous servir de nos énergies bas-carbone pour réduire nos émissions. D'hydrogène produit à partir du nucléaire est une chance pour le pays et pour l'Europe même aussi dans le monde ne partage pas du tout cette analyse. On a du mal à trouver une cohérence dans leur politique actuelle. Puisqu'il vient de fermer leurs trois derniers réacteurs nucléaires et annonce dans le même temps une fermeture totale des centrales à charbon en 2038. Comprenne qui pourra.

nous permettant d'aller dans le sens de notre souveraineté et notre indépendance européenne. Je parlais à l'instant d'innover. Et de décarboner nos modes de vie. Le nucléaire, l'hydrogène bas carbone constituent un espoir bien réel pour réduire drastiquement les émissions des secteurs comme les industries très émettrice type Syrie ou encore les transports. Sur ce dernier point, je suis de près le développement de l'aviation de l'avion à hydrogène notamment et les programmes d'incorporation de biocarburant dans le kérosène pour les gros porteurs dans le cadre lorsque l'Opecst avec mon collègue député haut-garonnais monsieur Portarrieu. Nous préparons un rapport sur ce sujet. Dans cette optique, le groupe les indépendants. Il sera donc très attentifs au projet de loi sur l'industrie verte, ainsi que sur celui de la programmation énergie climat. Madame la Ministre le texte que nous discutons aujourd'hui est extrêmement encourageant mais restons vigilants. Je pense à la sûreté et à la sécurité, où nous avons besoin de transparence et de la plus grande fermeté. Sur la formation professionnelle, le travail sera important. Nous avons besoin d'ingénieurs, certes en nombre mais aussi de technicien, d'autres filières professionnelles doit être renforcé pour que la. Relations c'est efficace. Nous devons agir vite. Parce que ce texte est le début d'un renouveau énergétique comme vous l'avez dit, madame la Ministre. Le groupe les indépendants votera en sa faveur. Merci la parole maintenant état Daniel Salmon pour le groupe écologiste solidarité et territoires.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente des affaires économiques. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Nous continuons à contester fortement l'opportunité, les modalités et les objectifs de ce projet de loi. Les propositions et modifications qui figurent dans ce texte constitue une régression du droit de l'environnement une atteinte au droit de participation du public au mépris des textes en vigueur. Il va bien au-delà de son objet initial et devient un texte programmatique. Nous déplorons vivement la suppression de 2 jalon majeur de la politique énergétique française. Introduit en 2015, l'objectif de réduction du nucléaire à 50% et l'article qui limitait la puissance installée à 63 2 gigawatts cela dans un souci de diversification du mix électrique et de maîtrise des coûts de production. Ces suppressions constituent des cavaliers législatifs. En inscrivant votre volonté de construire 14 réacteurs de type EPR2 dont l'ingénierie n'est toujours pas abouti et de SMR, qui sont encore à l'état de prototype. Vous. Vos engagements de respecter le débat sur la programmation énergétique à venir et ne respectait pas non plus les conclusions des débats publics qui viennent de s'achever. Si nous sommes bien lucide sur la nécessité de devoir faire encore un moment avec les centrales existantes. Notre position sur la construction de nouveaux réacteurs reste entière. Doit-on rappeler une nouvelle fois les déboires technologiques et les débordements financiers invraisemblable de cette filière des défaillances graves s'enchaînent. Ces dernières semaines avec la découverte de nouvelles fissures d'une ampleur inégalée sur les scènes de. Et quatre nomme. Vous persistez dans le mensonge de l'indépendance énergétique en maintenant la France sous perfusion des pays fournisseurs d'uranium naturel et d'uranium enrichi russe en particulier. Vous avez également souhaité introduire sans étude préalable un nouvel article qui visait à regrouper la fonction d'autorisation de contrôle des activités nucléaires de la SN avec les activités d'expertise et de recherche de l'IRSN. Fort heureusement, grâce à la mobilisation et aux nombreuses alertes de parlementaires de tous bords politiques et des acteurs de la filière elles-mêmes le texte final a écarté cette fusion. Il est essentiel de maintenir notre système dual face au changement climatique, l'urgence absolue et le renforcement de l'expertise, il faut au contraire augmenter si il a significativement les Budgets tant de l'IRSN que de l'ASN ne bradé pas la sûreté. Le texte laisse par contre la possibilité pour la SN de recruter des agents contractuels. Nous serons vigilants sur ce point qui pourrait mettre à mal l'indépendance de l'autorité. Autre point essentiel cette loi ne répond pas suffisamment aux enjeux d'une nécessaire adaptation des centrales aux impacts du dérèglement climatique, des prochaines décennies. Sur la question essentielle de l'eau dans un contexte de plus en plus difficile. Comment continuer à prélever plus de 26 milliards de mètres cubes d'eau par an. Tu as la part de l'eau consommée, le service des données études statistiques la fait passer du jour au lendemain, de 31% à 12%. Nous sommes passés de 72% d'eau évaporée à 22% cela interroge sur le sérieux de ces chiffres. ailleurs qu'en sera-t-il demain dans le cas d'une augmentation des températures de 4 degrés. Quid des centrales situées dans les zones vulnérables aux inondations. Le risque de submersion marine est un sujet central en matière de sûreté, sujet que vous refusez de prendre réellement en compte. Sur les autres points contournement des procédures environnementales et de participation du public détricotage du code de l'urbanisme. Autant de mesures dérogatoires que nous contestons. Vous en entendez un gain de temps, que l'on Conseil d'État lui-même ne peut estimer. Enfin, nous déplorons la réintroduction de la suspension des aides publiques à une organisation dont un membre s'introduit dans une centrale plutôt que de renforcer la sécurité des centrales, on préfère s'en prendre aux lanceurs d'alerte. Madame le Ministre, présenté cette relance comme une solution contre la crise climatique est un non-sens et va à rebours du consensus scientifique qui exige de réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Nous n'avons plus que 7 ans pour agir, alors que les éventuels nouveaux réacteurs ne verront pas le jour avant 2037 2037 au plus tôt. Nous refusons de donner un blanc-seing à cette relance sans nuance qui va être lourde de conséquences et engage les générations futures qui n'ont pas signé pour ce cadeau empoisonné. Planifions démocratiquement une sortie raisonnée et maîtrisée du nucléaire pensez avec les salariés et nos concitoyens. Pour l'ensemble de ces raisons, nous voterons contre ce texte issu de la CMP souvent. Merci Merci la parole est maintenant à Bernard bus pour le groupe du Rassemblement démocratique progressiste indépendant. Madame la présidente. Madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues si l'énergie nucléaire inquiète autant qu'elle fascine. Elle est aujourd'hui la première source de production d'électricité en France. Pourtant, au cours des dernières décennies, le développement du nucléaire a été délaissé. Il faut remonter 17 ans en arrière, le 5 janvier 2006 pour retrouver les dernières décisions importantes en la matière date à laquelle le président Jacques Chirac, annonça le lancement d'un prototype de réacteur nucléaire de 4ème génération qui devait entrer en service en 2020 le fameux EPR de Flamanville, ainsi que la création d'une autorité chargée de veiller à la sécurité nucléaire. L'ASN. Mais dans un contexte où la guerre en Ukraine et ses conséquences se mêle au dérèglement climatique. À l'heure où la décarbonation la transition et la souveraineté énergétique s'impose à tous. La relance du nucléaire en France doit redevenir une priorité. Je me réjouis donc que nous votions aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire conclusive sur ce projet de loi essentielle pour accélérer actualisé et dépoussiérer les procédures qui pour certaines d'entre elles datent de Mes chers collègues. Le texte sur lesquels nous sommes parvenus à trouver un accord est une première Pierre essentielle pour la relance du nucléaire civil et pour l'avenir de notre pays. Je crois même qu'il s'agit d'un texte majeur et cela pour 2 raisons. Un texte majeur sur le fond, d'abord dans l'esprit du discours prononcé par le président Emmanuel Macron à Belfort en février 2022, qui traduit une ambition forte, je le cite faire en 30 ans de la France, le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles et renforcer notre indépendance énergétique industrielle dans l'exemplarité climatique en quelque sorte, reprendre en main notre destin énergétique et donc industriel. Un projet de loi également important pour notre assemblée, puisqu'il s'agit d'un des premiers textes de la législature déposé en première lecture au Sénat. voté les conclusions de la commission mixte paritaire, c'est voter des mesures principales du projet de loi, à savoir simplifier et accélérer la mise en oeuvre des projets de construction de 14 nouveaux réacteurs électronucléaires en France d'ici 2050 et clarifier les dispositions de sécurité des centrales nucléaires vieillissantes. Mais le texte que nous votons aujourd'hui et surtout le fruit d'un travail de compromis auquel j'ai participé dont je me réjouis. Les grands équilibres trouvés lors de la navette parlementaire n'ont pas été modifiés et mieux encore, le texte a été enrichi par de nombreux apports du Sénat. Je pense aux mesures liées à l'actualisation de la planification écologique aux objectifs ambitieux fixés en matière d'hydrogène et de recherche et de développement nucléaire. Je pense également au renforcement de la sécurité juridique des procédures à l'image de la consolidation des garanties en cas d'expropriation et à la procédure de régularisation des contentieux et à la clause de revoyure pour favoriser l'enfouissement des infrastructures du réseau de transport d'électricité. Par ailleurs, je tiens également insisté sur le renforcement de la sûreté et de la sécurité nucléaire en intégrant, par exemple la résilience au dérèglement climatique dans la démonstration de sûreté des réacteurs au stade de l'autorisation comme du réexamen sans oublier la consolidation des attributions et les moyens de l'Autorité de sûreté nucléaire. À ce propos, je tiens à souligner le fait que l'amendement que j'avais défendue au nom du groupe RDPI portant sur la parité au sein du collège de l'ASN a été adopté est maintenu dans la version finale du texte sur lequel nous allons voter. De plus je tiens bien évidemment a salué le compromis trouvé en CMP s'agissant du zéro artificialisation nette sur un tel sujet ô combien sensible pour les élus locaux et par conséquent pour notre assemblée, il me semble que l'exemption des réacteurs du décompte de l'objectif than pour les collectivités territoriales est une chose positive dans la mesure où ces surfaces ne seront pas comptabilisés dans le crédit des communes et des régions d'appartenance mais fort bel et bien l'objet d'un comté à part dans une loi qui devra déterminer les modalités dérogatoires avant le 1er janvier 2024. Autant de raisons pour lesquelles le groupe RDPI votera ce texte, fruit d'un compromis qui symbolise le travail que l'on peut trouver et faire des consensus bâtir des solutions dans l'intérêt général du pays. Nous attendons désormais avec impatience la future loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat qui fixera la trajectoire énergétique de la France par source d'énergie sur la période 2028 2033 qui promet à n'en pas douter d'intenses débats et d'être une étape décisive pour assurer la souveraineté de notre pays. Je vous remercie. La parole est maintenant à Franck Montaugé pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues. Au terme de six années pendant lesquelles vos gouvernements successifs ont minimisé le rôle central de l'énergie dans la transformation profonde de notre pays, nous voilà avec cette loi de relance du nucléaire, situation de poser un second acte après celui relatif aux ENR. Un déni total de la logique la plus élémentaire et qui aurait nécessité que nous actualisons d'abord la stratégie nationale bas-carbone que nous discutions ensuite la loi de programmation énergie climat et comme. En En soit déduite la programmation pluriannuelle de l'énergie, la CMP propose d'actualiser la PPE en vigueur pour le nucléaire alors qu'il était apparu inutile oh emporter dit procéder suite au texte sur l'accélération des ENR comme prenne qui pourra. Le projet de fusion ASN IRSN au détour de l'amendement introduit après la discussion du texte au Sénat nous a confirmé l'intention de passage en force du gouvernement et accessoirement le peu de considération qui à Sienne et de la chambre haute. Le groupe socialiste a pris le temps de l'écoute des personnels de l'IRSN. Dont je tiens ici à saluer le sens des responsabilités et du devoir. Potentiellement toute évolution de la doctrine et de l'organisation française en matière de sûreté nucléaire doit être documenté discuté avec la représentation nationale et les acteurs de la société civile, c'est pour aller dans ce sens que notre groupe a proposé à la CMP un amendement visant à confier à l'Opecst une étude sur l'organisation des missions de la de l'ASN, La présidente de la commission des affaires économiques du Sénat a donné suite à cet amendement sous la forme d'une saisine officielle de l'organisme par le Sénat, c'est une bonne chose et nous nous en réjouissons. Cependant, nous n'avons pas voté l'amendement relatifs au recrutement par l'ASN de contrat privé.

La prise en compte de l'artificialisation des sols engendrée par les nouvelles installations nucléaires sur Lausanne. Des territoires concernés a bien entendu retenu notre attention. La solution consistant à renvoyer le traitement de cette question une loi spécifique prise au plus tard le 1er janvier 2024 nous paraît relever d'un pis-aller hein à part seule ne résoudra rien l'équité doit ici prévaloir et l'ensemble du territoire national doit prendre en compte l'impact des projets nationaux, la solution technique est simple, faut-il un peu de courage politique pour la mettre à oeuvre nous en reparlerons. Au final, ce texte permettra de gagner une année ou un peu plus après en avoir perdu cinq et pour des installations industrielles dans la durée de vie pourrait être de 60 ans ou plus. Cela relativise la portée des mesures proposées, mais nous sommes globalement favorable à des, à ces dispositions de simplification qui faciliteront le travail des opérateurs EDF production RTE et les filières industrielles concernées, tout en respectant les territoires et les collectivités locales directement concernées. De nombreux autres points touchant au nucléaire reste cependant en suspens qui conditionneront la réussite finale du plan engagé. Quelques exemples du côté de l'appareil industriel maîtrise technologique des EPR de coût de financement des programmes compétence des techniques nécessaires. Attractivité des métiers qui renvoie au statut et Cadre d'emplois organisation du groupe EDF. Et du côté des consommateurs, suppression de la reine et réforme structurelle des tarifs permettant la vente au plus près du coût moyen pondéré du mix électrique électrique élargissement des tarifs réglementés pour protéger les artisans, les TPE et les PME PME PMI, les collectivités locales dispositions que devient que viennent de voter l'Assemblée nationale et donc j'espère que nous débattrons ici prochainement. Tous ces sujets sont dans le Champ de responsabilité du gouvernement et de votre ministère à Madame dont nous attendons beaucoup dans l'intérêt du pays. En conclusion, ce texte sera utile. Malgré sa portée relative et notre groupe votera donc favorablement les conclusions de la CMP. Je vous remercie. La parole est maintenant à Fabien Gay pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Notre groupe est favorable à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires à côté du développement des énergies renouvelables pour acquérir une indépendance énergétique qu'il ne faut pas confondre avec souveraineté énergétique. Si notre groupe il y est favorable. C'est parce que la crise climatique nous impose de combiner les énergies de continuer à décarboner à un coût maîtrisé pour rendre les prix supportable pour tous les usagers résidentiels mais aussi les collectivités, les entreprises et comme il n'y a pas d'énergies propres car toute activité humaine n'aime pas que sur la nature c'est bien la combinaison des différents moyens de production d'énergie qui nous permettra une indépendance sachant que pour la souveraineté, il nous faudrait nous extraire de l'uranium et arrêté les livraisons du Kazakhstan et du Niger. Ce qui est impossible forme d'en venir au fond je voudrais Madame la Ministre vous dire un agacement. Au lendemain du vote en première lecture de ce projet de loi au Sénat. Vous avez annoncé que le projet de fusion entre l'IRSN et l'ASN seraient introduits dans la navette parlementaire. Au-delà des questions de fond de l'importance d'une séparation entre l'expertise scientifique et les activités de contrôle, il y a un sujet de forme. Pensez-vous respecter le Sénat en agissant de la sorte. Sans parler des salariés de leurs syndicats, qui ont découvert ce projet dans la presse, heureusement. L'affaire a été enterré à l'Assemblée nationale et pour cette fois votre coup de force ne passera pas. Mais nous resterons attentifs pour en venir au texte lui-même telle que nous l'examinons aujourd'hui le problème est le même qu'en première lecture vous segmenter le sujet sans donner quatre général sans évoquer le financement, EDF, la reine et la régulation. Pour vous, le seul problème, ce sont les délais administratifs. C'est comme si un constructeur automobile commencer par construire les enjoliveurs sans évoquer le moteur et l'habitacle. Un enjoliveur c'est joli mais ça ne fait pas rouler une voiture comme les délais administratifs ne construiront pas de centrale nucléaire. Tout d'abord le moteur du nucléaire c'est son entreprise historique EDF. Mais qui est amputée, aujourd'hui de 60 milliards de dettes, dont 8 sont issus de la reine plus que vous avez décidé seul avant que le Parlement ne donne son accord en août. Comment le groupe que vous êtes en train de ré-étatiser pourra-t-il investir plusieurs dizaines de milliards d'euros dans 8 nouveaux EPR avec un tel endettement, vous allez devoir céder des actifs comme Dalkia ou une partie d'Enedis mais où aller chercher le reste dans le privé mais qui Total énergies ne se dit pas intéresser les investisseurs privés et étrangers dans ce cas. Madame la ministre, il serait bon que la représentation nationale soit impliqué pour que nous donnions notre avis la question du moteur. Il y a été posée. Parlons maintenant de l'habitacle et du volant, à savoir la régulation. Vous voulez continuer la reine au-delà de 2025 dans le but escompté était de faire investir les alternatifs dans la production, c'est raté. Car aucun ne l'a fait, sauf Total énergies Angie tous les autres profitent du système et revendent sur les marchés pour leur propre bénéfice d'ailleurs avec ma collègue Dominique Estrosi Sassone nous rendrons prochainement un rapport sur ces abus qui ont eu lieu en 2022. Ça vous en révéler les conclusions, je peux déjà vous dire ce qu'il y a dans la presse, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus qui pèse sur le portefeuille d'EDF tout en raquettant les Français. Mais venons en même temps au marché européen, au principe du coût marginal qui lie le prix du gaz à celui de l'électricité c'est une invention de Marcel Boiteux. Qui s'entendent sur un territoire national mais qui une RB ration sur le marché européen la réformette que vous venez d'ailleurs d'adopter. Loin de s'en défaire continuera de favoriser l'industrie allemande à notre détriment. Et comme la demande de gaz repartira à la hausse avec l'industrie chinois cet été au moment même où vous mettrait fin au bouclier tarifaire aux tarifs réglementés du gaz. La facture sera lourde pour tous les usagers. Enfin. Dernier point Madame la Ministre pour que soit une belle voiture comme de belles centrales nucléaires, il faut des salariés bien qualifiés bien rémunérés. Hé bien protégé alors que votre gouvernement ne vient de casser le statut et les retraites des IEG que nous tenions de Marcel Paul, sans un mot de votre part. Comment comptez-vous redonner de l'attractivité à une filière qui souffre depuis 15 ans en partie du fait de l'inaction des pouvoirs politiques. puisque vous dites 100.000 recrues du chaudronnier à l'ingénieur. Vous allez donner envie à une génération de sauver investir notamment dans le nucléaire, là encore pas de réponse. Votre texte n'aborde aucune de ces questions structurelles qui pourtant indispensable aux objectifs que vous Lisieux a signé c'est pour toutes ces raisons que notre groupe s'abstiendra. Je vous remercie.

le 6 mars 1974, avait l'annonce du plan Messmer la France de l'énergie entré dans une nouvelle ère. Une ère ou souveraineté et indépendance économique rimer avec nucléaire et ambition. Une aire. Où les sphères, scientifiques, industriels et politiques ne faisait comme au service de l'intérêt national. Devenu grenier électrons d'origine nucléaire de l'Europe. Notre pays s'est progressivement imposé durant la fin du XXe siècle comme un acteur de 1er plan pour bâtir l'indépendance énergétique de la France et de l'Europe. Fort de nos certitudes. Nous ne vont pas su profiter de cette dynamique et nous remettre en question. Nous n'avons pas pris les décisions stratégiques qui s'imposaient pour continuer de développer notre capacité de production d'électricité nucléaire. Affaiblissement de la volonté politique sous les coups de boutoir de certains ayatollahs verts, absence de construction de nouveaux réacteurs tarissement des filières de formation du secteur. La déliquescence de l'entre-. Filière nucléaire était aussi manifeste que notre aveuglement. Pour nous en rendre compte. fait la fermeture de Fessenheim et la crise énergétique durant laquelle la France est devenue importatrice nette d'électricité en lieu et place de son rôle traditionnel exportateur notre myopie a été révélé au grand jour. À l'heure. Où nous avions plus que jamais besoin d'une politique nucléaire robuste efficience l'attentisme le court-termisme, de nos dirigeants ont déstabilisé grandement l'ensemble du secteur et de son acteur principal et phare EDF. Je crois que sur tous ces bancs. Nous devons saluer le sursaut que constitue le discours de Belfort et plus encore à la décision prise par le président de la République de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Cette relance est décisive pour la une. Défendant ce stratégique de notre pays et dans ton souveraineté énergétique. Ce projet de loi et donc le 1er pas à saluer pour rompre avec le déclin qui était celui de la production d'électricité d'origine nucléaire. Avec le groupe Union centriste. Nous saluons. Les compromis qui ont été trouvées afin de faire aboutir ce texte il est vital pour traduire a conclu concrètement la relance de l'énergie nucléaire dans notre pays.

Le Sénat. A je crois pris toute sa part dans la construction d'un texte intelligent en faisant fi de tout dogmatisme et de croyances dépourvue de fondement scientifique. L'abrogation des limites de production d'électricité d'origine nucléaire et du plafonnement de la part de celles-ci dans notre mix énergétique est à ce titre signal fort, adressé au secteur. La non-comptabilisation. Des nouveaux réacteurs et des infrastructures afférentes dans le Sam est également déterminante. En le fléchage du bénéfice de la taxe d'aménagement perçu sur les Rather vers les collectivités sera clé. Elle facilitera l'accessibilité local des nouveaux réacteurs et permettra d'embarquer l'ensemble des acteurs dans cette relance du nucléaire. Mes chers collègues. Je crois que nous avons agi en responsabilité pour améliorer un texte technique qui nécessiter manifestement des ajustements. À ce titre. Je tiens à saluer. Les efforts conjoints ne rapporteur des 2 commissions Daniel Gabri Remiller. Et Pascale Martin, de la présidente Sophie Primas et du président et Jean-François Longeot pour enrichir ce texte de loi. Je crois. Qu'il faut désormais poursuivre cette dynamique accélérer la formation des personnels et faire confiance aux acteurs scientifiques, industriels et administratifs mobilisés pour ce projet. C'est tout ce que nous attendons de la loi de programmation pluri-annulaire de l'énergie, que nous examinerons à l'Automne. Plus qu'un nouveau plan Messmer, j'espère qu'avec ces deux textes nous tirerons les enseignements de nos erreurs passées afin de doter notre pays d'une véritable ambition nucléaire et d'une vision stratégique pour les années à venir. Sans oublier. Je crois que Fabien Gay là dit au début, moi je le dis à la fête. Sans oublier la nécessité de continuer à travailler sur le mix énergétique. Je vous remercie. Merci. Alors sur ce projet de loi. Tels qu'ils résultent de la commission mixte paritaire. Je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les. J'ai de du scrutin va être annoncé dans le palais.

Le scrutin est ouvert.

ouvert. Ça ne demande à voter. Le scrutin est clos. Votants 343 exprimés, 328 pour 315 contre 13 le projet de loi et donc à deux. allons. Maintenant étudier le texte suivant. Et. Si les si tous les protagonistes sont là je vois la présidente de la commission d'affaires sociales et là je crois qu'. Un ministre n'est pas loin. La rapporteure elle là aussi. Non non mais, prenez votre temps. Madame la présidente. Gardez. Votre successeur attends patiemment.

Nous avons le ministre-, la présidente et la rapporteure. Nous allons donc pouvoir étudier les conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé et la parole est d'abord Madame la rapporteure Corinne Imbert.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues. La commission mixte paritaire est parvenue le 6 avril dernier à un texte commun sur la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Cet aboutissement en toute franchise n'était pas gagné d'avance. Nos deux chambres divergeaient sur plusieurs points essentiels. Il faut réjouir. Il faut se réjouir que l'approche équilibrée défendue par le Sénat sur ce texte et finalement été retenu rendant possible cet accord. Permettez-moi d'exposer brièvement les nombreux articles sur lesquels tout de même les textes adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat se rejoignaient déjà largement et que l'accord de CMP avalise. Il s'agit pour l'essentiel de mesures d'ajustement permettant de faciliter le parcours du patient et de valoriser les compétences des professionnels de santé. Les articles 4 et 4 bis prévoit ainsi de nouvelles compétences attribuées aux assistants dentaires de niveau 2 et un encadrement de leur nombre dans un même lieu d'exercice. L'article 4 sex IS réforme le diplôme de préparateur en pharmacie et reconnaît à l'initiative du Sénat la compétence des préparateurs pour administrer des vaccins listés par arrêté. L'article IV. Cette pièce a modifie les conditions de diplôme de la profession de diététiciens. Tandis que l'article IV des Siess reconnaît les assistants de régulation médicale comme profession de santé afin de renforcer l'attractivité de ce métier. Enfin, le texte qui vous est présenté aujourd'hui retient également l'article 4 quater des siestes ajouté par le Sénat. Les dispositions issu de la CMP contraignent le pouvoir réglementaire a publié annuellement la liste des tests rapides d'orientation diagnostique les TROD pouvant être utilisé par les professionnels de santé s'agit d'éviter une inertie quant à l'autorisation des tests innovants. Sur 3 autres points nos deux assemblées avaient adopté des textes plus éloignés. Toutefois le texte issu de la CMP préserve largement les apports du Sénat. En 1er lieu la CMP a validé la suppression, la suppression des dispositions relatives à l'engagement territorial des médecins. Celle-ci. Avait été écartée par la commission des affaires sociales du Sénat, au motif qu'elles interfèrerait avec les négociations en cours de la nouvelle convention médicale et contribué inutilement ahan dégradé le climat. Merci Monsieur le Ministre de votre écoute. À l'article 4 terre la CMP a adopté les dispositions permettant aux sages-femmes et aux infirmiers de concourir à la permanence des soins ambulatoires que nous avions soutenue. Elle a également choisi de maintenir la notion de responsabilité collective des praticiens en la matière qui avait été supprimé par le Sénat. Celle-ci inquiète les professions de santé alors que le gouvernement peine toujours à décrire les conséquences qu'elle emporte. Je ne peux que l'invité à clarifier rapidement les choses en confirmant que cette disposition ne modifie pas l'économie générale de la permanence des soins. Enfin aux articles 1er et de la CMP a suivi la voie tracée par le Sénat en réservant en ville l'accès Direct aux infirmiers en pratique avancée hé oh ma soeur kinésithérapeutes exerçant au sein des structures d'exercice coordonné. Il est plus intégrée, à savoir les maisons de santé. Pluri-pluriprofessionnelles. Les centres de santé et des équipes de soins primaires au spécialisé. Le Sénat avait considéré qu'il n'était pas souhaitable à ce stade de faire de l'appartenance à une communauté professionnelle territoriale de santé une CPTS une condition suffisante à l'accès Direct. Celle-ci ne permet pas de faire la preuve d'une véritable coordination entre professionnels. Les récentes annonces du gouvernement qui vise à rendre obligatoire l'appartenance une CPTS pour l'ensemble des professionnels conventionné tente d'ailleurs à nous donner raison. Le texte issu de la CMP prévoit l'expérimentation d'un accès Direct en CPTS pour cinq ans deuil dans 6 départements, dont 2 départements d'outre-mer. Nous souhaitons que le gouvernement prenne le temps d'en évaluer les effets de ces les prochaines années avant toute nouvelle évolution législative. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est le fruit d'un véritable travail d'échanges. Nous nous réjouissons que le Sénat et pu faire entendre sa voix sur des sujets importants qui ont ces derniers mois, nourri des tensions entre professionnels de santé. La CMP a largement retenue de l'approche raisonnable que nous avions défendu un amendement du gouvernement vous proposera de généraliser à notre invitation. Une nouvelle compétence des pharmaciens biologistes. C'est pourquoi je vous invite à adopter le texte qui vous est soumis ainsi modifié, je vous remercie. Merci madame la rapporteure. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Au coeur de la proposition de loi dont l'ultime étape de l'examen parlementaire nous réunit aujourd'hui, il y a une ambition. Celle d'accélérer le décloisonnement notre système de santé. Ce texte comporte de nombreuses dispositions qui sont autant de briques importantes du chantier de la refondation de notre système de santé dans les grandes lignes ont été fixées par le président de la République et sur lequel je me suis engagé avec constance et détermination. Depuis mon arrivée au ministère de la Santé. Cette refondation est basée sur de grands principes directeurs que j'ai rappelé devant les parties prenantes et les élus les réunis lors d'une rencontre plénière du Conseil national de la refondation en santé la semaine dernière. Une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs du système de santé entre les différentes professions, en ville comme à l'hôpital. C'est le principe de l'équipe. Une adaptation territoriale de notre politique de santé. Ce n'est pas à vous sénateur que je vais apprendre que s'il faut penser globalement il faut agir localement. Le principe du dialogue qui est aussi bien la méthode qui nous a permis de faire aboutir ce texte que ce qui permettra à tous les acteurs de la santé, de travailler ensemble au sein de collectifs professionnels renforcée. Et puis finalement l'éthique l'éthique d'un système de santé qui évolue pour toujours mieux répondre aux besoins de nos concitoyens et lutter contre les inégalités d'accès aux soins. Je sais que ses convictions, ses valeurs sont largement partagées à travers les bancs de cet hémicycle et nos débats en ont témoigné. Le Sénat a pu pleinement y faire entendre sa voix. Il y a eu des divergences, certes, mais nous avons tous toujours eu collectivement à coeur d'avancer ensemble. Nous sommes à présent arriver au stade de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire. Je me réjouis que celle-ci ait été conclusive et je tiens à remercier la présidente de la Commission, Catherine Deroche la rapporteure Corinne Imbert et dès l'ensemble des membres de la CMP dans les 2 assemblées qui ont travaillé dans un esprit constructif. Ensemble, nous avançons sur le chemin d'un système de santé ou chaque professionnel trouve sa place ou le cadre d'une collaboration rénovée et renforcée entre les métiers, permet de mieux répondre aux besoins de nos concitoyens et aux tensions auxquelles fait face, notre système de santé. En effet, mesdames vous avez messieurs les sénateurs. Si notre système de santé est mis à rude épreuve ces dernières années, c'est en grande partie lié au sujet de démographie et d'attractivité des professions de santé, de perte de sens des professionnels de fuite vers deux mais d'autres métiers et de crise des vocations, en particulier chez nos jeunes soignants qui s'il porte l'avenir du système de santé sur leurs épaules n'entendent plus exercer comme autrefois. Et c'est tout à fait légitime. Nous devons comprendre et nous devons surtout répondre à ces nouvelles aspirations, de recherche de qualité de vie et de perspectives d'évolution de recherche d'opportunités pour s'inscrire dans des projets des collectifs professionnels. Il faut investir durablement et avec une méthode dans les métiers de la santé pour maintenir nos forces vives, assurer leur équilibre professionnel et inciter les plus jeunes à les rejoindre sans jamais perdre de vue l'impératif de sécurité et de qualité des soins. Pour renforcer, sécuriser nos effectifs à long terme nous avons supprimer le numerus clausus est ainsi corriger une erreur ici de choix politiques d'un autre temps autour d'un grand pacte avec les régions que nous allons poursuivre et renforcer. Nous avons déjà permis de créer 5000 nouvelles places en formation infirmière 4000 en formation, aide soignante. Si ces nouvelles places sont pourvus. Il faut nous en réjouir. La formation en soins infirmiers fait partie des formations les plus recherchés sur Parcoursup. Plus de 100.000 lycéens la choisissent parmi leurs 3 premiers voeux. Et nous avons ailleurs. D'ailleurs diversifiées enrichi les voies d'entrée en formation paramédicale notamment par l'apprentissage les parcours réussi tout lavé. Ces nouvelles places, ce sont autant d'étudiants que nous accompagnement pour arriver au bout de leur cursus et décrocher leur diplôme. Préparer l'avenir ne dispense toutefois pas d'agir face à l'urgence, bien au contraire, c'est une action globale qu'il nous faut mener. L'urgence c'est d'arriver à mettre en adéquation aujourd'hui l'augmentation des besoins de santé des Français avec une offre de soins qui se raréfie. L'urgence de l'accès aux soins et là notamment le visage des quelque 700.000 de nos concitoyens en affection de longue durée qui n'ont pas accès à un médecin traitant une équipe traitante. Nous avons pris l'engagement que chacune et chacun d'entre eux soit suivi par un praticien ou une équipe traitante et ce d'ici la fin de l'année. Cette proposition de loi dont Stéphanie Rist est à l'origine met en place des outils indispensables pour poursuivre dans ce chemin. Au delà de sécuriser le renforcement de nos effectifs dans le temps long, nous devons mobiliser tous les leviers nous permettant de gagner immédiatement de l'efficacité du temps médical pour nos soignants au service des patients. Ainsi pour nos soignants et ce que nous formons cette proposition de loi permet de rénover leur cadre d'exercice et d'avancer sur un nécessaire repositionnement des professionnels dans le système. D'avancer dans la voie du renouvellement et de la diversité des pratiques de donner de nouvelles responsabilités et des perspectives de carrière à celles et ceux qui ont choisi de consacrer la vie aux autres. C'est un enjeu majeur d'attractivité et de fidélisation. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés grâce au levier que constitue la pratique avancée les partages de compétences et de délégation d'actes qui doivent se déployer dans des organisations territoriales collective et coordonnée autour du médecin. Je sais combien vous sénateur avait été attentif à ce point. Dans tous les cas d'accès Direct un masseur kinésithérapeute à un orthophoniste ou un infirmier en pratique avancée. Ah. Compte rendu des soins sera réalisée devra être systématiquement adressé au médecin traitant du patient est reporté dans son dossier médical partagé. Je veux ainsi prendre le temps ici d'assurer et de rassurer les inquiétudes légitimes de faire taire certaines allégations de mauvaise foi. Il n'y a jamais eu d'aucune manière la volonté de mettre de côté le médecin généraliste au contraire cette loi vient conforter et renforcer la place centrale du médecin généraliste traitant qui sera, et qui est le pivot autour duquel s'organisera cette coopération accrue entre les professionnels de santé. Je reviens à cette notion d'équipe traitante d'équipes soignantes qui est absolument fondamental, car c'est là que chacun dans son rôle pour apporter toute sa valeur ajoutée à la prise en charge des patients. Je pense aussi ici à la création du nouveau métier d'assistant dentaire de Nuvia ou de que permet ce texte. La présence d'un assistant à ses côtés, c'est près de 30% de temps gagné pour un chirurgien dentiste alors que l'accès à ces spécialités difficile dans de nombreux territoires. Tout cela est triplement gagnant gagnant pour les soignants qui sont mieux reconnus et gagne en autonomie et en compétence gagnant pour les médecins qui déchargée de certaines tâches ont plus de temps auprès des patients, gagnant pour les Français qui accèdent plus facilement aux soins. L'équipe toutes ses équipes locales, la grande équipe que doit être la santé c'est le lieu de collaboration et c'est aussi le lieu du partage des responsabilités autour de la permanence des soins. Cette proposition de loi introduit le principe de responsabilité collective des professionnels de santé à la permanence des soins, tant en établissements de santé qu'en ville. Je cite littéralement cette nouvelle disposition qui prévoit que les établissements de santé et les médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et infirmiers sont responsables collectivement de la permanence des soins. Je me félicite de l'inscription dans la loi de cette mesure, qui doit nous permettent de garantir aux patients un accès aux soins non programmés à toute heure du jour et de la nuit en répartition cet effort entre toutes les structures et tous les médecins d'un territoire. Aussi le règlement arbitral qui vient d'être publié entre les médecins et l'assurance maladie permet d'avancer sur plusieurs dispositions importantes pour faciliter cet accès territorial aux soins non programmés, avec notamment la pérennisation de la majoration de 15 euros pour les actes adressés par le service d'accès aux soins, ainsi que la rémunération au taux horaire de 100 euros des médecins libéraux régulateurs. J'en profite pour dire ici mon attachement à une reprise du dialogue avec les syndicats de médecins. Car c'est bien le sens des dispositions équilibré de cette proposition de loi de convaincre sans contraindre de créer des conditions d'une responsabilité partagée par la confiance aux professionnels de santé. La confiance et le dialogue plutôt que des mesures de coercition auquel je redis que je suis clairement défavorable qui ne serait que le vecteur d'une cristallisation des frustrations et de rigidité mortifère pour notre système de santé. Je serai assez attentif à ce que les partenaires conventionnels puisse dans les prochaines semaines échangé sur les modalités, le calendrier les axes pour une possible reprise des négociations pour aller au-delà de ce règlement arbitral dans la valorisation de cet engagement territorial. Cette proposition de loi entérine une autre mesure clé dans le déploiement de ses services d'accès aux soins dont la généralisation est un enjeu fondamental pour appuyer la réorganisation de l'accès à une offre de soins non programmés, adaptée aux besoins des Français. La reconnaissance des assistants de régulation médicale comme profession de santé à part entière et la première étape des efforts que nous poursuivons pour mieux valoriser ce métier essentiel. La responsabilité partagée autour de la permanence des soins. Le service d'accès aux soins, la valorisation des professionnels qui participent. C'est tout cela qui nous permettra d'accomplir l'objectif fixé par le président de la République et qui nous mobilise tous d'arriver à désengorger nos urgences d'ici la fin de l'année 2024. J'ai évoqué combien la confiance aux professionnels de santé la revendre, rénovation des carrières était essentielle pour l'attractivité de ces professions et pour les adapter aux évolutions d'un système de santé moderne. C'est également le sens de la refonte du métier infirmier que nous menons et dont nous aurons prochainement l'occasion d'annoncer les modalités pratiques très prochainement. Ces élargissements de compétences nous faisons bien sûr pour les professionnels mais toujours dans l'objectif de faciliter le parcours des patients et de leur changer la vie au quotidien. Derrière chaque article de loi derrière chaque expérimentation que nous mettons en place derrière chaque décret il y a bien des changements concrets dans la vie de nos concitoyens avec cette proposition de loi nous permettons donc aux patients atteints de maladies chroniques comme les diabétiques de renouveler leur ordonnance auprès du pharmacien pour une durée allant jusqu'à 3 mois dans l'attente de leur prochain rendez-vous médical à celles et ceux qui ont besoin de lunettes ou de lentilles de pouvoir faire adapter leurs prescriptions directement par l'opticien lunetier après accord écrit du praticien prescripteurs. À toutes celles et ceux qui souffrent de plaies chroniques. D'être pris en charge directement par un infirmier ou infirmière. Des professionnels de santé de proximité présent dans tous nos territoires. Nous permettons à un meilleur accès aux actes de prévention c'est toi multiplié garantit l'accès aux opportunités de vaccination qui nous protège tous en reconnaissant le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques des préparateurs en pharmacie et en permettant de manière pérenne détendre leurs compétences pour administrer certains vaccins sous la supervision d'un pharmacien. En complément de ce que nous avons déjà permis pour les infirmiers pharmaciens sages-femmes à l'occasion de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Tous ces professionnels permettent un recours plus large à la vaccination. Ce texte autorise à titre expérimental pour l'instant et je l'espère de façon définitive après. Le vote de l'amendement que j'aurai l'honneur de vous présenter autorise les biologistes a pratiqué des prélèvements dans le cas du dépistage du cancer du col de l'utérus. Un cancer dont je redis ici que nous pouvons de manière réaliste envisager d'éradication à moyen terme, grâce à la vaccination généralisée proposé à tous les élèves de 5ème contre le papillomavirus dès la rentrée prochaine. Toutes ces situations du quotidien que nous facilitons c'est la petite histoire qui permet la grande. Celle de nous projeter collectivement dans une vision systémique de la réponse aux besoins de santé où chacun à sa juste place sera le plus efficace et le plus utile. Aussi mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois, pour votre engagement. Depuis le mois d'octobre dernier sur cette loi importante donc je me réjouis avec vous qu'un texte de compromis juste et équilibré soit adoptée. Je sais pouvoir compter sur l'engagement et la compétence des sénateurs pour continuer ensemble d'avancer sur ce chemin de la refondation de notre système de santé. De nouvelles échéances législatives devrait nous réunir très prochainement autour de cet objectif. Encore une fois et toujours au service de la santé de nos concitoyens. Je vous remercie. Bien, je vous rappelle que le Sénat étant appelés à se prononcer avant l'assemblée nationale nous statueront en à la fin sur un seul vote mais auparavant nous allons examiner les 2 amendements du gouvernement, puis dans les explications de vote, des collègues, Monsieur le Ministre, vous avez la parole pour vos amendements. Oui madame la présidente, mesdames et messieurs les. Sénateurs l'amendement à l'article 2 est un pur amendements rédactionnels. Il corrige une erreur de référence dans l'article 2 et plus précisément au 6ème alinéa. Oui, étant donné la nature du premier vous pouvez présenter le deuxième. Merci madame la présidente. L'amendement de l'article IV vise en lien avec les positions exprimées par les rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ah généraliser toute de suite la passer banalité pour les pharmaciens biologistes de dépister par frottis le cancer du col de l'utérus. Les pharmaciens biologistes sont formés pour réaliser ce geste et nous estimons ne pas avoir besoin de passer par une expérimentation. Je vous propose ainsi d'offrir une nouvelle possibilité d'accès à la santé, en particulier à la prévention à nos concitoyens. Merci madame la présidente. L'article 4 terre des siestes autorise à titre expérimental, les pharmaciens biologistes a réalisé des prélèvements servi co-vaginaux dans le cas du dépistage du col du cancer du col de de l'utérus. Je précise que ça se fait en laboratoire d'analyses pas dans les pas dans les pharmacies d'officine. Voilà je, je préfère le le dire si les pharmaciens biologistes peuvent réaliser. L'ensemble des actes de biologie médicale. La réalisation des frottis du col de l'utérus. L'heure est aujourd'hui pas permise car il s'agit d'un examen référencé comme sitôt pathologique cet amendement va donc plus loin et propose de prévoir définitivement leur. De reconnaître leurs compétences. C'est une généralisation de bon sens que nous avions appelé de nos voeux de l'examen de la commission car pharmaciens et médecins biologistes poursuivent une formation identique est exactement le même cursus cette spécialisation la reconnaissance logique de la compétence des pharmaciens biologistes pour ce prélèvement permettra d'accroître les efforts de prévention déployés dans la lutte contre ce cancer, donc je vous le redis, la commission vous le savez, mes chers collègues, des affaires ça Affaires sociales n'ayant pas pu se se réunir, c'est un avis Je vais donc s'il n'y a pas de d'explication de vote sur cet amendement les mettre aux voix je pense l'amendement numéro 2 amendements d'ActionAid, pas d'opposition. Il est adopté. Quant à l'amendement numéro 1 qui a reçu un avis favorable de la rapporteure. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Nous passons maintenant aux explications de vote, à raison d'un orateur par groupe et nous commençons par madame la présidente de. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Sur cette proposition de loi aboutir à une CMP conclusive n'était pas acquis. Notre fil rouge était le maintien des mesures adoptées par notre assemblée qui visait à faciliter le parcours du patient et à valoriser les compétences des professionnels de santé lors de l'examen de ce texte en première lecture nous avions en effet trouver un équilibre fragile. Grâce au travail de notre rapporteure Corinne Imbert. Nous avions fait en sorte de réduire les tensions parmi les professionnels de santé de garantir la sécurité des soins et de préserver le rôle du médecin dans le suivi du patient. Nous avions à ce titre alerter le gouvernement sur le fait que ce texte faisait l'effet d'un chiffon rouge dans le cadre des négociations conventionnelles et Monsieur le Ministre, le gouvernement doit être conscient des craintes des médecins par rapport à l'exercice futur de leur métier, notamment en ce qui concerne la place du médecin généraliste avec le manque actuel de médecins nous faisons trop supporter à ceux qui sont en exercice qui voient de nombreux patients et puis pour certains prennent des gardes assure la permanence des soins et qui, sans remettre en cause la qualité de leur travail se sentent parfois considérés comme des boucs émissaires. Nous avions tenu compte de ces paramètres pour bâtir un texte devant répondre aux fortes attentes de la part des professions paramédicales, mais également prendre en compte ces inquiétudes. Permettez-moi de revenir sur 2 points le 1er concerne le contrat d'engagement territorial dans un objectif d'apaisement avec les professionnels de santé, le Sénat a supprimé les dispositions relatives à l'engagement territorial des médecins. Nous avions jugé que celle-ci interféraient inutilement, avec les négociations en cours de la convention médicale et-on détérioré le climat le contrat d'engagement territorial proposées par la Caisse nationale d'assurance maladie a d'ailleurs été largement rejetée. Quelques semaines plus tard. La suppression de l'article 4 quater, qui consacrait les la législative Mons ce principe d'un engagement est donc maintenu dans le texte de la CMP. Le second sujet porte sur les communautés professionnelles territoriales de santé les CPTS si le Sénat a validé le principe d'un accès Direct aux infirmiers en pratique avancée. Oh ma soeur qui n'hésitent thérapeute aux orthophonistes. Il a toutefois souhaité le réserver. S'agissant des infirmiers et des masseurs kinésithérapeutes aux structures d'exercice coordonné les plus intégrée. Comme l'a justement souligné Corinne Imbert. PTS ne sont pas des structures de soins. Elles font de la coordination elles organisent les soins certes mais cette corne. Ordination elle-même très disparates selon les territoires. Le texte de la CMP Reuters donc les CPTS du périmètre de l'accès Direct. Il maintient cependant une expérimentation pour 5 ans dans 6 départements, dont 2 d'outre-mer visant à autoriser les IPA à prendre en charge directement des patients dans le cadre de ces La prise en charge directe. Des patients par les IPA. Or ces territoires désespérément assure ainsi autorisée dans les établissements de santé et dans le cas de structures de soins primaires de maisons de santé pluri-professionnelles. Une parenthèse, Monsieur le Ministre, lors de l'examen de la LFSS 2022 nous avions voté des expérimentations d'accès Direct qui doit débuter au mois de juin dernier mais les dispositions n'ont jamais été prise donc il n'y a pas eu d'expérimentation. Par ailleurs, lorsque certains voient dans le CPTS, la solution au problème de pénurie médicale. Je fais référence à la PPL des groupes de la majorité gouvernementale déposée le 28 avril dernier, visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels. Nous considérons pour notre part qu'il ne suffit pas de décréter qu'il faut des CPTS sur tout le territoire pour régler les problèmes. Mais le débat aura lieu un autre moment, les syndicats de médecins nous avait également alerté des difficultés auxquelles il faisait face en raison de rendez-vous non honorés. Plusieurs enquêtes montrent que chaque semaine 6 à 10% des patients ne se présente pas à leur rendez-vous. Ce qui correspond à une perte de temps de consultation de près de 2h hebdomadaires pour le médecin, le Sénat avait ainsi adopté l'article 3 bis prévoyant une indemnisation des rendez-vous non honorés par les assurés. L'Arctique certes difficile peut-être d'expliquer, n'a pas été retenue par la CMP mais comme le demande l'Académie nationale de médecine et l'Ordre des médecins. Nous souhaitons que le gouvernement prenne des mesures afin de responsabiliser les patients sur cette défection. la CMP a donc maintenu en grande partie le texte adopté par le Sénat qui a retenu une approche équilibrée visant à fluidifier le parcours des patients à valoriser les compétences des professionnels de santé à garantir la sécurité des soins et à conserver le rôle et à conserver le rôle central du médecin dans la coordination et le suivi. C'est pourquoi notre groupe Les Républicains votera en faveur des conclusions de la CMP. Je vous remercie. Et la parole est maintenant à Daniel Chassain pour le groupe les indépendants. Madame Madame la présidente, madame la présidente de la commission même leurs porteur. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous partageons tous ce constat l'accès aux soins doit être améliorée dans notre pays beaucoup de territoires sont de désert médical et 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Il est aussi nécessaire d'améliorer la confiance envers les professionnels de santé. Toutefois la première mouture de la loi Rist ne répondait pas à cela, notamment pour les médecins et aurait désorganisé l'accès aux soins de 1er recours. En effet l'accès Direct aux IPA dans le cadre d'une CPTS étaient pour beaucoup de médecins un non-sens les CPTS. Sont chargés de prendre en charge les soins non programmés. Dans le cadre de plusieurs patients-t-elle alors que les IPA. Justement travailler en coordination autour d'une patiente par exemple dans une maison de santé avec un logiciel commun et surtout avec un médecin généraliste traitant et un protocole de coopération entre permettant ainsi à l'équipe médecin IPA de voir plus de patients. Les IPA en formation que j'ai rencontré d'ailleurs souhaitent travailler dans une MSP, en coordination avec le médecin et non dans le cas de de de ces BTS. Je voudrais donc Je voudrais donc féliciter madame le rapporteur qui a pendant la CMP pu faire modifier le texte qui permettra un fonctionnement pragmatique et utile l'encadre coordonnées d'un centre de santé d'une maison de santé. Nous saluons donc le retrait des. BTS du centre d'application de l'accès Direct aux IPA l'intervention du kiné. Auraient dû rester soumis à l'adressage préalable d'un médecin même si l'accès Direct dans la version issue de la CMP demeure limité à 8 séances par an et pense utile dans la plupart des cas mais là encore, nous saluons. Au moins le retrait des CPTS. Du Champ d'application du texte, nous avions lors de l'examen du texte en première lecture. Proposé d'autoriser des kinés intervenant n'est pas d'a renouveler une fois la prescription des séances avec l'avis du médecin traitant du médecin Co pour ce qui est de l'extension du Champ des prescriptions des infirmiers à la prise en charge des plaies et à la prescription d'examens complémentaires. Nous pensons toujours que celle-ci reduce accompagnée d'un avis préalable du médecin traitant en effet une plaie chronique peut être le signe d'une pathologie de votre prise en charge par un médecin comme trouble artères ou d'une mauvaise contention effectuerez fut une insuffisance veineuse, il en est de même de l'accès aux pédicures podologues podologue des patients diabétiques dont un besoin très fréquentes séances au delà d'une fois par semaine peut traduire la nécessité de consulter un médecin. Nous saluons. Le maintien dans le texte de la CMP des nouvelles compétences octroyées aux assistantes dentaires dit ne Dubau ainsi qu'aux opticiens l'accès Direct aux orthophonistes a été maintenu. Il nous étions favorable compte tenu du type de prise en charge très ciblée de ces professionnels sont amenés à faire et parce qu'il représente une profession formés au diagnostic je soutient largement la possibilité étendue de Roubaix, des prescriptions par le pharmacien pour le traitement des pathologies chroniques, ainsi que la possibilité de fac de vaccination sous la responsabilité sous leur responsabilité. Le maintien de l'expérimentation pour les pharmaciens biologistes. À pratiquer les prélèvements dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus amendement. Monsieur le ministre est une avancée selon moi. Nous aurions pu aller plus loin dans l'extension des compétences du pharmacien. J'avais d'ailleurs proposé qu'il puisse participer aux prescriptions dans le cap du sevrage sabbatique. Tabagique. De des examens sitôt. Bactériologique des urines et du traitement de ces sites en informant le médecin. Les professionnels de santé. Doivent travailler ensemble et en coordination et la place du médecin doit rester central dans le parcours de soin du patient quand le professionnel détient la compétence en matière diagnostiques et thérapeutiques. Et c'est sur quoi repose la sécurité quand de la prise en charge du patient que de la sécurité de l'activité des professionnels de santé. Monsieur le Ministre, cette proposition de loi a été heureusement amélioré par le Sénat et madame le rapporteur et elle permettra d'abord aux IPA et au médecin et à l'ensemble des professionnels de santé, et au médecin et à l'ensemble des professionnels de santé, de travailler ensemble en cohérence et en coordination dans les formes les plus intégrée d'exercice coordonné et ainsi gagner du temps pour moi plus de malades, le groupe les indépendants votera cette PPL ainsi améliorer. Bien. La parole va être maintenant Mélanie Vogel. Pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Merci. Oui madame la présidente. Monsieur le ministre, chers collègues. Madame la rapporteure avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre le temps de remercier les membres de la commission mixte paritaire pour leur travail. Les conclusions de cette commission comprennent des avancées que notre groupe avait porté néanmoins nous restons critiques sur d'autres points. Commençons par les avancées. Premièrement, je me réjouis que le texte prévoit l'accession diagnostic préalable et sans prescription ont masseurs-kinésithérapeutes. Cela facilite sans aucun doute la vie des citoyennes et des citoyens en facilitant la prise de rendez-vous dans la même veine, nous saluons l'accès Direct aux infirmières et infirmiers en pratique avancée. Leur permettent de prescrire des produits médicaux soumis à prescription médicale obligatoire est une mesure je crois utile. Toutefois, nous souhaitons rappeler que c'est le médecin qui coordonne les soins des patientes et des patients. Troisièmement, les pharmaciens et pharmaciennes biologiste pourront désormais dépister le cancer du col de l'utérus et nous le saluons. À côté de la vaccination, le dépistage et le moyen le plus efficace pour lutter contre ce cancer et moins de 60% des personnes concernées se font dépister. Sur le fond, cet amendement est donc très bien, j'ai juste pas compris pourquoi il était arrivé aujourd'hui le jour du vote, mais on va peut-être m'expliquer. En fait, nous saluons le fait que la commission mixte paritaire et supprimer l'article qui prévoyait des sanctions financières pour chaque rendez-vous médical manqué bien sûr, je l'avais dit la dernière fois c'est pas bien de pas honoré ses rendez-vous et il faut pouvoir s'assurer que les créneaux bénéficie. À d'autres, au cas où on ne soit pas en capacité de l'honorer. Toutefois le dispositif prévu allez pénaliser de façon disproportionnée des publics, nous le savons déjà précarisés, et donc les les éloigner encore plus du soin, ce qui est exactement l'inverse de ce que nous voulons faire. Je l'ai dit ce compromis comprend aussi des dispositions critiquables. C'est le cas de l'encadrement des effectifs des assistantes et assistants dentaires. D'une part le texte leur accorde davantage de compétences il il et elles pourront désormais contribuer aux actes d'imagerie à visée diagnostic comme les radios aux actes prophylactique aux accords aux et au soir post-chirurgicaux. De l'autre côté le compromis prévoit qu'il ne pourra pas y avoir plus d'assistantes et d'assistante dentaire qu'il y a 2 chirurgienne dentiste et de chirurgiens dentistes dans un établissement. évidemment il faut éviter la dérive de la montée en compétence. Je pense qu'on est tous bien d'accord pour dire que ce ne serait pas une bonne idée qu'il y ait des structures qui emploierait quasiment uniquement des assistantes et assistants dentaires et qui pourrait avoir un effet délétère notamment sur la qualité des soins. Toutefois, il faut aussi penser à la charge de travail des assistantes et des assistants dentaires il elles auront plus de travail comme le texte leur accorde plus de compétences. Sans aucune contrepartie cette contradiction, elle relève d'un problème général qui est malheureusement inhérents à ce texte au fond la solution proposée par ce texte, c'est de faire monter en compétences. Toutes les personnes qui constituent la colonne vertébrale de notre système de santé, mais en améliorant en aucun cas leurs conditions de travail et en les payant pas un euro de plus et c'est là qu'on a un problème parce que le problème de nos systèmes de santé. Nous ne savons ce sont des années de sous-investissements. Le résultat c'est que nous manquons cruellement de professionnels de santé, alors que nous comptons 58 professionnels de santé pour 1000 personnes en France, on en compte 84 pour 1000 aux Pays-Bas, 90 au Danemark, 111 en Norvège. Soit 2 fois plus. Nous pouvons donner plus de responsabilités à toutes ces personnes qui sont déjà là qui se lèvent tôt qui travaille toute la nuit les jours fériés. Mais ces efforts seront vains ses efforts de court terme, moyen terme seront Vincent, amélioration des conditions de travail, sans revalorisation des salaires et sans investissement dans le soin en général donc au lieu de demander à toutes ces personnes de faire toujours plus de soigner plus vite plus efficacement, il faut s'attaquer au sous-investissement chronique dans notre système de santé. Il faut accélérer les formations embaucher plus de professionnels de santé améliorer leurs conditions de travail et enfin leur payer une juste rémunération. Mettre plus de pression sur des personnes pas plus nombreuses pas mieux payé n'améliorera pas l'accès aux soins, ni la confiance, la confiance. Je crois qu'elle réside par exemple dans le fait de penser que lorsque son enfant a besoin de s'avril contre l'épilepsie, hé ben il pourra y avoir accès. Qu'on va pouvoir trouver un médecin quand on en a besoin et pas 3 mois plus tard que l'accès la pu amortir n'est pas en danger en France qu'on va pouvoir régler la pénurie où les tensions d'approvisionnement que le gouvernement a pour objectif de bâtir un système de Sendai qui est fondée sur les besoins et non sur les coûts. Pour toutes ces raisons, le groupe écologiste s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie. Merci la parole est maintenant Abdallah Hassani pour le groupe du Rassemblement démocratique progressiste et indépendant. Madame la présidente. Mais c'est le ministre, chers collègues. Nous savons tous, l'inquiétude des Français face aux difficultés d'accès aux soins. Elle est réelle partout même si certains territoires sont particulièrement touchés. Dans mon département, Mayotte, le nombre de médecins généralistes est inférieur à 50 pour une population de plus de 300.000 habitants. Nous manquons de professionnels de santé et la transition démographique médicale risque d'accentuer la pénurie. Il est plus que jamais indispensable de valoriser les professions paramédicales, tout en rassurant les médecins sur l'exercice de leurs compétences et de leur Diane diagnostic. L'accord de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi améliorant l'accès aux soins par la confiance et donc très bienvenue. C'est un texte pertinent. Équilibré qui. S'il ne répond certes pas à tous les défis, permet d'avancer de façon consensuelle et pragmatique. Il favorise les synergies partage les tâches au bénéfice des praticiens et des patients. Il permet un accès Direct aux infirmières en pratique avancée. Hé ho masseur kinésithérapeute. Qui exerce à l'hôpital en clinique dans un établissement socio. Social. Médico-médico-social ou en ville, dans une maison ou un centre de santé. Une expérimentation sur 5 ans. Dans 6 départements, dont 2 d'outre-mer permettra un autre cet accès Direct au sein L'accès Direct aux orthophonistes. Également facilité, y compris dans le carde d'un set c'est TPS, si le projet de santé prévoit. Toujours faciliter le port. Pour des patients. Le texte élargit les compétences des y'pas infirmiers assistants d'Inter. Pédicure peu peau de l'ogre orthoprothésiste et opticien lunetier. Les pharmaciens pourront renouveler une ordonnance expirée pour le traitement d'une pathologie chronique pratiqué des prélèvements dans le cadre de dépistage de cancer du cancer du col de l'utérus. La profession de préparateur en pharmacie et réformer ses préparateurs pourront administrer des vaccins et des tests rapides d'orientation diagnostique. Enfin les assistants de régulation médicale sont reconnus comme profession de santé. Un consensus s'est fait autour d'un principe de responsabilité que collective des professionnels de santé à la permanence des soins les efforts seront partagés. Par toutes les structures et soignants pour n'est pas privés de soins les malades parfois le consensus n'a pas été possible, je pense au rendez-vous non honorés auprès des médecins et des professionnels de santé ainsi qu'à la revalorisation de l'engagement territorial des médecins. les réflexions pardon vont néanmoins se poursuivre ainsi que l'a dit le président de la République le 26 avril lors d'une visite d'une maison de santé avant d'hommes je cite l'objectif c'est de continuer ce qui a été lancé. La formation des davantage de médecins prendra des années. Priorité est donc donnée aux délégations date. La la Premier ministre, au-delà des mesures déjà mises en oeuvre vient de réaffirmer la volonté d'apporter des réponses rapides et concrètes à l'une des préoccupations majeures des Français. Un décret va donner davantage de marge de manoeuvre aux ARS pour adapter les règles à la réalité des territoires il natation toute particulière sera accordée aux conditions d'exercice des professionnels de santé, logement, sécurité mobilité le travail sera menée avec les élus, nous en avons l'assurance. Et des Comptes publics Gabriel Attal a confirmé le souhait du gouvernement d'un mécanisme qui permet de sanctionner les absences à un rendez-vous médical avec un remboursement minoré du rendez-vous suivant respecter un rendez-vous médical n'est pas privé. Une personne qui cherche en vain Et la parole est maintenant Rémi Cardon. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.

Alors que nous examinons aujourd'hui cette PPL portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance au Bruxelles de santé une nouvelle PPL visant à, je vous le donne dans le 1000. Améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels nous parviendra avant l'été la novlangue elle se porte bien. Mais Monsieur le Ministre, c'est le déficit d'une loi santé qui se fait criant. Par la voix de cette PPL, le gouvernement a notamment souhaité répondre à la pénurie de médecins généralistes par de nouveaux partage de tâches. Le groupe socialiste, écologiste et républicain reconnaît de longue date, l'opportunité de ces partage nouveau à 2 conditions que ceux-ci soient articulées aux soins de parcours de soins et qu'il garantissent un haut niveau de compétence. Condition sine qua non d'une prise en charge, assurant l'égalité des soins. Le texte initial était loin de l'équilibre. D'ailleurs l'appel à manifester inédit d'un autre professionnel en est une illustration. La marche était donc autre et pourtant je me réjouis qu'un consensus ait pu être trouvé en commission mixte paritaire sur le fondement du texte amendé par le Sénat. Plus encore, alors que les rapporteurs avait indiqué lors de l'ouverture des travaux de la CMP que les conditions d'un accord n'étaient pas réunies. C'est un travail parlementaire qu'un travail de fond qui a permis de faire émerger un compromis satisfaisant, notamment sur l'accès Direct aux infirmières de pratique avancée quand le travail parlementaire est respecté. Il s'était fructueux et ainsi les infirmières, les orthophonistes, les kinésithérapeutes, les pharmaciens biologistes les pédicures podologues les assistants dentaires les opticien lunetier se verront d'opter de le rôle pivot du médecin généraliste a été préservé et les dispositions inadaptés et donc inefficiente ont été retirés. Désormais cette proposition de loi est globalement équilibrée, elle ouvre de nouveau partage de tâches sans désorganiser les parcours de soins pour cette raison, notre groupe votera en faveur de ce texte. Comme je l'indiquais préalablement cette proposition demeure cependant parcellaires. Un de ses angles morts. Par exemple l'un des plus saillant concerne la question de la formation, aussi longtemps que les moyens manqueront la pénurie de médecins persistera et on en forme toujours pas assez, et le déploiement des IPA restera théorique. Il est inutile de se concentrer à l'excès sur le cadre législatif de ce déploiement sans en assurer la réalité. La réalité c'est que ce texte permet le déploiement de plusieurs milliers d'infirmières de pratique avancée en ambulatoire. Monsieur le Ministre en assurez-vous les conditions. Enfin le parcours législatif de cette proposition illustre bien la nécessité d'une véritable concertation avec les corps intermédiaires ici avec les professions concernées. Et en miroir il illustre aussi l'impasse des propositions et des décisions technocratiques ou brutal d'où qu'elle provienne les injonctions ne font pas une politique. Tout au plus, certaines en masquer les échecs. À ce titre, la proposition de loi à venir que je citais porte à nouveau des mesures inutilement clivante et potentiellement contre-productif. Monsieur le Ministre recherchons les voix d'accord et négocions, la loi n'est pas un bâton qu'on brandit face à des professionnels qui inévitablement se braque. Après l'échec cinglant des négociations conventionnelles. Il est plus qu'urgent que la majorité. Et le gouvernement. Face à ces professionnels et pour que la priorité affichée sur la santé amène une nouvelle politique associant étroitement l'ensemble des acteurs, change de méthode définitivement je vous remercie. Merci. La parole est maintenant Laurence Cohen. Pour le groupe. Républic. Communistes, écologistes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans un entretien aux lectrices et aux Lecteurs du Parisien dimanche 23 avril, le président de la République s'est inquiétée je cite de ne plus avoir assez de soignants dans le pays avant d'invoquer une réponse multifactoriel. Il était temps de s'inquiéter alors que toutes les propositions soumises ici même notamment par notre groupe ont toujours été balayées d'un revers de main. Alors qu'on attend toujours une grande loi santé, l'une des pistes envisagées par le gouvernement consiste à ce que les personnels des caisses primaires d'assurance maladie trouve un généraliste en priorité au quasi 800.000 patients en affection longue durée. Hors j'ai été récemment alerté par le syndicat nader. CFTC sur les risques de réduction des effectifs des caisses de la Sécurité sociale. Dans le cas de la négociation des futurs convention d'objectifs et de gestion 2023 2027 entre 2004 et 2019 près de 25.000 postes ont été supprimés dans les organismes de Sécurité sociale, dont 80% proviennent de la Caisse assurance-maladie ainsi un emploi sur 5 a disparu en 15 ans. Je relaie donc avec l'ensemble des membres de mon groupe. L'inquiétude des agentes et agents d'accomplir leur mission correctement et pour les usagers d'accéder au service public de la sécurité sociale, il y a une contradiction monsieur le ministre, entre la logique de réduction des effectifs, d'un côté et la volonté de confier au personnel de l'assurance maladie, le soin de contacter chaque patient Le gouvernement souhaite également améliorer l'accès aux soins en libérant du temps médical avec le recrutement de 6000 assistantes et assistants médicaux et en favorisant la délégation des tâches qui sont les deux principales avancées de cette proposition de loi le 6 avril dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur cette proposition de loi qui ouvre un accès Direct sous conditions aux infirmières en pratique avancée au kinésithérapeutes et aux orthophonistes. Nous regrettons que cet accès Direct soit conditionnée à l'adhésion à une structure d'exercice coordonné ce qui va limiter considérablement la portée de cette mesure. À l'inverse, nous saluons la suppression de la taxe lapin à nouveau évoqué par le président de la République et le ministre des Comptes publics pour sanctionner les absences au rendez-vous de santé. Or, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre de la Santé. Je vous cite, attention à ce que le remède ne soit pas pire que le mal et qu'on n'entraîne pas le renoncement aux soins qui serait dramatique, en effet l'idée de pénaliser financièrement les patientes et les patients est économiquement, socialement et d'un point de vue sanitaire, une hérésie, il faudrait au contraire améliorer l'information et la prise de conscience des usagers et revoir le fonctionnement des plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Enfin, nous regrettons que ce texte ne s'attaque pas au coeur du problème de l'accès aux soins qui demeure le manque de moyens financiers et le manque de moyens humains. Il y a urgence à financer notre système de santé à partir des besoins des usagers d'instaurer une réelle démocratie sanitaire d'élargir la permanence des soins à l'ensemble des professionnels de santé, avec notamment le rétablissement de l'obligation de garde. Le remplacement du numerus clausus par le numerus apertus à augmenter le nombre d'internes en médecine seulement de 12% alors que les besoins sont largement supérieur. Le noeud gordien de l'accès aux soins demeure l'augmentation des moyens financiers et humains pour les universités et pour le système de santé, il faut le répéter, il paraît que la répétition et pédagogique mais ça a du mal quand même à aller jusqu'au gouvernement, cela est possible si l'on refuse les injonctions de Bruxelles de réduire toujours davantage les dépenses publiques et si on accepte de relever l'Ondam pour 2024 de de 8% à 5% au minimum. Cette proposition de loi va dans le bon sens, mais elle ne résoudra pas les difficultés profondes d'accès aux soins. Comme plusieurs de mes collègues l'ont déjà souligné pour cette raison ne notre groupe le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste maintiendra son abstention comme en première lecture. Je vous remercie. Olivier Henno. Pour le groupe Union centriste a maintenant la parole. Madame Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de commission madame la rapporteure, chers collègues. Difficile, en étant le 7ème orateurs de ne pas exprimer quelques redites. Mais c'est aussi l'occasion de profiter de ce temps de parole pour faire quelques constats exprimé quelques convictions. Permettez-moi tout d'abord de renouveler mes remerciements et félicitations pour le remarquable travail de Corinne Imbert rapporteure sur ce texte, mais aussi pour tous les textes sur la santé en général. Une fois encore, mes chers collègues, nous abordons le grand sujet de la santé, par l'intermédiaire d'une PPL certes après une commission mixte paritaire conclusive, mais nous abordons le sujet santé. Par l'arme à la marge. Or, je le répète inlassablement, il nous faut une grande loi santé de remise à plat afin d'aborder de front la pénurie de médecins, la crise hospitalière ou encore les difficultés de la médecine de ville. Notre conviction c'est que la crise hospitalière par exemple s'amplifie les événements dramatiques de Grenoble en sont la démonstration comment se fait-il qu'en France, pays renommé pour son système de santé universel nous puissions à ce point manqué de lits disponibles le constat et et donc le contexte est donc alarmant ce contexte ne freine pas l'ardeur de la majorité sénatoriale d'être à la hauteur des enjeux ainsi grâce à ces apports le texte final adopté par la commission mixte paritaire. Conserve plus de plusieurs dispositions majeures du texte du Sénat telle que la suppression des dispositions relatives à l'engagement territorial des médecins mais aussi la reconnaissance de la compétence des préparateurs en pharmacie par exemple pour administrer des vaccins listés par arrêté hein, c'est bien la notion d'équilibre fragile exprimée par la madame la présidente, qui est assez juste. Par ailleurs, l'initiative du Sénat d'obliger le pouvoir réglementaire a publié annuellement les listes. Des tests rapides d'orientation diagnostique innovant qui peuvent être utilisés par les professionnels de santé constitue une avancée majeure en matière de transparence et de modernisation de notre système de santé. Le Sénat a également souhaité encadrer strictement l'accès Direct aux infirmiers en pratique avancée. Oh ma soeur kinésithérapeute. Enfin cette. Proposition de loi permettra également aux patients de bénéficier d'une offre de soins élargie. D'une part les patients pourront accéder directement à certains professionnels de santé tels que les IPA exerçant à l'hôpital, les masseurs kinésithérapeutes et les orthophonistes. Cette loi prévoit d'attribuer de nouvelles compétences à certains professionnels de santé les ITA, qui pourront par les IPA qui pourront par exemple pris moins prescrire certains produits ou prestations non soumis à ordonnance. À noter aussi que les pharmaciens pourront également renouveler les ordonnances et administrer certains dépistage et vaccins contre la grippe. Le Covid-19 ou encore la variole. Pour le groupe UC se soit donc pour ce texte, adopté en CMP ah oui sorti donc de quelques réserves. Oui, car cette. Proposition de loi s'inscrit dans une mission double tenter de garantir des soins de qualité à tous les Français mais surtout conserver le rôle central du médecin dans la coordination et le suivi des patients, c'est l'essentiel pour notre groupe UC se tu équilibre fragile. C'est une expression. Je le répète qui est juste car il est vrai que les médecins ont de plus en plus ce sentiment d'être des boucs émissaires de la crise de la démographie médicale des réserves. Parce que le renforcement des compétences du personnel paramédical doit être affiné et expérimenté. C'est le cas d'ailleurs. Mais multiplier les expérimentations et je pense, ça a été dit mais nous le disons à notre tour, qu'il va falloir approfondir et travailler cette question de, de la formation pour les médecins comme. Pour les professions para-médicales ces réserves exprimées nous voterons donc ce texte car. La désertification médicale qui au fond justifient ce ce texte, je le crains est inscrit pour longtemps. Il restera une préoccupation majeure pour de nombreux territoires et de nombreuses communes. Je vous remercie. Et maintenant dernier orateur. De ces explications de vote, le président Jean Claude Roquier à la parole. Un

L'amitié française né dans le tablier de Micha comme. Elodie Gustave Faubert s'est développé grâce à Trousseau Claude Bernard et bien d'autres. Autant de grands noms qui ont prêté la place de la France dans le parmi les meilleurs sans système de santé au monde. Pourtant le modèle français connaît aujourd'hui la crise la plus grave selon nées de l'histoire. Il les réformes menées ces dernières années n'ont pas permis d'enrayer la dégradation. À l'heure depuis plusieurs décennies, bien au contraire, on devrait dire. ni sur de travail dégradées épuisement du personnel médical. Perte d'activité d'attractivité, manque de reconnaissance. Les symptômes sont nombreux aujourd'hui. Plus de 7 millions de Français sont dépourvus de médecin traitant et 600.000 d'entre eux sont atteints d'affections longue durée. La désertification médicale le plus en plus de territoires. Prévoit ainsi les populations de plus en plus importante d'un suivi médical de qualité. Le 6 janvier dernier à l'occasion des voeux aux acteurs de la santé, le président de la République a rappelé la nécessité de réformer le système de santé ou à monsieur le Ministre. Avait reconnu qu'il y avait urgence car mon système de santé fragilisée à bout de souffle, grâce à la vigilance extrême des hommes et femmes de terrain. Il est plus que nécessaire de repenser le système de santé avant qu'il ne s'effondre comme vous l'avez rappelé, la semaine dernière lors de la présentation du bilan du conseil national de la refondation en santé. Refonder. Ce n'est pas colmater les brèches. Le groupe du RDSE ne peut que souscrire à ces propos. Bon temps ce texte ne plus nous serons bien loin de la grande loi santé que nous appelons tous de. Cette refondation doit se faire avec la coopération des acteurs de terrain, notamment des professionnels de santé qui pendant la crise sanitaire ont su relever des défis extraordinaires et nous montrer qu'il fallait leur faire confiance. C'est pourquoi notre groupe regrette que l'examen de cette proposition de loi sur intervenue après les négociations conventionnelles avec l'assurance-, maladie qui était en cours et que les conclusions et les conclusions du Conseil national de la refondation qui n'était pas n'était pas encore rendu. Notre collègue, Véronique Guillotin là j'ai déjà annoncé le 14 février dernier. Alors que la proposition de loi vise à améliorer l'accès aux soins par la conférence aux professionnels de santé, les médecins ils y ont cru. On y ont vu de la défiance. Bon nombre d'entre eux craignent en effet que ce texte se dégrade la qualité de prise en charge des patients, c'est surtout la question de l'accès Direct qui a cristallisé le l'essentiel des oppositions. D'autant que la je dirais qu'on JPA ma soeur qui a thérapeutes et orthophonistes dans le cas de structures d'exercice coordonné on dû faire l'objet d'expérimentations, c'est du moins ce que les deux dernières lois de financement de la Sécurité sociale. Prévoyez. Sur la forme je tiens toutefois salué le travail de notre rapporteure qui en première lecture avait amélioré la proposition de loi. Nous nous réjouissons que le texte adopté en commission mixte paritaire reprennent très largement les modifications apportées par notre assemblée. S'agissant de l'accès Direct aux IP ma soeur kinésithérapeute là ça me plaît ici réservé aux structures d'exercice coordonné les miens intégré partageant une pote une patiente telle commune à l'exclusion des CPTS qui feront toutefois l'objet d'une expérimentation. Cette relation permet de préserver le rôle pivot du médecin dans la coordination des soins et le suivi des patients. Plusieurs dispositions va dans le bon sens j'citerai que quelques-unes. La reconnaissance. De la qualité de professions de santé aux assistants de régulation médicale et qui est déjà attendu et permettra je suis sûr de renforcer notre activité d'une profession indispensables à l'organisation du système de souris. Pérenniser la possibilité pour les préparateurs en pharmacie d'administrer certains vaccins nous semble également une bonne chose. Tout comme l'extension du délai de renouvellement des prescriptions de un à 3 mois pour les patients atteints d'affections de longue durée. Je pense surtout à la possibilité pour le pharmacien biologiste de pratiquer le dépistage du cancer du col de l'utérus. 3000 nouveaux cas et 1000 décès sont à déplorer chaque année en France. Multiplier les moyens de dépister est indispensable. Nous nous félicitons que le gouvernement est déposé un amendement visant à pérenniser cette compétence pour toutes ces raisons, le groupe vous dire déesse votera en faveur de cette proposition de loi. Bien, mes chers collègues. Les explications de vote sont terminées. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé telle qu'elle résulte de du texte élaboré par la commission mixte paritaire et avec les amendements du gouvernement que vous avez adoptée en début d'examen. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Elle est donc adopté. Nous allons enchaîner avec le texte suivant, Monsieur le Ministre reste au ban puisque c'est encore vous, madame la présidente de la commission des affaires sociales reste au ban puisque c'est encore elle. Et nous songeons juste deux rapporteurs. Et notre collègue Jean je crois va venir au banc des rapporteurs. merci madame la rapporteure. Nous allons donc maintenant examiner la discussion deuxième lecture de la proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale visant à améliorer l'encadrement des centres de santé le, la parole est d'abord à monsieur le ministre de la Santé de la prévention. Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Assainir notre système de santé est un impératif pour l'avenir. Je l'ai répété la semaine dernière devant les représentants des professionnels, les élus et toutes les parties prenantes réunis et au ministère pour. La rencontre plénière du Conseil national de la refondation, santé. On ne construit bien que sur des bases saines et solides. On avance bien qu'en suivant des principes fermement établi. Nous sommes déterminés à mener à réussir toutes les réformes permettant de replacer l'éthique au coeur de notre système. Cela passe par la régulation des dérives la juste utilisation des deniers publics, la lutte contre la fraude et contre la financiarisation excessive de certaines Patrick Mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Je me réjouis de retrouver aujourd'hui pour je l'espère l'adoption définitive d'un texte important en ce sens qui a déjà été par trois fois voté unanimement à l'Assemblée et au Sénat. Je tiens tout d'abord avoir un mot pour la présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, la députée fait Lydia Khattabi, que je remercie d'avoir été à l'initiative de cette proposition de loi et de l'avoir porté. Je salue également le travail conjoint des commissions des 2 assemblées notamment des sénateurs et du rapporteur Jean-Sol qui, dans un esprit constructif, ont travaillé ensemble pour façonner un texte cohérent et efficace. En effet il est important que cette loi soit adoptée et entre en vigueur rapidement. Le développement soutenu des centres de santé, principalement des centres optiques et dentaires qui sont visés par le texte, nous l'impose. Les chiffres ont été rappelés à de multiples reprises au cours des débats ont compté aujourd'hui près de 1000 centres dentaires sur le territoire français. Leur nombre a progressé de 60% en l'espace de 5 ans, la tendance est similaire pour les centres de soins ophtalmologiques. Je tiens à le rappeler l'objectif de cette loi n'est en aucun cas de s'attaquer au modèle des centres de santé ni de jeter l'opprobe sur les professionnels qui exerce et qui fournissent pour la très grande majorité d'entre eux, un travail de qualité au service des patients. Au service de leurs patients et d'un meilleur accès à la santé de tous. En effet, héritier des premiers dispensaires municipaux dans les villes ouvrières de la banlieue parisienne qui ont vu le jour dans les années 1920 pour nombre de nos concitoyens. Les centres de santé qu'il soit urbains ruraux ou situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont reconnues comme des lieux qui leur permettent d'accéder facilement et rapidement à des soins. Près de 2500 structures rassemble aujourd'hui 38.000 professionnels à travers le pays. Leur présence au coeur des territoires répond à l'objectif de responsabilité populationnelle qui nous est cher. En effet, mesdames et messieurs les sénateurs. Je sais que vous en conviendrez avec moi, réguler n'est pas empêché réguler ses protégés. C'est accompagner le déploiement d'un mode d'exercice collectif, de la médecine qui correspond aux aspirations des professionnels de santé et qui est utile, a donc aux citoyens, c'est garantir aux opérateurs fiable que l'État s'assure de la qualité et de la sécurité des soins. C'est protéger les Français contre des dérives inacceptables qui mettent en danger notre santé en décrédibilisant tout un modèle. Ces dérives si elles sont minoritaires n'en sont pas moins extrêmement grave. Certaines affaires emblématiques ont suscité un émoi légitime dans la société. Je pense notamment aux scandales qui ont constitué les affaires proxy Nanterre et Dentexia avec des abus ayant mérité les chefs d'accusation de violences volontaires et de mutilations avec certains patients souffrant aujourd'hui d'infirmité permanente. Les abus physiques mais aussi financier à coups de surfacturation de sur traitement et de multi-facturation. Outre le coût pour la sécurité sociale de ces pratiques tarifaires frauduleuse. C'est d'autant plus choquant que ces centres de santé ont généralement abusé de la confiance de patients précaires qui voyait dans ces structures, une solution à leurs problèmes de santé. Atteints dans leur intégrité physique et escroquer pour les victimes, c'est la double peine. Je refuse que des investisseurs malhonnête capitalisent sur les difficultés d'accès aux soins de nos concitoyens les plus vulnérables. L'ordonnance du 12 janvier 2018 a permis sans attendent la mise en oeuvre de premières avancées concrètes pour contrôler davantage les conditions d'ouverture et de fonctionnement de ces centres. Nous avons également consolider l'arsenal de notre système de santé en matière de lutte contre la faute sociale. Ce qui nous permet notamment en cas d'infraction grave de déconventionner beaucoup plus rapidement ces centres. Des mesures ont également été étudiés dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022. C'est l'Union des différentes forces de contrôle qui nous permettra d'être plus efficace. Ainsi, au mois de novembre dernier. 10 centres de santé dentaires dans 10 régions ont fait l'objet d'une mission d'inspection, contrôle des agences régionales de santé conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie, les services d'expression du travail et les services fiscaux. Cette mission d'inspection, contrôle a également bénéficié du soutien de la Mission interministérielle de coordination anti-fraude. Cette proposition de loi nous donne aujourd'hui l'occasion d'avancer encore et d'ancrer ces mesures afin de toujours mieux sécuriser les prises en charge et d'assurer la qualité des soins à tous nos concitoyens. Ainsi pour sécuriser le développement des centres de santé nous adoptons aujourd'hui des mesures concertées nécessaire et équilibrée. La logique d'agrément permet de renforcer la démarche de projet de santé autour de laquelle doivent être construits les centres de santé dentaires et ophtalmologiques l'agrément envisagée à l'échelon régional permet également d'inscrire les structures dans un projet territorial plus large définis localement par les agences régionales de santé avec les acteurs du territoire. Nous garantissons la qualité des soins grâce à la transmission, puis la vérification des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens dentistes assistant dentaire ophtalmologistes et orthoptistes dans le dossier de demande d'agrément. Comme à chaque nouvelle embauche nous ne transigerons pas avec la sincérité de la gestion financière en actant l'obligation de certificat d'si on des comptes par un commissaire et leur transmission aux ARS. Nous nous donnons les moyens de procéder plus largement à des contrôles et des vérifications notamment durant la première année puisque l'agrément délivré ne deviendra définitif qui à l'issue d'une période de 12 mois. Nous renforçons les sanctions, grâce à des amendes pouvant aller jusqu'à 500.000 euros et qui viendrait en complément d'éventuelles sanctions pénales pour les cas les plus graves. Nous prévenons les récidives puisqu'un gérant malhonnêtes ne pourra plus ouvrir un centre dans une autre région, après la fermeture d'un premier un répertoire national recensera toutes les décisions de suspension ou de fermeture et sera à disposition de tous les services de l'État et des organismes de Sécurité sociale. Mesdames, et messieurs les sénateurs. Je suis déterminé à assainir notre système de santé et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre les dérives éthiques et financières qui mettent en péril notre modèle social. On nous on nous attaquer à l'intérim dérégulé en plafonnant les rémunérations des praticiens intérimaires. Nous n'avons pas fait autre chose. Cette mesure n'a pas été facile à mettre en oeuvre, j'en conviens, mais c'était absolument nécessaire. De prochaines échéances législatives nous permettront d'ailleurs de nous retrouver bientôt pour débattre de l'interdiction de la pratique de l'intérim en début de carrière pour sécuriser l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes soignants. Aussi mesdames et messieurs les sénateurs. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une fois encore du travail fourni. Et pour votre investissement sur ce texte. Je vous invite à le voter unanimement une dernière fois pour assurer un développement éthique des centres de santé au service d'un accès à des soins adaptés et de qualité pour chacun de nos concitoyens. Je vous remercie. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission. Mes chers collègues. La proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé. Déposée par la présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Fatila cata dit ah d'octobre 2022 a été adopté en 2ème lecture par l'Assemblée nationale le 14 février dernier. Je regrette que nous devions l'examiner à nouveau. Car nous avions travaillé dans un esprit consensuel en première lecture pour permettre à l'Assemblée nationale de l'adopter définitivement. L'Assemblée nationale a certes adopté conforme 3 articles relatifs à la prévention des conflits d'intérêts à l'identification des professionnels de santé par un numéro personnel. Distincte de la structure et au régime de sanctions applicables et elle a approuvé la suppression de 2 articles dont les dispositions avaient par cohérence été transférés par le Sénat au sein d'autres articles de la présente, proposition de loi. Mais 8 articles restent en discussion et des modifications réalisées par l'Assemblée nationale de justifier guère de reporter l'adoption définitive de ce texte. À l'article 1er relatif aux procédures d'agrément. L'Assemblée nationale a ainsi choisi d'intégrer les activités hors optique dans le Champ des activités soumises à l'agrément du directeur général de l'ARS, mais aussi de supprimer la possibilité de de consultation des projets de santé par les conseils départementaux de l'eau. Je me bornerai à constater. Que les activités hors optique. Sont a priori réalisées dans les centres qui ont une activité ophtalmologique, d'une part et que loin de mettre à disposition. Les projets de santé de tous les centres. Nous n'avions donné qu'un droit de consultation aux ordres. Qui me paraissait légitime au regard des missions qui sont données à ces derniers. Surtout, l'Assemblée nationale a introduit une disposition nouvelle concernant les modalités de réalisation de la visite de conformité en prévoyant la possibilité. Pour la personne mandatée de ne pas annoncer son identité ni l'objet de sa visite. Ces dispositions qui aurait pu tout à fait relever d'un décret d'application me semble tâcher délicate dans leur mise en oeuvre. En effet. Comment la personne mandatée aura-t-elle accès à l'ensemble des éléments lui permettant de juger de la conformité du Centre de santé au delà d'une simple observation sur les modalités d'accueil. La visite de conformité a bien pour objet d'apprécier les pratiques du centre et de ces praticiens et gestionnaire. À l'article 1er bis relative à la conservation des dossiers médicaux des patients et à leur transmission en cas de fermeture du centre de santé si l'Assemblée à préserver l'obligation de conservation dans des conditions garantissant la continuité de prise en charge des patients. Elle a privilégié en cas de fermeture, une information des ordres à une transmission aux ARS des dossiers. Nous avions introduit cet article en première lecture pour répondre à une préoccupation forte concernant le rôle de prise en charge pour certains patients dont les dossiers médicaux manquait à la fermeture du centre de santé et dont la reprise des soins a été largement obéré. Concernant l'article 1er quater. Relatif aux modalités transitoires applicables aux centres existants. L'Assemblée nationale. Contenté de modification rédactionnelle. À l'article de. Les députés ont pour l'essentiel rétabli leur rédaction de premières heures c'est-à-dire réinscrit dans la loi les précisions relatives au fonctionnement du comité médical ou dentaire et à l'obligation pour les gestionnaires d'assurer la transparence du Centre sur l'identité des professionnels de santé qui prennent en qui prennent en charge des patients. Sans doute peut-on partager la crainte que le pouvoir réglementaire ne soit tenté d'amoindrir des obligations nouvelles que l'on souhaite vouloir contribuer à l'amélioration de la qualité des soins. Mais fallait-il pour autant rétablir la mention selon laquelle le gestionnaire s'assure que le règlement intérieur de l'établissement prévoit le port d'un badge nominatif indiquant la fonction d'un professionnel de santé. Les modifications touchent tutsi également au fond. Du dispositif puisque le comité médical être rendus coresponsables de l'amélioration de la qualité des soins et de la formation continue du dispositif les contours d'une telle rançon responsabilité ne sont pas plus claires qu'en première lecture. C'est pourquoi nous l'avions retoucher et devront de toute façon être précisées par le pouvoir réglementaire. À l'article IV. Les députés ont complété l'obligation de publicité des décisions de sanctions financières. En étendant ses effets au site internet des autorités sanitaires. Appropriées et en l'accompagnant d'une mise en demeure du gestionnaire de les publier sur le site du Centre lui-même. Ils ont un autre transformer en compétences liées. Ce qui n'était qu'une faculté offerte aux directeurs d'ARS de refuser de délivrer. Pisser ou l'agrément de l'ouverture d'un centre lorsque les membres de son instance dirigeante ont fait l'objet d'une mesure de suspension ou de fermeture. L'article 7 a été complétée par une disposition améliorant l'information des patients en cas de déconventionnement d'un centre par l'assurance maladie. Enfin, les députés ont tu rétabli l'article 9 qui prévoit la remise par le gouvernement d'un rapport sur les moyens des agences régionales de santé. Le rétablissement de cette demande de rapport et pour moi, l'exemple le plus frappant des désaccords très surmontable à l'égard du texte que nous avions adopté. Monsieur le Ministre, je crois. Difficile de nier que la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture aurait pu sans préjudice aucun pour la bonne application de la loi, être adoptée telle quelle, par l'Assemblée nationale en 2ème lecture. C'est pourquoi, mes chers collègues. La commission vous propose d'arrêter ici la navette parlementaire pour ce texte en préconisant son adoption définitive par le Sénat dans l'intérêt des patients et ce d'autant que le nouveau signalement pour détournement de fonds publics d'un centre de santé a récemment fait la une, je vous remercie.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

3 mois après l'examen de ce texte en première lecture, le voici de nouveau soumis au vote notre chambre ce texte intervient en réponse aux nombreux scandales qui ont surgi depuis 2016 et aux dérives survenues dans certains centres dentaires dit low cost. Pensant pouvoir bénéficier de soins à des tarifs compétitifs, plusieurs milliers de victimes ont ainsi été surfacturés escroqué voire mutilé les centres de santé ont connu une forte expansion depuis 2009 grâce à la loi dite HPST qui a supprimé l'obligation d'agrément pour leur ouverture et la remplacer par une simple déclaration de conformité. Ce changement de procédure est intervenu pour pallier les difficultés de certains Français à payer leurs soins dentaires et qui soit, partez, partez, se faire soigner à l'étranger soit y renoncer. Suite aux dérives constatées depuis le texte que nous avons à examiner propose de réinstaurer l'obligation d'agréments nécessaires à leur ouverture et plus largement de renforcer de façon accrue, le contrôle des centres de santé exerçant une activité dentaires ou ophtalmologiques l'examen en 2ème. Lecture à l'Assemblée nationale a par ailleurs étendu le périmètre d'application des dispositions au centre ayant une activité or tu optique. Le texte propose de ne délivrer qu'un agrément provisoire qui ne deviendra définitive que lors de la transmission à l'ARS d'un dossier comprenant notamment les contrats de travail et les diplômes des professionnels du Centre. À cela s'ajoute la possibilité d'une visite de conformité du Centre. L'instauration d'un comité médical au sein de chaque centre est l'une des mais des mesures les plus intéressantes du texte, chargé de l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Ce comité devra se réunir au moins une fois par trimestre. Il permettra aux professionnels d'échanger et de s'interroger régulièrement sur le respect des bonnes pratiques et les comptes rendus devront être transmis transmis à l'ARS. Par l'obligation de transmission des comptes annuels d'information. En cas de suspension de fermeture de l'activité ou encore la publicité des sanctions financières éventuellement prononcer. Le texte prévoit également une meilleure transparence du fonctionnement descente par une information accrue de l'ARS du conseil départemental de l'ordre de l'assurance maladie, mais aussi des patients. L'ensemble des mesures proposées permettra assurément de renforcer les conditions d'ouverture et le contrôle de l'activité de ces centres et surtout et c'est là l'objectif de ce texte. Il permettra de sécuriser la prise en charge des patients afin que nous ne découvrions plus de patients victimes de mutilations. Dans des établissements censés être des lieux de soins. Nous saluons l'adoption conforme par l'Assemblée nationale de plusieurs articles comme celui visant à prévenir les conflits d'intérêts ou celui aggravant le montant des sanctions financières prévues en cas de manquement à la qualité ou à la sécurité des soins, même si nous regrettons que des modifications, parfois mineures aient été apportées au texte et retarder son adoption définitive. Nous espérons aujourd'hui une adaption une adoption enfin conforme pour résoudre dès que possible ces situations inacceptables. Notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi, je vous remercie. La parole est maintenant Raymonde Poncet Monge pour le groupe écologiste solidarité et territoires.

madame la présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. Ces dernières années des scandales sanitaires impliquant des centres de santé ont mis à jour des pratiques maltraitante et de fraude à la sécurité sociale. Au coeur de ses affaires, encore et toujours la recherche de profits qui impacte plus durement les plus modestes et prospère sur un système de santé désormais à plusieurs vitesses. Car dans la majorité des cas de fraudes. Les fraudeurs ne sont pas les assurés qui ici s'avère en fait les victimes en 2022, l'assurance maladie a détecté et relever un montant de fraudes inégalée jusqu'alors. Plusieurs centaines de millions d'euros dont les 3 quarts porte sur les frais de santé pour l'essentiel facturés à tort par des professionnels de santé. De fait, l'instrumentalisation du modèle des centres de santé dans une finalité lucrative a été rendue possible par la raréfaction de l'offre de soins et l'augmentation des inégalités d'accès aux soins sur les territoires, lors du 2ème. Examen de ce texte à l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre de la Santé et de la prévention. Vous avez déclaré le premier principe qui doit guider toutes nos décisions de politique de santé et la lutte contre toutes les inégalités d'accès aux soins. Il faut pour cela. Améliorer la proximité de l'offre non lucrative pour que le 100% santé ne se traduise pas par l'offre de service à bas coût de fait à basse qualité opportunité de solvabilisation pour des acteurs attirés par la la pâte de gains rapides. En vertu des améliorations déjà engrangés lors de la navette. Le groupe écologiste se prononcera pour le vote conforme. Car nous nous félicitons que notre amendement adopté en première lecture au Sénat et conserver. Rendent obligatoire la publication de la sanction financière prononcée à l'encontre d'un centre frauduleux par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé et ce sur le site de l'ARS. Un amendement proposé par nos collègues aussi du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et adopté en 2ème lecture complète cette mesure en rendant effectivement obligatoire la publication par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé des décisions de sanctions financières sur le site de toutes des autorités sanitaires appropriées. qui a complété par la mise en demeure de l'organisme gestionnaire, sanctionné de publier cette décision sur son site internet. Ces mesures renforcent la transparence et donc la protection à l'égard des usagers. Étant donné que l'agrément par l'ARS avait été supprimé, faute de moyens humains suffisants, nous adhérons rétablissement à l'Assemblée nationale du rapport sur les moyens alloués aux ARS afin qu'elle s'inquiète des nouvelles missions fixées par la proposition de loi. Les moyens humains d'inspection, contrôle de l'État ainsi que des organismes d'assurance se sont raréfiés au fil des années, il nous faut les rétablir. Il nous faudra il faudra les augmenter. Enfin, nous tenons à saluer le travail effectué par la majorité. La quasi-majorité des centres de santé, loin des affaires. Loin de ces affaires qui explique cette proposition de loi la lucrative IT est antinomique du modèle social et économique des centres de santé qui s'inscrit-elle dans un projet collectif. Une des priorités étant de favoriser l'accessibilité financière et géographique aux soins. Si les centres de santé demeurent des piliers de l'accès aux soins et de lutte contre les déserts médicaux. Leur forme associative ne peut être toléré à être détournés afin de contrer ces pratiques frauduleuses et malgré quelques réserves déjà exprimées à la première lecture. Le groupe écologiste votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Et la parole. Sera maintenant à Patricia Schillinger. Le groupe. Rassemblement démocratique progressiste et indépendant. Madame Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues à l'occasion de la rédaction du rapport les collectivités à l'épreuve des déserts médicaux, l'innovation territoriale en action. J'ai pu avec mon collègue et co-, auteur de ce rapport Philippe mouiller prendre toute la mesure du rôle des centres de santé dans l'amélioration de l'accès aux soins en mettant en oeuvre une organisation qui libère du temps médical au profit des professionnels et de leurs patients. Ces centres constituent un moyen déterminant de lutte contre la désertification médicale et qui gagne de nombreux territoires et c'est bien là leur vocation originelle et la force de leur projet, en dépit des scandales qui ont mis en lumière l'usurpation et à des fins purement lucratives de leur cadre juridique et institutionnel. Dans ce contexte, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en seconde lecture rêver d'une importante importance particulière. Elle répond à à l'impérieuse nécessité de mieux encadrer l'activité de ces centres de manière à prévenir les dérives auxquelles ont pu se livrer des gestionnaires peu scrupuleux en profitant de l'assouplissement du régime d'ouverture voulue par la loi HPST de 2009 surfacturation sur traitement problème majeur d'hygiène et de sécurité des soins. Mutilation non pertinence des actes réalisés autant d'abus qui ont conduit le gouvernement sous le précédent quinquennat en 2018, a adopté plusieurs ordonnances visant à s'assurer de la qualité des soins. Dispensés dans les centres de soins et à mettre un terme à des pratiques contraires à l'éthique, à la suite d'un nouveau scandale proxy dentaire en 2021. Force est de constater que notre cadre juridique reste trop permissif et commande. Au législateur qu'il se saisisse du sujet. À ce titre je tiens ici à saluer une nouvelle fois au nom du groupe RDPI l'initiative de Madame la Présidente Khattabi qui s'est emparée de ce sujet et je la remercie pour son engagement. pas bien sûr le travail de notre rapporteure les sénateurs. Qui a su dans le courant de la navette enrichir le texte de plusieurs dispositions qui durcirent un peu plus les conditions d'ouverture des centres de santé. Le texte renforce ainsi le rôle des ARS en consacrant le retour et à une procédure d'agrément préalable, dont la délivrance et le maintien sont notamment conditionnée à la transmission des diplômes et des contrats de travail. Les pouvoirs de sanction du directeur de l'ARS sont renforcées ces derniers sont désormais capacité de mettre hors d'état de nuire des gestionnaires dont les comportements frauduleux ont été constatés. Je me réjouis globalement du consensus transpartisan qui a entouré l'examen de ce texte et notre comme notre rapporteur a pu l'observer en commission que la version issue des travaux de l'Assemblée nationale en seconde lecture ne présente pas de désaccord majeur avec le texte tel qu'issu du Sénat en première lecture, dès lors, on peut toutefois regretter que l'Assemblée nationale n'est pas adopté qu'on se conforme la version du Sénat, ce qui aurait permis une entrée en application plus rapide du texte dans le plus grand intérêt des patients aussi dans l'espoir d'une entrée en vigueur rapide de cette proposition de loi avec le groupe RDPI, nous n'avons pas souhaité apporter de modifications au texte et soutiendront avec force son adoption conforme les logiques de rentabilité et le profit ne saurait se déployer au détriment de l'accès de tous à des soins de qualité et encore moins aux dépens de la santé, santé de nos concitoyens, ceci n'est pas négociable, je vous remercie.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la présidente de commission. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cet hémicycle du Sénat pour examiner en 2ème lecture la proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé. Cette proposition de loi a été élaboré en réaction à plusieurs scandales sanitaires impliquant des Centres Dentaires dont Dentexia en 2015. Qui a affecté 2400 patients et le scandale proxy dentaire en 2021 qui a lui aussi donné lieu à des soins superflu dangereux dans des structures uniquement mus par la recherche de super profits. Ces scandales illustrent malheureusement certaines dérives qui affectent notre système de santé. 2544 centres de santé ont été recensés dans notre pays en 2022 et leur répartition n'est malheureusement pas homogène sur l'ensemble du territoire. Les centres de santé sont majoritairement implantés dans des zones urbaines. À forte concentration démographique de la région PACA Auvergne Rhône-Alpes et bien sûr l'Île-de-France. Ainsi, en Île-de-France, le nombre de centres de santé a augmenté de 160% entre 2016 2022. Il y a là clairement, la recherche de la part. De ses structures d'une Maxima maximisation des profits. Des centres de santé aurait pu contribuer à l'amélioration de l'accès aux soins pour une population. Or force est de constater que les centres de santé ne contribue pas au rééquilibrage de l'offre de soins et en cela ils ne répondent pas à mes attentes. Moi qui suis l'élu d'un département, le Finistère, où une partie de la population n'a pas correctement, accès aux soins. Depuis juin 2017. Des différents gouvernements qui se sont succédé ont malheureusement accru la financiarisation de notre système de santé et cette proposition de loi ne contribuera malheureusement pas à atténuer le phénomène. Cette proposition de loi contient cependant des dispositions qui vont dans le bon sens, comme la réintroduction de l'agrément des centres dentaires ophtalmiques et orthoptiste. Cet agrément des centres de santé n'avait été supprimé en 2009. Dans le cadre de la loi hôpital, patients, santé et territoires suppressions de l'agrément dans l'espoir de faciliter l'installation des centres de santé comme outil de lutte contre la désertification médicale. Espoir déçu, on l'a vu. Cette suppression de l'agrément en 2009 a malheureusement permis l'installation de certaines structures ayant des pratiques frauduleuses. Le groupe des sénateur socialiste, écologiste et républicain. preuve, donc la réintroduction de cet agrément mais s'interroge sur le choix fait de limiter cet agrément au Centre de santé dentaires ophtalmiques et orthoptiste. Pour notre groupe, tous les centres de santé. Devraient être soumis à la procédure d'agrément. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui ne prend pas en compte la multiplication des centres de santé spécialisés en psychiatrie. Gynécologie ou le lien avec le médecin spécialiste se fait uniquement par téléconsultation. La réintroduction de l'agrément abandonné en 2009 nécessite une augmentation conséquente des moyens des agences régionales de santé afin que les nouvelles missions. Que nous allons par le vote de cette proposition de loi leur confier ne restent pas lettre morte. À l'image des contrôles des Ehpads. Pas ou mal fait, comme le démontre le scandale Orpea. L'augmentation des moyens des agences régionales de santé relève de votre responsabilité, monsieur le ministre. Il en va de la santé de la sécurité de concitoyens. C'est pourquoi d'autres groupes est favorable à l'article 9. De cette proposition de loi qui prévoit la remise d'un rapport gouvernemental au Parlement sous 6 mois après la promulgation de la loi. Sur les moyens alloués aux ARS. Pour remplir ses nouvelles missions. Même si notre chambre haute n'est pas favorable à la multiplication des rapports mais là en l'occurrence, il nous semble plus qu'utile. Comme je l'ai dit et sénateur socialiste, écologiste et républicain approuve. Plusieurs dispositions de cette proposition de loi comme celle prévue à l'article 4 qui vise à interdire le nomadisme des fraudeurs et des structures commerciales déviantes. Toutes les dispositions visant à améliorer la qualité des soins. Comité médical comité dentaire dans les centres de santé concernés sont bien sûr à soutenir. Tout ce qui va dans le sens de l'amélioration de la transparence de l'information des patients de la lutte contre les conflits d'intérêts reçoit le soutien de notre groupe. Même si cette PPL ne lutte absolument pas contre le fléau de la financiarisation de notre système de santé. Et sénateur socialiste. Écologiste et républicain s'abstiendront donc sur cette proposition de loi trop parcellaires. Bien que certaines dispositions soit utile aux patients. Comme je le martèle depuis 2017. Il est urgent de réécrire une nouvelle loi de santé qui structure l'offre de soins sur l'ensemble du territoire au service des Français et dans le respect des professionnels de santé. Je vous remercie de votre attention. Laurence Cohen à la parole pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les discours du président de la République et de la Première ministre aux portes une omission difficilement compréhensible en matière d'amélioration de l'accès aux soins, c'est la référence à l'utilité des centres de santé. Face aux difficultés d'accès aux soins, la proximité, les modalités de fonctionnement des centres de santé apporte une solution utile et intéressante que le gouvernement devrait au contraire revaloriser développer nous portons groupe CRCE le projet d'une implantation d'un centre de santé adossé à chaque hôpital dans chaque bassin de vie afin de garantir l'accès aux soins de toutes et tous. Lorsque le 20 avril dernier, les représentants du CSE du Cosem ont adressé un signalement au parle au parquet national financier pour je cite. Malversations financières présumées pouvant relever d'un détournement de fonds publics de prise illégale d'intérêts et d'abus de confiance, j'ai immédiatement exprimer ma solidarité avec le personnel. Profondément attaché aux valeurs des centres de santé qui repose sur l'absence de lucratives malheureusement ce type d'affaire de détournement jette l'opprobre sur l'ensemble des centres de santé publics municipaux mutualistes ou associatifs qui assure une prise en charge des patientes et des patients par une équipe pluridisciplinaire en salariat avec le tiers payant intégral et sans dépassements d'honoraires. L'implantation de marchands d'actes ces dernières années, depuis la suppression du régime d'agrément préalable démontre à la fois la faiblesse des moyens financiers et humains des agences régionales de santé pour assurer leur mission de contrôle des établissements, mais également l'inaction des autres professionnels, y compris lorsque les agissements délictueux sont dénoncés par les personnels des centres de santé, ce dentiste pardon, ah ce dentiste de Marseille. Condamné à 2 ans de prison ferme après avoir mutilé 320 patientes et patients et frauder 1,7 millions d'euros à la sécurité sociale entre 2006 et 2012 et pour lequel l'Ordre des chirurgiens-dentistes attendu plusieurs années avant de réagir. Cette proposition de loi est donc la bienvenue, mais sera-t-elle suffisante et efficace. Nous avons quelques doutes rétablir un agrément pour les centres ayant une activité dentaires ou ophtalmologiques activités pour lesquelles les dérives sont les plus fréquentes, est une bonne chose la joue par l'Assemblée nationale, du rétablissement de l'agrément pour les centres de santé or tu optique est également positif même si l'agrément ne remplacera pas les contrôles des autorités sanitaires. Je l'ai déjà dit mais en l'absence de moyens supplémentaires pour les agences régionales de santé. Nous sommes circonspecte sur l'amélioration effective des contrôles des de santé l'obligation pour le gestionnaire d'assurer la transparence du Centre sur l'identité des professionnels de santé qui prennent en charge les patientes et les patients est également une mesure positive, même si nous aurions souhaité que ce texte aille plus loin et supprime la possibilité d'ouvrir des centres de santé pour des gestionnaires à but lucratif. Il faut en finir avec ces structures privées lucratives, qui voit la carte vitale comme une carte bleue. Cette proposition de loi est toutefois un 1er pas que nous avons soutenu en première lecture et je tiens à remercier notre rapporteur Jean-Sol pour ces enrichissements en attendant des moyens financiers supplémentaires dans la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale. Que j'appelle de mes voeux. Le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste votera donc en faveur de ce texte. Je vous remercie. Et maintenant Olivier Henno à la parole pour le groupe Union centriste. Hé oui madame la présidente. On prend les mêmes et on recommence comme vous disiez tout à l'heure. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteur de commission. Monsieur le rapporteur. Depuis le débat en première lecture de ce texte. Notre constat n'a pas changé, il y a urgence à à mieux encadrer certains centres de santé afin d'en finir avec certaines carences et j'allais dire certains abus même excès. Ce constat est d'ailleurs largement partagée par les acteurs de terrain. Jean Sol notre rapporteur à qui je rends hommage à parfaitement identifié les nécessités de mieux encadrer et contrôler les centres de santé. Je n'ai pas de doute sur l'urgence de légiférer en la matière, la suppression de l'agrément préalable en 2009 et l'assouplissement du cadre juridique que permettez la forme associative ont été à l'origine du détournement du modèle descendre de santé et des dérives constatées en effet le résultat est accablant, qu'il s'agisse. De patients mutilés. Ça a été dit ou des multiples fraudes à l'assurance maladie. Cependant, pour faire le lien avec le débat précédent, je veux à nouveau souligner le côté ubuesque de légiférer à tour de bras, toujours à la marge sur l'organisation du système de santé, lors du débat en première lecture de ce texte j'avais cité Euripide. Ce n'est pas l'abondance. Mais l'excellence qui est richesse la pédagogie c'est l'art de la répétition et donc pour nous, l'urgence c'est une grande loi santé cela sonne comme une évidence. J'en viens maintenant au fond du, du texte rapporté par Jean seul qui répond à des souffrances. Oui des souffrances d'un certain nombre de patients. L'ordonnance du 22 janvier 2018 prise après le scandale Dentexia a certes précisé un peu le droit mais elle n'a visiblement pas été suffisantes. C'est pourquoi le rétablissement de l'agrément délivré par le directeur de l'ARS, l'obligation pour le gestionnaire de transmettre les contrats de travail des praticiens. À l'ARS et l'obligation pour les restes de communiquer ces contrats de travail au aux ordres. Nous sommes tout à fait pertinent. Ça lui aussi. L'article qui prévoit d'obliger les centres à se doter d'un comité dentaires ou ophtalmologiques pour ceux qui exerce ses activités. Un tel comité serait chargé de contribuer à la politique d'amélioration de la qualité des soins et à la formation continue des salariés. Attendu par les patients qui ont vécu de. Véritables. Par les chirurgiens dentistes dans la mesure où les excès de certains cabinets dentaires. Entaché l'image d'une profession qui ne le méritait pas et par l'assurance mal hâtive, victime de nombreuses fraudes. Ces mesures doivent s'appliquer le plus rapidement possible. Toutefois, mes chers collègues. Ça a été dit, rappelons que les centres de santé dans leur grande majorité, qu'ils soient communaux mutualiste ou l'associatif à but non lucratif effectuer un travail de qualité. Je le redis, hein, je le dis les brebis galeuses n'entache pas la bite et de la totalité du troupeau. Les brebis galeuses n'entache pas la probité de la totalité du troupeau, ce que nous devons combattre sans relâche. C'est une forme de logique low-cost si l'Holocauste peut parfois se justifier dans certains secteurs de l'économie comme le tourisme et encore j'avoue être assez dubitatif sur ce principe. J'ai des doutes. Sur qui sont fondées sur low cost. Mais en matière de santé, c'est encore plus inacceptable. Nous n'avons pas peur d'affirmer que l'Holocauste est l'ennemi de la bonne santé. Une autre logique

Voir aussi pour les biotechs. Je veux aussi ajouter que le low-cost ou la surconcentration ne concourent en rien, bien au contraire, à lutter contre les déserts médicaux dans les zones rurales ou dans les zones dites périphériques je tiens enfin à saluer de mesures, premièrement l'introduction d'une obligation pour le représentant légal de l'organisme gestionnaire d'informer dans les 7 jours, le directeur général de l'ARS. Le directeur de la caisse locale d'assurance maladie et le président du conseil départemental de l'Ordre compétent en cas de fermeture d'un centre de santé ou de l'une de ses antennes. Une telle mesure apportera une réponse au problème des cartes de professionnels de santé qui continue parfois de circuler sans contrôle alors que le Centre de santé dans lequel leurs détenteurs exercer ont fermé. Deuxièmement, l'obligation pour les professionnels de santé, salariés d'un centre de santé identifié par un numéro personnel hé bien une telle traçabilité est une exigence morale. chers collègues. Soucieux de lutter contre toute fraude et de rechercher en permanence l'amélioration de la qualité des soins. Notre groupe UC votera ce texte, je vous remercie. Merci. Et maintenant c'est Henri Cabanel qui a la parole pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Madame la présidente. Monsieur le. Le ministre madame la présidente de la commission. Je suis le rapporteur, mes chers collègues. Je pars au nom de ma collègue. Véronique Guillotin. Dans la lutte contre la désertification médicale. Le développement des centres de santé est apparu indispensable. C'est dans cet esprit que la loi hôpital patients santé territoires de 2009. 2009. Faciliter l'implantation les procédures et les contrôles ont ainsi été fortement allégé l'autorisation préalable des ARS n'est plus nécessaire. Une simple déclaration accompagnée de la transmission d'un projet de santé suffit. Dans un contexte de fortes inégalités dans l'accès aux soins dentaires. C'est ça représente une alternative très intéressante en proposant des prix bien moins cher que ceux pratiqués par les chirurgiens-dentistes un exercice libéral attirant ainsi les patients les plus démunis. Rappelons qu'en 2016 le renoncement pour raisons financières a représenté un quart des non-recours aux soins dentaires ou le reste à charge des patients s'élève à plus de 22%. Malheureusement la loi Bachelot a permis à certaines structures d'échapper à la vigilance des autorités et des personnes presque plus. Plus intéressés par l'aspect lucratif que médical ont trouvé la faille. Pour reprendre les propos du Docteur Patrick sur les rares, président de la Fédération des syndicats dentaires libéraux. On a fait rentrer le loup dans la bergerie. Cette course à la rentabilité à Léonie ces structures de leur vocation première notamment dans les centres de santé dentaires associatifs dont la plupart sont spécialisés sur la prothèse et l'aime planétologie beaucoup plus rémunératrice que les soins conservateurs. Et si le nombres de centres de santé dentaires a fortement augmenté ces dernières années. Ces structures sont principalement implantées en Île-de-France et dans la région PACA bien loin, bien loin des déserts médicaux. Avec les conséquences dramatiques que l'on connaît pour des milliers de victimes mutilées et endetté. Les scandales date Dexia ou Proxi dentaires ont permis de mettre en lumière les malversations de quelques-uns qui jette l'eau propre surtout le secteur. Lutter contre ces dérives et encadrer le développement des centres de santé sont indispensables pour garantir la survie du modèle originel de ces structures dans l'intérêt de nos concitoyens et de nos territoires. C'est l'objectif poursuivi par cette proposition à laquelle le RDSE apportera tout son soutien. Comme en première lecture. Certes, quelques mesures ont été prises ces dernières années mais il fallait aller plus loin pour empêcher de nouveaux drames. Le rétablissement de l'agrément le renforcement des sanctions, la mise en place d'un répertoire national de toutes les décisions de suspension ou de fermeture. L'interdiction de demander le paiement intégral des soins avant leur réalisation sont autant de mesures qui permettront de garantir un développement éthique de ces centres de santé. La navette parlementaire a permis d'enrichir le texte, certes, j'ai bien entendu les regrets de notre rapporteur quant aux modifications introduites par l'Assemblée nationale le 28 mars dernier. Remportant ainsi l'adoption définitive de ce texte. un doute aurions-nous pu faire l'économie d'une d'un énième rapport donne ton dossier qui ne sera probablement pas remis de la même façon, nous aurions peut-être pu éviter le rétablissement de mesures relevant du domaine réglementaire. En revanche je salue la décision du député d'avoir imposé l'information systématique des patients en cas de fermeture ou de déconventionnement d'un centre il arrive en effet que la structure oublie déformé ses patients que la sécurité sociale ne prendra pas en charge les soins que sur une base très faible. Quand on sait que certains centres font payer à leurs patients de grosses sommes d'avance et les poussent à souscrire un crédit. Cette mesure est une très bonne chose. Je vous remets. Et maintenant Corinne Imbert à la parole pour le groupe Les Républicains. Nouveau madame

Madame la présidente. Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Nous poursuivons donc en en séance publique, l'examen de la proposition de loi visant à améliorer l'encadrement des centres de santé cette deuxième lecture fait suite aux modifications adoptées par l'Assemblée nationale qui a fait le choix en adoptant non conforme. Le texte du Sénat de reporter l'adoption du texte. Malgré l'importance du sujet. En dépit de l'esprit consensuel du Sénat sur cette proposition de loi qui avait dessiné un terrain d'entente entre les 2 champs 8 articles demeurent encore aujourd'hui en discussion. Si je regrette les modifications apportées par l'Assemblée nationale puisqu'elles sont le signe d'un refus de faire front commun. Je regrette davantage qu'elle ne soit finalement qu'accessoire et que par conséquent, elle ne justifiait pas de reporter l'adoption de ce texte. Mais le sujet bien trop sérieux pour faire l'objet de zizanie. Vous le savez, mes chers collègues. Il s'agit ici de lutter contres les dérives constatées de certains centres de santé qui sont diverses. Non respect du code du travail fraude à l'assurance maladie, fraude fiscale et surtout et surtout, mise en danger de la sécurité des patients. Le scandale Dentexia n'est malheureusement pas un cas isolé et très récemment encore des salariés d'un centre de santé du paysage. Oh les c'est dans le Loiret ont adressé au parquet national financier, un signalement dans lequel il dénonce des faits pouvant être qualifiés d'abus de confiance, de prise illégale d'intérêts d'escroquerie à la sécurité sociale et de harcèlement moral. Rien que ça. Il devient urgent de mettre un terme à ces pratiques qui bien que ne concernant qu'une minorité de structures sont inacceptables. C'est pratique entache la qualité de l'offre de soins et nuisent gravement aux relations de confiance entre patients et entre professions médicales. Cette confiance est pourtant essentiel, voire structurelles puisque d'elle dépendent la qualité et la sécurité des soins. La médecine le soin sont bien trop nobles et précieux pour faire l'objet de doutes de fraude ou de suspicion de mise en danger du pression. Ce n'est pas ici la conception du soin que nous défendons ni l'offre de soins que méritent les patients. Nous devons rendre à la médecine des valeurs qu'elle a toujours porté des valeurs de probité de qualité et d'intégrité. Si les centres de santé ont permis de résoudre certaines difficultés en matière d'accès aux soins, ce dont nous nous réjouissons ne doivent pas déshonoré l'offre de soins ni nuire à la qualité de la prise en charge des patients. Nous devons veiller à ce que la simplification de l'accès aux soins qui est un enjeu crucial ne soit pas synonyme du qui d'une sécurité moindre l'assouplissement du cadre juridique permettant un meilleur accès aux soins à nos concitoyens ne doit pas laisser la porte ouverte aux opportunistes et aux escrocs qui verrait l'appât du gain. Pour ces raisons. Cette proposition de loi établira un encadrement rendue nécessaire par les pratiques frauduleuses de certains centres de santé que trop constaté. Je me réjouis par ailleurs que l'amendement que j'avais déposé en première lecture visant à introduire un ratio de 1 pour 1 dans les centres de santé ophtalmologique qui correspond au ratio entre le nombre d'assistants médicaux, et le nombre de médecins adopté au Sénat ait été conservé à l'Assemblée nationale cette limitation sera un véritable garde-fou et évitera des dérives dans des centres de santé peu scrupuleux. Gage de solidarité le droit à la santé est une composante essentielle du pacte républicain. Parce que l'accès aux soins doit être éthique équitable et le service rendu authentique. La situation actuelle, certains centres de santé. Parsemé de nombreuses dérives nous oblige. Dans l'intérêt des patients. Le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi. C'est bien là l'illustration de la sagesse du Sénat puisque nous soutenons. Ainsi notre rapporteur et le texte en l'état, je vous remercie. Merci. Enfin dernière oratrice. De cette décision générale la présidente Pascale Gruny.

Madame la présidente. Monsieur le Ministre même la présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Le Sénat se prononce aujourd'hui en 2ème lecture sur la proposition de loi qui doit permettre enfin d'encadrer plus rigoureusement et concrètement les centres de santé et nous nous en réjouissons. La prolifération des ces né au centre au sein des zones déjà bien dotées s'est accompagné de fraude à la sécurité sociale d'entorses aux règles déontologiques d'exercice illégal de la profession. De soins non pertinents et de mauvaise qualité, entraînant parfois des dégâts irréversibles sur la santé des patients. Il y avait donc urgence à renforcer notre arsenal pour lutter contre ces abus. Je tiens à rappeler l'engagement précurseur et constant des républicains sur ce sujet avec une première proposition de loi visant à rétablir l'agrément et déposé il y a 3 ans et demi. Mais malheureusement restées lettre morte. À l'époque. Sans doute avions-nous eu raison trop tôt. Le texte que nous examinons aujourd'hui comporte plusieurs avancées majeures. Outre l'indispensable au rétablissement de l'agrément. Je citerai l'obligation d'information des autorités en cas de fermeture d'un centre de santé pour stopper la circulation illégale illégale des cartes professionnelles de santé ou encore la transmission annuelles obligatoires des comptes du gestionnaire à l'ARS pour mieux lutter contre la financiarisation excessive des centres de santé. Je voudrais également et à nouveau salué le travail remarquable des membres de la commission des affaires sociales et surtout de son rapporteur Jean Jean-Sol qui ont eu à coeur de renforcer l'efficacité pratique de cette proposition de loi en en précisant certaines modalités opérationnelles et en veillant à la coordination d'ensemble de ces dispositions. Je pense entre autres à la garantie d'une conservation des dossiers médicaux des patients en cas de suspension ou de fermeture d'un centre de santé mais aussi au renforcement des pouvoirs des ARS après la délivrance de l'agrément afin de faciliter les contrôles sur les Liens d'intérêts ou les contrats liant les organismes gestionnaires à des sociétés tierces. En 2ème, lecture, l'Assemblée nationale a adopté conforme à la version du Sénat Sénat 3 articles relatifs à la prévention des conflits d'intérêts à l'identification des professionnels de santé par un numéro personnel distant de la structure et au régime de sanctions s'appliquent Pour le reste, les députés se sont surtout contentés d'ajustements cosmétiques à la version votée au Sénat. Entre l'ajout de dispositions qui aurait pu relever de décrets d'application, le rétablissement d'articles dans la rédaction de première lecture ou encore de légères modifications rédactionnelles dont on aurait sans doute pu se passer. L'Assemblée nationale n'a apporté aucun complément indispensable à l'économie générale du dispositif. Alors disons-le clairement, la rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture aurait pu sans porter préjudice à la bonne application de la loi, être adoptée telle quelle, par l'Assemblée nationale en 2ème lecture nous évitant ainsi de retarder de plusieurs mois. L'adoption du texte par le Parlement. Alors que le texte aurait pu entrer en application février une modification par le Sénat renverrais une nouvelle fois sa mise en oeuvre qui ne pourrait alors intervenir avant l'été. Je vous invite donc, mes chers collègues à faire preuve de responsabilité comme nous le faisons toujours dans cette maison. En préférant toujours le pragmatisme à l'excès de zèle législatif. Nous devons favoriser dans l'intérêt des patients. Une adoption définitive de cette proposition de loi le plus rapidement possible. Parce que les modifications apportées au texte par l'Assemblée nationale en 2ème lecture ne témoigne d'aucun désaccord sur la rédaction transmise par le Sénat. Et parce que cette proposition de loi reprend un combat que nous menons de longue date. Je vous appelle à soutenir ce texte sans modification et à l'adopter définitivement. Merci pour votre attention. Merci madame la présidente. La discussion générale étant Close. Nous allons passer la discussion du texte de la commission. Alors je vous rappelle la procédure les articles qui ne sont mis en discussion ne sont que les articles. qui n'ont pas été adopté conforme dans les 2 assemblées. Il n'y a pas d'amendement. Pas de demandes de prise de parole sur les articles en discussion. Je vais donc mettre aux voix l'article 1er et si vous en êtes d'accord, mais uniquement si vous êtes d'accord on considérera que le vote sur l'article 1er vos votes sur les autres articles récents en discussion. On y va comme ça. Alors j'ai mis au vote de l'article 1er qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté, les suivants sont donc également adopté je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Est ce qu'il y a des explications de vote, où est-ce qu'on peut considérer que c'était Très bien. Donc je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Elle est adoptée, je vais suspendre la séance quelques instants afin de permettre aux protagonistes du texte suivant de venir s'installer au banc. Merci Monsieur le Ministre.

La séance est reprise pour la discussion de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale a pris un engagement de la procédure accélérée et visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérive des influenceurs sur les réseaux sociaux et dans la discussion générale. La parole est d'abord madame Olivia Grégoire Olivia Grégoire pardon Ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat et du tourisme. Madame la Ministre c'est à vous. Madame la présidente, madame la présidente Prima. Madame la rapporte. Mesdames, messieurs les sénateurs. Il est très rare que nos débats législatifs toujours studieux, parfois fastidieux suscite autant d'intérêt sur TikTok et chez les jeunes que cette proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérive des influenceurs. Sur les réseaux sociaux. Nous allons en effet parler aujourd'hui d'un sujet qui est à la mode. Mais qui est en réalité un sujet qui dépasse la mode un sujet de toujours réguler la publicité. Un sujet qui mobilise mais aussi un sujet qui rassemble comme en témoigne l'adoption du texte à l'unanimité par l'Assemblée Nationale nous examinons donc aujourd'hui une proposition de loi qui attendu à la fois parce qu'elle vient combler un vide juridique. Un vide inhérent à l'évolution des technologies, mais aussi parce qu'elle vient d'une demande populaire et avec elle un questionnement sur cette évolution des technologies concernant le vide juridique, il est assez clair que la publicité a beaucoup évolué depuis l'époque où Sarah Bernard vanter les mérites d'un fer à friser, je vous rassure tout de suite cette publicité pour l'exposition du Petit Palais ne m'a donné droit a absolument aucun bénéfice économique ni avantages en nature, si ce n'est celui de vous la recommander la publicité a également énormément évolué depuis l'époque des lois Evin ou encore Toubon qui consistait comme vous le savez à réguler des annonceurs et des médias dont la publicité était le 1er métier. Aujourd'hui. N'importe quel individu croit pouvoir vendre ce qu'il veut comme il veut, d'où qu'il le veut. c'est bien cela qui pose problème et qui suscite cette demande populaire pour une meilleure régulation un meilleur encadrement. J'en veux pour preuve le succès en tout cas le l'audience de la consultation publique que nous avons à Bercy avec Bruno Lemaire sur le sujet. J'en veux pour preuve également l'abondance de témoignages de ces femmes, de ces hommes faisant part spontanément d'abus d'escroquerie parfois très graves dont ils ont été victimes et nous parlons ici de graves dangers, pas seulement financiers auxquels nos concitoyens se retrouvent exposé alors que le rapport individuel créé par Internet démultiplie les possibilités et complexifie les moyens de contrôle. Les services de l'État sont à l'oeuvre certes depuis des années, depuis que les pratiques des influenceurs se sont multipliées. Ainsi, la DGCCRF a déjà eu l'occasion de rappeler à l'ordre les contrevenants. Elle rendra d'ailleurs bientôt publics les noms de ceux une trentaine à ce jour, qui se sont livrés à des pratiques commerciales trompeuses. Pour autant, force est de reconnaître que les nouvelles facilités ouvertes par les réseaux sociaux demande impose même que notre droit se dote de nouveaux outils de la même manière que par le passé, le législateur à adapter son arsenal juridique pour adapter l'encadrement de la publicité aux nouveaux médias qui était alors la radio ou encore la télévision. C'est dans ce contexte. Qu'est née cette proposition de loi et je veux ici saluer le remarquable travail des parlementaires. D'abord celui des députés qui s'en sont saisis de façon transpartisane à l'Assemblée nationale. Ensuite des sénateurs dont la rigueur a déjà permis en commission de lever quelques doutes et de corriger les imperfections. J'ai à coeur que nous puissions aujourd'hui achevé ce travail dans le même esprit de dialogue, de concertation qui nous guide depuis plusieurs mois, depuis décembre dernier. Si l'on s'en tient à la consultation publique lancée par Bruno Lemaire et qui a recueilli les avis de plus de 400 professionnels et de près de 20.000 de nos concitoyens. Depuis bien avant. Si l'on regarde la persévérance avec laquelle les services de l'État et je veux ici encore salué l'action de la DGCCRF surveille le phénomène. Il me semble que nous arrivons dans ce texte à une définition équilibrée a une définition plus claire de ce que doit être l'influence commerciale, à savoir une pratique commerciale qui doit respecter aussi bien les principes généraux du commerce que l'encadrement de la promotion de certains biens et services. Nous prévoyons donc des règles spécifiques. C'est le cas de la chirurgie et la médecine esthétique, compte tenu de leur danger immédiat humiliant irréversibles sur la santé humaine. Nous aboutissons également un rappel nécessaire des droits mais aussi des devoirs qui s'applique à ceux qui exerce cette influence commerciale au même titre et strictement au même titre que l'ensemble des émetteurs et canaux de promotion et publicité à des sanctions dédié et adapté à ce cadre spécifique qui dit droit et de voir qui s'applique à tous et donc aux influenceurs dit aussi eux qui ne s'appliquerait qu'à eux-constituerait une rupture d'égalité difficile à justifier. Nous devons ainsi collectivement veiller à ne pas trop créer une publicité je dirais à 2 vitesses, avec des règles. Qui serait très très stricte, voire exagérément. Qui ne s'appliquerait qu'aux influenceurs et c'est une ligne à laquelle le gouvernement tient. Non pas par rigidité, encore moins par rigidité dogmatique mais au contraire par pragmatisme, tout le monde vous moi les influenceurs les annonceurs, les consommateurs. Tout le monde veut un cadre juridique clair et fort et pour que ce cadre soit fort, il doit être clair à l'abri de toute contestation litigieuses. Nous sommes donc ici pour adapter la protection du consommateur aux nouvelles formes de l'influence commerciale pas pour interdire les nouvelles formes de cette influence commerciale, nous ne créons pas d'entrave. Nous proposons de ce cadre découleront ensuite les outils déjà ou bientôt à notre disposition et sur lequel vous mesdames, messieurs les sénateurs avaient apporté des précisions nécessaires. D'abord des outils légaux comme les contrats écrits entre les annonceurs et les influenceurs et entre les agences et les influenceurs dont le gouvernement demandera avec vous la systématisation. Par ailleurs, des outils d'accompagnement comme le guide de bonne conduite des influenceurs présenté il y a quelques semaines maintenant par Bruno Lemaire et qui sera bien sûr actualisé à l'issue du vote de la loi, le gouvernement proposera durant cette lecture quelques modifications qui semble répondre au besoin de clarté de solidité surtout que nous partageons tous à l'aune du règlement Digital Services is acte le DSA, qui prévoit une meilleure régulation des réseaux sociaux et des activités qu'il génère. Je disais en préambule que nos débats a été particulièrement suivi par les plus jeunes. Je souhaite précisément conclure. En rappelant que cette proposition de loi ne doit pas être prise pour ce qu'elle n'est pas ce n'est pas une loi pour ou contre la publicité pour ou contre les jeunes ils loi qui définirait ce qui serait moral ou ne le serait pas. C'est une loi de régulation économique au service d'un métier naissant composé de personnes qui ont à coeur pour l'immense majorité d'entre eux de bien faire leur travail et c'est pas ce que nous voulons soutenir leur métier que nous soutiendrons évidemment cette proposition de loi de régulation de l'influence commerciale, je vous remercie. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui adopté à l'unanimité par la commission des affaires économiques. La semaine dernière vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérive des influenceurs sur les réseaux sociaux. Cette proposition de loi est importante car très attendu de nos concitoyens et c'est grâce à une initiative parlementaire transpartisane que cette demande populaire a pris la forme d'un texte de loi. Je tiens ainsi a salué les travaux des 2, rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Messieurs donc Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte, qui ont su collaborer pour aboutir à une initiative commune et concertée. Les premiers travaux parlementaires menées sur ce sujet nouveau pour les législateurs que nous sommes vont dans le bon sens et mérite d'être conforté. Ce sujet est nouveau car c'est la première fois en Europe qu'un texte de loi transversale visant spécifiquement à réguler l'activité des influenceurs sera adopté. Encore une fois les parlementaires français sont à l'avant-garde de la régulation de l'économie numérique. Et je ne vous apprends rien, on vous disons qu'ici au Sénat, il s'agit d'un sujet qui attire particulièrement notre attention et qui fait l'objet. De nombreux travaux. Ce sujet est nouveau car même si les influenceurs et les réseaux sociaux font des hommes désormais partie du quotidien de nos concitoyens. Ce secteur d'activité demeure peu documentée et mal connue des pouvoirs publics. Ainsi, selon les premières estimations à notre disposition, il y aurait 150.000 influenceurs en France, dont seulement 15% exercerait cette activité à temps plein. Ce sujet est nouveau également car il pose la question de l'adaptation de notre droit national de nos outils de contrôle et de régulation aux spécificités de l'économie numérique. C'est votre droit est suffisamment souple et robuste pour s'adapter à cette nouvelle forme d'activité commerciale nos outils de contrôle et de régulation mérite quant à eux d'être largement renforcé. C'est dans cet état d'esprit. C'est dans cet esprit que j'ai abordé mes travaux au sein de la commission des affaires économiques avec un seul objectif, mieux comprendre le secteur de l'influence commerciale sans aucun préjugé et adapter en conséquence la proposition de loi qui nous a été transmise enfin d'en améliorer la portée et l'effectivité. Je tient ainsi à remercier mes collègues pour avoir contribué à l'élaboration de ce texte collègues issus de tous les bancs de l'hémicycle, je tiens à le souligner et je ne manquerai pas de les citer lors de l'examen du texte. Ils ont permis à la Commission d'adopter un texte plus juste, plus ciblée et rééquilibrer. Pour définir ma feuille de route politique sur ce texte. Je me suis posé 3 grandes questions, la première celle de savoir si l'influence commerciale est une activité comme les autres. Si la question peut sembler un peu provocatrice. Il faut bien reconnaître un paradoxe, l'activité d'influence commerciale est désormais bien imbriquées au sein de notre économie présentant des avantages certains. Pour les entreprises mais nos concitoyens ont le sentiment que ce secteur demain demeure totalement dérégulé. Les mauvaises pratiques de certains acteurs mal intentionnés masque aujourd'hui la réalité d'un secteur en plein développement. Les difficultés de régulation du secteur de l'influence commerciale par les pouvoirs publics sont réelles d'abord en raison de la hausse du nombre d'influenceurs du volume de contenus publiés et du caractère de plus en plus éphémère de ces contenus jeta je parle notamment des stories des la, c'est-à-dire des Publications instantanée ou en Direct. C'est pourquoi il est apparu indispensable d'adapter les missions des autorités de régulation en renforçant, par exemple les pouvoirs de police administrative de la DGCCRF ou encore d'étendre la procédure de blocage judiciaire de l'Autorité des marchés financiers aux promotion d'offres illicite. Ensuite parce que de très nombreuses publications touchant un public français sont émises par des influenceurs français résidant en dehors de l'Union européenne, notamment aux Émirats arabes unis et aux États-Unis alors même que leur notoriété s'est construite auprès de ce public. Il m'a semblé indispensable de rattacher ces influenceurs à la proposition de loi que nous examinons en maintenant le principe de soumission au droit français des contrats d'influence commerciale et en leur imposant de désigner un représentant légal établi sur le territoire de l'Union européenne et ce afin de faciliter la coopération avec les autorités administratives et judiciaires nationales. Les travaux de la commission des affaires économiques ont permis de poser les jalons les premiers jalons d'un dispositif que je vous proposerai de conforter tout à l'heure pour démontrer à nos concitoyens que l'activité d'influence commerciale. Peut être une activité économique comme les autres, nous devons donc renforcer son contrôle sa régulation et son encadrement. Je me suis posé également une 2ème question celle de savoir si l'influence commerciale. Et es un canal publicitaire pardon comme les autres. C'est sans doute sur ce point que le sujet sur lequel nous des des bâtons n'est pas si nouveau, devons-nous appliqué aux influenceurs les mêmes règles, interdictions encadrement que celles existantes, par exemple pour la télévision, la radio ou les plateformes de partage de vidéos. Contrairement aux idées largement exprimé ces derniers temps l'activité d'influenceurs n'est pas totalement dérégulé toutes les règles existantes aujourd'hui en matière de publicité et de promotion s'applique aux influenceurs, nous devons le rappeler. En revanche, nous devons reconnaître que ces règles ne sont aujourd'hui pas connue, mal comprise et non respecter pas connu et mal comprise. Car il n'y a pas de formation de diplôme ou de certification obligatoire pour devenir influenceur ou agent d'influenceur. Mal appliquée car il y a aussi des abus intentionnel de la part de certains influenceurs et de certains annonceurs, d'ailleurs semble pardon donc important avant d'interdire et de sanctionner davantage de commencer par faire preuve de pédagogie à l'égard des acteurs du secteur de clarifier les règles du jeu, afin d'accompagner un secteur qui doit encore se structurer. C'est notamment pour cela que nous avons voté en commission l'affichage obligatoire de la mention unique publicité sur les publications commerciales des influenceurs. Nous avons également voté l'affichage obligatoire de la mention images virtuelles afin d'anticiper les conséquences de l'Intelligence artificielle sur la publicité en ligne et le marketing d'influence dans tous les cas, les objectifs de ces mentions sont les mêmes, faire preuve de davantage de sincérité et de transparence à l'égard des internautes et des consommateurs. Une fois le caractère commercial d'une publication clairement identifiés. Nous devons déterminer les propos promotion réalisées par les influenceurs qui mérite d'être autorisé interdite ou encadrer la commission a donc souhaité. Rééquilibrer les dispositions votées qui concernent les secteurs de l'agroalimentaire du commerce en ligne et des crypto-actifs. Un durcissement excessif des dispositions votées sur ces 3 sujets risquerait d'avoir des effets de rebord de bord pardon. Indira indésirable par ricochet sur le bon fonctionnement de notre économie. Un pan global qui ne doit pas être pénalisé par une proposition de loi visant spécifiquement l'influence commerciale. L'influence commerciale est ainsi à la fois un canal publicitaire comme un autre mais avec des spécificités, nous devons donc être prudent et ne pas adopter des dispositions trop contraignantes pour notre économie mais en même temps être vigilants au regard des conséquences spécifiques sur notre santé publique et notre jeunesse. 3ème et dernière grande question que je me suis posé sur les dérives de l'influence commerciale. Précisément de quelle dérive parle-t-on spécifiques sont tout à fait. Justifiée en matière de protection de la santé publique. En plus de l'interdiction de promotion de la chirurgie esthétique. La commission a souhaité interdire toute forme de promotion incitant directement ou indirectement à l'abstention thérapeutique au profit de la consommation de biens ou services présentés comme substitut à préférable comparables un traitement médical. Au regard de la hausse des dérives sectaires, sur les réseaux sociaux. C'est indispensable en matière de protection des enfants et des adolescents. La commission a souhaité également renforcer le régime d'informations portant sur les promotions de jeux d'argent et de hasard en obligeant les influenceurs à afficher un bandeau interdit aux moins de 18 ans. Il s'agit ici de sensibiliser à la fois les internautes, mineurs qui contournerait les systèmes déclaratifs de vérification d'âge mais aussi leurs parents et leurs familles. en matière de protection des consommateurs et des épargnants. La commission a souhaité être à l'écoute des collectifs de victimes et interdire la promotion d'abonnement à des pronostics sportifs au regard des grands événements sportifs à venir le risque d'arnaque est particulièrement élevé. Voilà donc mes chers collègues. Notre feuille de route pour l'examen de cette proposition de loi, vous l'aurez compris, l'objectif n'est pas tant d'interdire l'influence commerciale mais d'encadrer son développement afin de ne pas sanctionner de 2 sanctionné pardon que les acteurs mal intentionnés qui déciderait. Malgré cette proposition de loi de ne pas respecter le cadre légal. Je vous remercie. Merci la parole dans l'addition générale et d'abord. Monique de Marco pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi bien venues tendant à encadrer l'activité d'influenceurs. Ce texte répond en effet à une réelle nécessité de structuration et de régulation de ce secteur en pleine expansion. Afin de mieux définir les contours et les enjeux de ces nouveaux métiers issus des réseaux sociaux. Des youtubeurs au streaming de switch en passant par Instagram et TikTok, on compte en France 150.000 créateurs du contenu. Selon l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, je cite, une filière qui peut être créative, inventive, mais dans laquelle la place proéminente de la publicité de la consommation, nous oblige à agir pour enfin créer un cadre légal car l'autorégulation des acteurs ne suffit pas et l'audience est souvent constitué d'un public jeune et influençable qu'il faut protéger, Parmi ces influenceurs une part certaines ne respectent pas la législation en vigueur en matière de publicité, souvent par méconnaissance des règles existantes et une minorité utilisent leur notoriété pour tromper le consommateur avec des pratiques qui peuvent être dévastatrices, notamment en matière de santé publique. Certains exemples sont à Téhéran. C'est pour quand. Pourquoi il convient d'agir pour permettre un développement responsable cette filière adapté à la réalité économique et poser un cadre de référence pour protéger influenceurs comme consommateur. Ce texte entend tout d'abord inscrire la définition d'influenceurs commercial dans le code de la consommation et du commerce. Il s'agit là d'une première Pierre qui devra nécessairement s'adapter. Compte tenu de l'évolution constante du secteur. Nous aurons un amendement pour mieux ajuster cette définition. Nous soutenons les autres points importants du texte sur l'encadrement et l'interdiction de certaines promotions, bien qu'elle n'aille à notre goût, pas assez loin sur la contractualisation entre influenceurs son agent et l'annonceur sur la régulation des plateformes numériques et l'aspect éducatif. Si la commission. Certains aspects du texte un adoptant par exemple l'interdiction de la vente et l'offre promotionnelle d'un produit en échange d'une inscription à une formation professionnelle ou bien l'encadrement de la promotion du contrat d'abonnement. Elle reste en deçà de son que nous souhaitons sur d'autres plans. Nous estimons qu'il faudrait être bien plus exigeants sur des interdictions de promotion et d'ajouter d'autres catégories de produits qui n'ont clairement pas leur place dans des discours publicitaires à destination de jeunes publics je pense à particulier aux produits amincissants aux produits pharmaceutiques aux produits alimentaires et boissons trop riches en sucre en sel ou en matière grasse ou encore aux jeux d'argent et de hasard. La commission a également actée quelques reculs dommageables qui mettent à mal l'ambition somme toute mesurée du texte initial. Je pense principalement aux dispositions supprimées visant à mieux encadrer la promotion des produits alimentaires particulièrement néfaste pour la santé. Nous constatons que là aussi le dogme de la croissance économique et la défense de l'industrie agroalimentaire pas ça va la santé nutritionnelle de nos enfants. À l'heure où les maladies liées à la malbouffe atteignent des niveaux record. Rappelons que la France, contre 4 millions de diabétiques et 47% des Français sont en surpoids. Donc à 17% d'obèses. Nous ne pouvons nous passer d'une ambition plus forte sur ce sujet. J'en viens à l'autre enjeu majeur que soulève ce texte le renforcement des moyens budgétaires et humains à la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. Il s'agit là bien d'un débat à avoir, cette année encore dans le prochain cadre du projet de loi de finances. Si les moyens de contrôle ne sont pas là. Nos voeux d'encadrement du secteur resteront pieux. Acte donné que cette année la droite sénatoriale votera favorablement les amendements renforcent ne drastiquement les crédits affectés à la mise en oeuvre de leurs mission toujours plus nombreuses. Nous serons vous le rappeler. Les 15 agents annoncée récemment par le ministre de l'économie pour former, je cite, une brigade de l'influence commerciale. Ne seront clairement pas suffisant. Pour conclure ce texte aurait pu être davantage ambitieux notamment pour interdire la publicité de plus du produit on et des pratiques dont on connaît la nécessité la nocivité pardon, surtout pour les produits les les publics les plus vulnérables. Devrons-nous encore longtemps sacrifié la santé des publics les plus fragiles au nom de la sacro-sainte croissance économique. La collectivité devra-t-elle encore longtemps assumer des coûts exponentiels du traitement du diabète et des maladies cardio-vasculaires. La surconsommation encore de beaux jours devant elle. En 2023, c'est pour le moins désolant. Ce texte acte malgré tout des avancées pour de nombreux points ces nombreux. C'est pourquoi nous voterons pour. Je vous remercie. Et la parole est maintenant à Jean-Baptiste Lemoyne pour le groupe du Rassemblement démocratique progressiste éteint et indépendant. madame la présidente, madame la Ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, même la rapporteure mais mes chers collègues. Que de chemin parcouru en en 10 ans. Oui, c'était en 2013 précisément, que le célèbre non mais à l'eau quoi prononcée par Nabilla Vergara s'est répandue comme une traînée de poudre sur Internet la propulsant à des sommets de notoriété et 10 ans plus tard. Mesurer que l'intéressé en est à 9 millions de personnes qui la suivent sur Instagram. 9 millions de personnes c'est juste deux fois et demie. Plus que le président de la République et c'est juste 140 fois plus que l'Instagram de notre vénérable institution le Sénat. Ce sont des ratios donc qui interpelle. Et qui monte que lorsque l'intéressé fait la promotion de services boursiers sur Snapchat, sans mentionner qu'elle était rémunérée pour cela. On imagine le rôle que cela a. Dans la souscription de ces produits, d'où d'ailleurs une amende prononcée par la DGCCRF. En 2021, pour pratiques commerciales trompeuses. Alors on voit bien avec cet exemple que on ne parle pas d'une feuille vierge. Il y a eu un dévoiement. Il y a eu une sanction mais il y avait un besoin impérieux. De préciser des définitions de renforcer les sanctions de travailler aussi sur l'éducation et c'est d'ailleurs tout l'objet du travail qui était conduit par les députés. Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte avec cette proposition de loi transpartisane qui nous est soumise et je veux saluer dans le même temps parce que les initiatives ont été convergentes se sont. Renforcés confortés également le gros travail de concertation menée par le ministère de l'Économie. Et des Finances avec naturellement Bruno Lemaire Olivia Grégoire. pas loin de 20.000 contributions 400 professionnels qui ont également. Contribué et tout cela a permis. Eh bien je crois de cheminée de trouver un équilibre. C'était important de trouver cet équilibre parce que vous l'avez vu notoriété plus algorithmes dans la société, qu'on connaît. Cela peut faire un, un mélange détonant. Alors comment rappeler à la fois aux 150.000 influenceurs français leurs devoirs et à tous nos compatriotes leurs droits, les droits qui sont les leurs, en tant que consommateur, c'était l'équation que la proposition de loi transpartisane souhaite résoudre alors quelques points peut être la définition de l'influence commerciale, elle a été. été. Ajustée à la fois à l'Assemblée nationale en séance à la fois par la commission des affaires économiques. Je crois qu'on, on atteint là désormais un bon équilibre avec justesse avec clarté il faut saluer également le fait que la définition de l'agent d'influence est également. Été posée avec une responsabilité solidaire ensuite 2ème point de nos travaux, ça a été celui des outils pour encadrer cette pratique. Alors il y a naturellement un certain nombre de. D'outils qui sont d'ordre général, je pense aux directives européennes sur la vie privée sur les communications électroniques sur les pratiques commerciales déloyales dans le marché intérieur. Ou bien des textes, relevant d'interdictions sectorielles de la publicité mais on l'a vu ce cadre était mal connu, méconnu parfois inadapté était donc très important que nous puissions. Ajuster des dispositifs et il était nécessaire que les contrats écrits soit obligatoire pour lier les influenceurs les agences les annonceurs ainsi que le Sénat l'a décidé, il était nécessaire également d'avoir une vraie responsabilisation des plateformes en ligne avec. Clairement une coopération accrue de la DGCCRF important aussi de la conforter cette DGCCRF en terme de prérogatives par les pouvoirs d'injonction prévues par le texte par les moyens complémentaires effectivement il est très important que cette direction soit conforté dans son action. Alors on pourrait se dire, mais toutes ces. Comment dire. Toutes ces mesures, toutes ces contraintes. Ne vont-elles pas. Hé bien avoir raison du secteur, je crois que. Il faut avoir en tête que on a là une véritable activité économique qui s'est structurée qui doit pouvoir se développer mais se développer avec des règles claires. C'est pas un secteur à part, c'est un secteur à part entière. 40 millions de nos compatriotes ont fait des achats en ligne. Chaque année, et d'ailleurs je sais que le. Le ministère est très attentif aux risques de de commercialisation et de ce point de vue là un certain nombre de travaux ont été enclenché à la suite des états généraux du commerce. Il était important, hé bien de rappeler que. Un certain nombre d'obligations incombant aux activités de promotion et de publicité. De façon générale s'appliquer à l'influence commerciale et puis nous avons renforcé les mesures de protection en matière de santé publique vis-à-vis des mineurs. Je pense à la chirurgie esthétique soit. À l'abstention thérapeutique également aux produits financiers et tout cela fait que, hé bien nous espérons que la protection des consommateurs sera réelle avec une relation commerciale de confiance entre les influenceurs leur public, les mentions publicité lorsqu'ils prennent la parole de cette façon-là nous sommes tout à fait justifiée. Avec une meilleure information des influenceurs grâce au guide des bonnes pratiques qui va être actualisé une mise à jour il y a besoin de de connaissances. Quand on voit 60% des 50 influenceurs. Permet si qui ont commis un certain nombre d'infractions. Hé bien on doit progresser. De ce point de vue-là et puis naturellement la démarche éducative hé bien le citoyen soit éclairé lorsque. Il est, il consomme voilà quelques points. Mes chers collègues. Madame la ministre madame la rapporteure sur lesquels le groupe RDPI. Voulait attirer l'attention. Accompagné protéger. Et voilà ce que cette fois propose cette oeuvre utile que de la voter, nous la voterons et merci encore à toutes celles et de ceux qui ont permis ce progrès en l'écrivant noir sur blanc dans la loi. Merci à vous. Et la parole est maintenant Rémi Cardon. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente. Madame la ministre, madame la présidente Prima. Madame la rapporteur, mes chers collègues. Avant de débuter plus en détail mon propos. J'ai évidemment une pensée pour Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta pour le travail qui a été accompli ces dernières mois et qui prouve. Qu'une loi. Étaient et sont nécessaires et essentielles pour réguler le Far-West, de l'influence. Que parfois les propositions de loi peuvent traverser tous les clivages politiques. Dans le cadre de nos débats j'en profite d'ailleurs pour remercier madame la rapporteure qui a suivi cet esprit au Sénat. Et pour preuve une dizaine d'amendements présentés par mon groupe ont été satisfaits en commission. manifeste manifestement que cette proposition de loi porte un sujet crucial pour notre société et son adoption et son d'option pardon pourrait avoir un impact significatif sur notre économie en plein boom, l'économie justement de l'influence commerciale. Le marché mondial du marketing d'influence est en pleine croissance et il atteint 15 milliards d'euros en 2022, en hausse de près de 20% en un an Difficile de connaître précisément le montant de ce marché, puisqu'il ne figure pas dans l'Observatoire de l'ePub qui conserve son à l'issue aux recettes des médias et des supports numériques pourtant. Les Français passent en moyenne 1h46 par jour sur les réseaux sociaux, un tiers des Français déclare d'ailleurs suivre des créateurs et des créatrices de contenu et ce chiffre culmine à 63% pour les 18 34 ans. Surtout c'est la relation nouée avec le créateur de contenus qui interpelle. Parmi les personnes qui suivent les influenceurs 61% approuvent de la sympathie. Pour eux en particulier. Et même des sentiments plus engagé comme la confiance à 43% et l'admiration à 41%. Apporter au monde de la publicité, les créateurs de contenus représente donc un puissant levier d'achat pour les annonceurs. Cependant, malgré leur influence croissante il y a des préoccupations légitimes. Quant à la matinée à la matière et à la manière dont certains d'entre eux ont décidé d'opérer pour en faire une rémunération principale. Il y a de nombreux cas d'influenceurs faisant par exemple à la promotion de produits dangereux ou trompeurs. Ou en ne respectant pas certaines règles éthiques déjà existantes dans le code de la consommation notamment je citerai par exemple Dylan Thierry qui cumulent plusieurs millions de followers, et qui est accusé de pratiques frauduleuses. Avec le dropshipping de publicité mensongère ou plus près ou plus récemment de tentative de trafic d'enfants. À ce titre, le collectif eux à vie a notamment été précurseur dans la lutte contre ces pratiques frauduleuses et dangereuses. Vous l'aurez compris. Il est temps pour nous parlementaires de prendre les mesures nécessaires pour encadrer cette activité et protéger les consommateurs. Cette proposition de loi vise à atteindre cet objectif de plusieurs manières. Tout d'abord. Elle propose de clarifier les règles. Régissant la publicité sur les réseaux sociaux les influenceurs seront tenus de divulguer clairement les partenariats publicitaires et les promotions via leur contenu qui réalise. Dans cette optique. Nous souhaitons. Aller beaucoup plus loin en créant un badge influenceurs qui permettrait aux créateurs de contenus de s'afficher en tant que telle en tant que telle auprès des des utilisateurs par souci de transparence et par volonté de faciliter le travail des autorités compétentes en charge de la régulation de l'influence commerciale. Les personnes relevant de l'influence commerciale devront également respecter certaines normes éthiques telles que l'interdiction de promouvoir des produits dangereux et illégaux. La proposition de loi rappelle à juste titre des interdictions déjà en vigueur pour la publicité à la télé à la radio. Il s'agira pour notre groupe de répondre aussi à d'autres pratiques douteuses comme l'usage détourné de certains médicaments. Vous en avez peut-être entendu parler. Mes chers collègues. Le cas de l'Ozempic par exemple. Ce qu'Allah est alarmant, c'est de ce, ce médicament anti-. Diabétique est détourné par. Par plusieurs personnes pour mincir ah a justement à cause de recommandation de ce produit sur TikTok. L'engouement autour de ce médicament a entraîné une crise sanitaire puisque des laboratoires se sont retrouvés en rupture de stock. Alors que des personnes diabétiques dépendent vraiment de ce traitement. Nous espérons donc que le texte pourra évoluer. Afin de stopper ces pratiques dangereuses qui nuisent à la santé publique. Ensuite. Concernant l'exercice d'une activité d'influence commerciale. Nous souhaitons avec le groupe socialiste être. Des points de vigilance. Parce que à l'âge de 11 ans, plus de la moitié des enfants sont déjà présents sur les réseaux sociaux. Un chiffre qui dépasse un peu, un peu plus de 70% pour les ados de 12 ans. Un âge où il est encore difficile de distinguer. Un contenu publicitaire et de prendre du recul sur la relation que l'on a avec l'influenceur con ce que l'on suit. C'est pourquoi. Nous souhaitons aller plus loin que les dispositions actuelles du texte en interdisant par exemple aux créateurs de contenus. Adultes Adultes de faire la promotion de la malbouffe auprès des mineurs et ce afin de ne pas générer et ne pas générer une génération TikTok jusqu'à la génération Mc Donald 2.0. Aussi, cette proposition de loi instaure un mécanisme de surveillance pour garantir le respect des règles. Les autorités compétences compétentes seront chargés de surveiller les influenceurs et de prendre des mesures en cas de violation des règles éthiques. hein. Pour pour aller justement de l'amende à la suspension temporaire ou permanente même des comptes de l'influenceur. Ce travail a déjà commencé et ça a été dit par Madame le Ministre puisque le ministre de l'Économie a annoncé mercredi dernier que la DG. CRF avait contrôlé presque autant d'influencer en en trois mois que sur l'année 2022. 60% des influenceurs contrôlé soit. 30 sur 50 ont fait l'objet de 2 constats d'infraction. Ce qui monte de choses. La nécessité de premièrement la nécessité de réguler plus fortement cette activité. Deuxièmement, la nécessité de renforcer les moyens de contrôle. Au rythme de 50 influenceurs contrôlée par trimestre. Il faudrait toutefois 750 années pour contrôler l'ensemble des 1500 influenceurs reconnu en France. En sachant que la brigade de la DGCCRF est composée de 15 personnes. À Nogent peut donc. Être en charge, potentiellement, je dis bien de 10.000 influenceurs à lui tout seul. Ce n'est pas acceptable. Cela représenterait un travail titanesque surtout. Que pour constituer ses dossiers. Les enquêteurs doivent collecter les preuves et les identités ce qui est une mission parfois impossible. Le manque de moyens, de moyens est criant et j'alerte Madame la Ministre une nouvelle fois. Cette proposition de loi vise donc à réguler l'activité de l'influence commerciale et nous devons dès à présent, espérer que les moyens de l'État suis vont suivent. Et que la loi puisse exercer son son plein potentiel. Et surtout que d'ailleurs les tweets de du ministre de l'économie ne soient pas justement des, des coups de com. Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincus avec l'ensemble du groupe socialiste, écologiste et républicain que cette proposition de loi est nécessaire. Pour protéger les consommateurs et garantir les influenceurs agissant justement de manière responsable et éthique et respectueuse de leur public. Il est également nécessaire de souligner que cette proposition de loi ne vise pas à restreindre la liberté d'expression ou la créativité des influenceurs. C'est la raison pour laquelle je tiens à rassurer les influenceurs signataire d'une tribune parue dans le JDD. Juste avant la, l'examen du texte à l'Assemblée. vous souhaitez que notre seule boussole soit la protection des consommateurs des dérives d'une minorité qui se croient tout permis. Je peux vous assurer que ce texte il répond. Pour conclure. Je suis convaincu que cette proposition de loi est une étape afin de Peseux de poser les premiers jalons de la régulation commerciale. Même si je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire parce que j'ai des craintes sur la mise en application de ce texte notamment avec les moyens humains air je l'ai dit, il faudra renforcer les moyens. Et j'espère que le midi le les 15 TP vont augmenter a plu à plutôt à 50 ETP dans les prochaines années. Merci. Merci. La parole. Et maintenant à Fabien Gay pour le groupe républicain communistes, écologistes.

Madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure, mes chers collègues. Les métiers de l'influence. Voici l'exemple type. D'une activité qui s'est développé à vitesse grand V sans que le pouvoir politique ne s'en saisisse car elle n'a pas vu venir son émergence et mesurer son importance. Vous me direz qu'il est difficile. De réguler une activité récente qui vient d'apparaître, c'est vrai. Mais aujourd'hui. Vu l'ampleur du phénomène qui se chiffrent à plus de 150.000 influenceurs. Qui agissent sur tous les réseaux sociaux et regroupe des agents économiques de différents ordres. Il est temps de mettre fin au Far-West. Car qui dit nouvelle. Activité économique dit évidemment que beaucoup le font en bonne intelligence mais qu'il existe aussi des abus voire des escroqueries. Pour empêcher ces dérives. Il ne servirait à rien d'interdire des partenariats rémunérés aux influenceurs, ce serait une aberration mais surtout même si on le voulait. On ne le pourrait pas. Donc ni moralité, ni interdiction mais bien régulation et encadrement. Il faut poser des règles et cette proposition de loi va dans le bon sens. Alors pourquoi des règles parce que ce sont des agents économiques qui s'adressent principalement un public jeune, âgé de 15 à 25 ans très influençable et qui parfois façonne à travers eux, leur vision du monde de leur corps ou encore des espoirs de devenir riche en quelques clics. Certains influenceurs sont drôles d'autres cuisine d'autres jouent aux jeux vidéo et certains sont payés pour placer des produits ou des voyages. Nous regardons de la publicité sur tous les écrans. Et ce n'est pas interdit. Mais cela ne doit pas nous empêcher à continuer à dénoncer la société de consommation qui ne peut être le seul horizon offert à notre jeunesse. Alors. Il faut bien sûr pouvoir avertir le fond loueur que c'est une publicité. Mais l'affaire se Corse lorsque l'influenceur parle de cryptomonnaies. De copies Trading qui l'incite à parier. Qu'ils vendent des produits aux beautés frelatées ou fait la promotion de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Et c'est la même chose avec l'incitation à la chirurgie esthétique. Car au moment de l'adolescence où les complexes sont nombreux. L'espoir de ressembler aux standards de beauté que nous voyons partout et qui s'impose comme un modèle à suivre, peut avoir des conséquences très graves. Oui, dans un certain nombre de domaines, il faut interdire l'Exposition de nos jeunes adolescents voire préadolescents à des produits qui peuvent soit les isoler socialement soit les maîtres mal dans leur peau, soit les ruiner soit mettre leur santé en danger car contrairement à la publicité. L'influenceur nous un lien amical et le jeune veut lui ressembler et limité et donc le tort peut aller beaucoup plus loin qu'une simple publicité que nous regardions à l'époque du Club Dorothée. Pour ma génération. Il est donc logique que nous définissions pour la première fois ce qui est un influenceur ou une influenceuse mais aussi un agent d'influenceur pour le Laurent solidaires et que les deux soient sanctionnés. Lorsque la promotion d'arnaque et constater comme par exemple les influenceurs qui font la promotion de sites d'arnaque au compte personnel de formation, il faudra vraisemblablement aller plus loin. La prochaine fois. Et offrir aux influenceurs un véritable statut, au même titre que les mannequins et journaliste pigiste dans le livre 7 du code du travail pour permettre au code de la consommation de protéger leur public mais aussi pour permettre aux influenceurs de se protéger face à des contrats qui pourraient les exposer et qui dit loi dit encadrement dit sanction éventuelle la police dans ce domaine, c'est la Dgccrs. Même si on ne règle pas cette question avec une loi même un projet de loi, madame la ministre, il faudra que nous ayons le débat lors du projet de loi des finances qui arrivera en fin d'année et il faudra se battre pour obtenir des moyens supplémentaires car aujourd'hui, seulement 10 agents sont affectés aux activités d'influence sur les 1800 et je pense que toutes et tous, ici, nous pouvons dire, c'est largement insuffisant. La communication c'est bien comme l'a fait Bruno Lemaire en annonçant l'ouverture d'une enquête sur 50 influenceurs mais les 30 infractions révélées montre bien qu'il faudra mettre les moyens humains pour faire appliquer la loi et 50 influenceurs contrôler sur plus de 1150 1000 c'est évidemment une goutte d'eau. Nous en conviendrons toutes et tous. Enfin je voudrais finir par là, il nous faudra avoir un débat avec les influenceurs et notamment les plus connus, qui sont tous résidant à Doha, Dubaï ou Abou Dhabi. On sait que pour une Story Instagram, il vaut mieux le soleil éclatant de ces villes du Moyen-Orient plutôt que les paysages pluvieux très joli comme le chantait Jacques Brel, mais moins vendeur comme chacun le sait. Parce que ce sont surtout les taux d'imposition qui avoisine les 0% qui les attire, là-bas au même titre que pour les évadés fiscaux. Il faut leur dire une chose, lorsqu'on fait du Business en France, on paye ses impôts en France, voilà qui sera en tout cas un très bel exemple à donner à notre jeunesse. Je vous remercie. Madame la présidente, madame la Ministre. Madame la rapporteur se ramène, mes chers collègues. La semaine dernière, nous avons adopté en commission à l'unanimité la proposition de loi encadrant les influenceurs sur les réseaux sociaux et ce de manière équilibrée. La place prépondérante des réseaux sociaux a conduit à l'émergence des influenceurs nouveaux acteurs économiques dont l'activité consiste à produire des contenus numériques. Qui visent en général à promouvoir des produits ou services moyennant rémunération. Il pourrait s'apparenter à des vendeurs de téléachat. 2.0. Léna situations où se cuise, ils sont en quelque sorte les versions 2023 de Maryse Corson et de Pierre Bellemare. J'espère que certains s'en souviennent. Il s'agit ainsi de nouvelles activités économiques et de nouveaux vecteurs de diffusion et pourquoi pas. On entend souvent le bruit médiatique de celle qui vend l'eau de son bain, mais on découvre aussi des vulgarisateur de connaissance des humoristes ou des développeurs personnels tels que Hugo décrypte les adorable ou science étonnante. Près de 150.000 influenceurs actif sur les réseaux sociaux français touche entre 17 et 52 millions d'utilisateurs en France avec des revenus très disparates. 29% des créateurs de contenus gagnent moins de 5000 euros par an. Beaucoup de ces nouveaux entrepreneurs se Servent donc de leur expérience numérique. Comme d'un tremplin vers d'autres métiers journaliste animateur photographes ou que sais-je. Ne s'agit pas de tuer le potentiel économique de ces jeunes chefs d'entreprise, ils doivent, comme toute entreprise classique trouver leur marché. Par former leur savoir-faire et progresser. Mais comme toute entreprise, ils doivent respecter les lois. Or l'action de certains influenceurs est porteuse de dérives. Parmi lesquels des escroqueries diverses publicités mensongères ou clandestine, fraude, contrefaçon et des incitations des conduites à risques paris en ligne régime alimentaire drastique chirurgie esthétique et cetera. Sachant que l'essentiel de leur audience est constitué de mineurs et de jeunes adultes 40% entre 15 et 24 ans. Il est salutaire de mettre des garde-fous pour protéger les mineurs pour garantir la santé des consommateurs. Rapporteur l'année dernière d'un rapport sur l'information du consommateur. Il me paraît essentiel de cadrer des publications des influenceurs pour qu'elle satisfasse l'intérêt des acheteurs en toute transparence afin qu'ils sachent par exemple qui sont face à une publicité. Attaquer la nouvelle économie. Cette loi permet de réguler les réseaux sociaux et ça, ce qui est dans la définition d'un modèle européen du numérique. Alors ou sont en train de s'appliquer en 2023 et 2024. Les directives européennes DSA. Emma se présent texte propose une originalité à la régulation des influenceurs et réseaux sociaux. Face à un modèle américain ou la responsabilité de la régulation est totalement dévolue aux entreprises privées. Face à un modèle chinois ou russes, qui contrôlent à outrance les publications numériques sur leur territoire. L'Europe et la France offre un modèle responsable et protecteur pour les usagers, notamment les mineurs tout en conservant la liberté des influenceurs de créer et de faire du Business. Permettez-moi néanmoins de rappeler ce que je dis à chaque rapport budgétaire, ce que nous avons répété dans le rapport d'information du consommateur. Madame la Ministre, il faut des contrôles de la DGCCRF pour faire appliquer la loi et pour cela il faut recruter des personnels plutôt que de refaire une autre loi dans quelques années. Le groupe Union centriste votera favorablement cette loi équilibrée et responsable et je vous remercie.

Madame la présidente. Madame la ministre. Madame la rapporteure chers collègues dans un 1er temps saluons cette initiative parlementaire transpartisane et remercions les auteurs de cette proposition de loi qui va permettre, si elle est votée pour la première fois en Europe d'élaborer un cadre légal à ces nouvelles pratiques commerciales fréquemment douteuses qui envahissent les réseaux sociaux. Le législateur a une grande responsabilité, parce qu'il lui appartient de protéger les consommateurs des dérives de ce qu'on appelle les influenceurs. Entre ceux qui proposent de gagner de l'argent d'un coup de baguette magique par des jeux de hasard. Celles qui vendent les services de chirurgie plastique et esthétique et se promettant de guérir de. D'un cancer via une pilule miracle. Nous prenons conscience que ce milieu peut aller trop loin et mettre en danger, non seulement les consommateurs, mais aussi la jeunesse, 87% des adolescents âgés de 11. Et 12 ans utilisent les réseaux sociaux. Ce sont surtout les jeunes qui sont les premières victimes du marché de l'influence parce que perméable aux contenus qui vendent les nouveaux standards de beauté corps ultra musclée body lifter lève le fil pulpeuse etc. Les influenceurs s'invite dans notre foyer sans que nous puissions les déloger de nos téléphones en 2021 la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression indique que six influenceurs sur 10 ne respectent pas la réglementation en vigueur sur la publicité et les droits des consommateurs parce que oui les influenceurs sont déjà soumis au respect des règles existantes en matière de publicité. Selon la dernière étude Médiamétrie. Nous passons environ 2h par jour sur internet, il est de notre responsabilité de réguler ce qui s'y passe de donner les outils juridiques nécessaires pour. Encadrer sanctionnés et retirer s'ils le font les contenus en ligne susceptibles d'influencer les plus jeunes et les plus vulnérables d'entre nous. Ce texte de loi n'est pas là seulement pour les prix mais, mais avant tout pour prévenir et protéger les créateurs honnête de contenus. Ainsi professionnel de l'influence agences annonceurs mais aussi plateforme auront enfin un cadre légal de référence, avec un renforcement des sanctions en cas de non-respect protéger les Français doit être notre seule ambition est notre principale préoccupation, il y a des sujets sur lesquels les désaccords sans grand mais il y a aussi et c'est le cas aujourd'hui des débats qui font l'unanimité. Je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre. Madame la rapporteure, Toute influence est immoral influencer quelqu'un c'est lui donner son âme Et si cela peut choquer certains d'entre nous qui ne comprennent pas cet engouement généré par plusieurs milliers d'influenceurs l'image et la notoriété se monnaye désormais. Mais un État honnête cela n'est pas nouveau depuis des décennies, les acteurs, les sportifs 3 au-delà de leur art et de leur discipline en jouer de leur image via des publicités. c'est un Eicher personne au connus ou des anonymes devenus célèbres sous un à la téléréalité ont emboîté le pas. Mais et c'est toute la différence, leurs médias ont changé il utilise des vecteurs nouveau peu. Et qui méritent de l'être. Nous examinerons d'ailleurs très prochainement une proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine. Ah ligne. L'activité de l'influence du commercial méritait de sortir de l'opacité. Surtout avec les chiffres posé par la commission des affaires économiques. Près de 150.000 influenceurs en France et 87 contrôles de la DGCCRF depuis 2022. Ce texte ne veut répondre à ces enjeux de clarification en offrant un cadre à une activité qui est devenue une profession et dont les rémunérations sont au sommet pour certains. Depuis qu'il a été monétiser avant il s'agissait d'davantage ânes nature et de cadeau ce secteur nécessite d'abord une définition de l'activité et un rappel de la loi. Car certains des règles de base de commerce et de la publicité. Les évacuations doivent évidemment également appliquer des dispositions législatives concernant les mineurs, les jeux d'argent. La loi Évin, les secteurs très variés, qui a rejoint aujourd'hui la RTS concerne tous des animaux de compagnie à la santé, rien n'échappe aux influenceurs qui ont tous, tous ont pris de notre société de consommation. Si nous pouvons nous interroger sur ces évolutions nos états d'âme n'ont pas de place dans nos débats, seule la protection du public fragile. C'est-à-dire dans le secteur de l'influence soit les mineurs et les jeunes et le respect du droit doivent opprimé et nous guider. J'ai proposé à mon groupe RDSE amendement pour rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale car la commission des affaires économiques ne mentionne que les communications à titre onéreux, ce qui exclut les avantages à nature. Or ces derniers qui peuvent être très fréquents et très conséquent d'doivent être expressément prises en compte en étant considéré comme une rémunération un montant minimal des avantages ânes nature serait fixé par décret par exemple 150 euros comme c'est le cas actuellement pour les parlementaires les d'après et de représentants d'intérêts. D'où la nécessité de contrat clair entre les parties. Le commerce d'influence à Paris aujourd'hui complètement intégré dans les stratégies marketing qui passait souvent jusqu'alors sous les radars. Je porte également 2 amendements pour accroître la responsabilité. L'un d'entre eux étant les interdictions et donc des sanctions applicables en cas de violation de ces interdictions aux personnes physiques ou morales qui sollicitent les services des influenceurs en effet pour être efficace les sanctions doivent s'appliquer à tous les acteurs bénéficiant de l'influence commerciale qui enfreindraient la loi. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur sol sur une seule catégorie de personnes. Il faut assainir l'ensemble de la chaîne de de l'influence. Des influenceurs jusqu'aux annonceurs en passant par les plateformes car tous sont interconnectés. Et certains qui n'ont pas droit à la publicité dans le secteur de la santé notamment usé de l'influence pour enfreindre les règles. Les polémiques générées notamment sur les interventions chirurgicales oblige à poser des questions de déontologie. Il faut donc alerter les consommateurs a fortiori les plus fragiles. Au-delà de l'aspect commercial. Il était pourtant également de mettre des garde-fous sur des propos les influenceurs. C'est pourquoi une formation, une charte éthique qui engage toute influenceurs me semble nécessaire. Mes chers collègues, qu'il s'agit que qu'il s'agisse pardon Dali Man in vitro comme on a pu le voir dans notre commission des affaires économiques d'Intelligence artificielle des réseaux sociaux ces sujets nouveau nous privent parfois ils nous font peur, mais il vaut mieux toujours anticiper et ne pas faire la politique de l'autruche. On peut être contre hein on peut être pour, mais cela existe et existera il faut s'adapter et réfléchir à comment nous pouvons clarifier encadrer ces évolutions techniques et si il y a ah et scientifique qui débouche sur de nouveaux métiers. Et surtout protéger le consommateur pour restaurer ne connaît sèche de ces évolutions et une relation de confiance. Cette proposition de loi, il répond un parti c'est pourquoi ça faisait plus personne. Mon groupe RDSE votera pour ce texte. Très bien merci. Maintenant c'est Patrick Chaize qui a la parole pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la Ministre. Madame la rapporteur se ramène, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui je le rappelle une nouvelle fois été adopté à l'unanimité par la commission des affaires économiques. La semaine dernière. Est importante car très attendu nos concitoyens et scruté par nos homologues européens. En effet, il s'agit de la première fois au sein de l'Union européenne qu'une loi transversale dédié à la régulation de l'influence commerciale et discuter. Certes la grande partie des dispositions existantes en matière de protection des consommateurs de concurrence ou encore de santé publique s'applique, il n'y a pas vraiment de vide juridique, mais plutôt un halo d'incertitudes autour de l'influence commerciale. Les arnaques, les escroqueries et les dénonciations répétition nous ont conduits à se saisir de ce sujet et j'espère que nos homologues européens, en font de même. Encore une fois les parlementaires français se montre à l'avant-garde de la régulation de l'économie numérique et font preuve de justesse et de créativité en la matière. Nous en savons quelque je trouve Cette proposition de loi est effectivement une Pierre de plus à l'édifice d'une société numérique plus responsable qui exploite pleinement les opportunités offertes par la numérisation de notre économie tout en protégeant les plus vulnérables et en évitant les abus afin que ceux et porte unité profite au plus grand nombre. Je tiens ici à saluer les travaux de la rapporteur de la commission des affaires économiques Amel guéguerre qui dans un temps très contraint à mener à bien l'instruction cette proposition de loi. Nous avons su démontrer qu'au Sénat nous travaillons sans préjugés et indépendamment de toutes idées reçues. En l'espèce le travail mené a permis des apports significatifs visant à mieux protéger notre santé publique les consommateurs et les épargnants que nous sommes. D'abord en allégeant ou en supprimant les interdictions, les effondrements qui nous paraissait injustifié trop stricte ou trop pénalisant pour notre développement économique. C'est le cas de l'alimentaire mais aussi du commerce en ligne ou des cryptoactifs. Le texte adopté par la commission des affaires économiques me semble être parvenu à un bon équilibre qui n'aura pas pour conséquence de freiner l'innovation de nos entreprises et de nos entrepreneurs du numérique. C'est une bonne chose. Ensuite en rappelant les règles applicables aux acteurs de l'influence commerciale en les responsabilisant et en faisant preuve de pédagogie à leur égard. Autrement dit, désormais il n'y a plus d'excuse pour les acteurs malintentionnés qui décideraient malgré ce texte de ne pas respecter les règles. Je me satisfait ainsi des sanctions particulièrement dissuasive qui ont été votés dans la continuité des travaux de l'Assemblée nationale, ainsi que des interdictions supplémentaires qui ont été adoptés. Je pense notamment à l'interdiction de la promotion de l'abstention thérapeutique, les sachets de nicotine ou encore des abonnements à des pronostics de paris sportifs. Tout cela va dans le sens d'une meilleure protection collective. Vous le savez. Je suis sincèrement persuadé que parfois il faut savoir se montrer offensif pour obtenir des changements significatifs et durables. Surtout lorsqu'il y a des abus impunis. Je crois que je prêche ici hein. Convaincu en témoignent les débats que nous avons eu la semaine dernière sur d'autres sujets du numérique. Cette proposition de loi est une Pierre de plus à l'édifice d'une société et d'une économie numérique plus responsable. Elle s'inscrit d'une certaine façon dans la continuité de nombreuses autres initiatives parlementaires visant à civiliser l'espace numérique. Sans être exhaustif. Nous pouvons citer la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. La loi visant à lutter contre les contenus et n'est et ne sur Internet la loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image des enfants de moins de 16 ans. La loi visant à encourager l'usage du contrôle parental ou encore la loi sur le cyber score. Demain, nous discuterons. Une nouvelle proposition de loi relative aux droits d'image des enfants et la semaine prochaine d'un texte visant à instaurer une majorité numérique. Nous devrons ainsi chers collègues être vigilant à la cohérence des dispositions que nous adopterons. Au milieu de toutes ces initiatives. Je ne vous cache pas Madame la Ministre que j'attends avec impatience l'arrivée du projet de loi sur le numérique. Si je comprends bien ce texte et passera la seule adaptation de notre droit national au règlement européen sur les services numériques et les marchés numériques afin de devenir un véritable projet de loi programmatique pour le numérique. Vous l'aurez compris en la matière les par la les parlementaires que nous sommes ont des choses à dire et des propositions à formuler pour définir notre stratégie numérique des années à venir. En attendant mon groupe et moi-même voterons ce texte important est attendu sur la régulation des pratiques commerciales des influenceurs. Je vous remercie.

Madame la présidente. Madame la ministre madame la rapporteure. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, les choses ont beaucoup évolué. Nous sommes passés de la possibilité de retrouver des anciens camarades de classe avec le site Les Copains d'avant. A la possibilité de faire des connaissances. Puis de se créer un nouveau réseau de s'informer de communiquer nous élu en somme un parfait exemple. Et puis à celle de faire du commerce et de l'influence commerciale. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok pose de nouveaux défis auxquels les sociétés essayer de répondre. Déjà la transparence sur le fonctionnement des algorithmes. Pour éviter la mise en avant des contenus les plus trash qui font le plus d'audience. Et puis sur l'établissement d'une forme de responsabilité des plateformes dans la publication des contenus pour mettre fin aux attaques aux insultes et aux mensonges qui sont trop peu sanctionnée alors qu'ils peuvent avoir des conséquences graves. Et puis enfin la captation et la gestion des données personnelles, notamment à des fins commerciales qui n'a jamais eu la surprise de voir apparaître sur son fil d'actualité une pub qui correspond à une recherche ou à une discussion évoquait quelques minutes avant. Internet et les réseaux sociaux par essence, ce sont des espaces de liberté et d'expression totale qui ont abouti nous le vérifions chaque jour à une forme d'impunité et de jingle. Nous savons que pour vivre en société, la liberté ne peut s'exercer que dans un cadre avec des règles. C'est tout le sens de cette proposition de loi qui vise à lutter contre les dérives de l'influence commerciale. Qu'est-ce qu'un influenceur. Au final, rien de très nouveau, c'est le principe de l'homme ou de la femme sandwich. C'est le retour des réunions Tupperware. Tu me connais donc il me fait confiance. Donc tu achètes. Évidemment les marques sont à l'affût des influenceurs puisqu'ils sont suivis par un public jeune, voire très jeune, c'est la meilleure façon de leur parler de leur, de faire de la pub et de déclencher l'acte d'achat mais c'est aussi la meilleure façon d'abusé de leur crédulité. On peut penser ce qu'on veut des influenceurs sur le fond c'est un nouveau métier qui lui d'ailleurs n'a pas de problème à recruter. C'est une nouvelle forme de commerce. Et disons-le, une grande majorité des influenceurs exerce sérieusement leur métier. Nous avons été sensibilisés aux dangers de ces nouvelles pratiques grâce à des documentaires. Grâce à des films je pense aux films selfie qui décrit avec humour le comportement d'une famille qui n'hésite pas à utiliser ses enfants pour être reconnu parmi les influenceurs. Mais aussi grâce à des rappeurs connus Booba, qui dans son Style nous a alerté sur ces dérives. Face à tout ça il y a une réalité, celle des victimes. Des victimes qui ont cru en certaines et certains influenceurs qui se comportent comme des embobines heures des menteurs, voire des escrocs qui font sans scrupule la promotion de produits de luxe contrefaisant. Qui pousse à investir dans des banques Collins ou des NFT totalement bidon. Qui vendent des produits cosmétiques composés de substances dangereuses et interdites. Et plus grave qui encourage à recourir à des interventions de chirurgie esthétique qui laisseront des séquelles à vie. C'est pour ça qu'il est essentiel que les influenceurs soit également soumis aux règles de la consommation et du commerce qui régissent la publicité. Nous saluons le travail de notre collègue. Et de tous ceux qui ont contribué à poser un cadre et à instituer des sanctions utile. Avant d'en terminer, vous me permettrez d'insister sur un point auprès du gouvernement. De bien se donner les moyens de faire respecter les sanctions financières et pénales à l'endroit de celles et ceux qui sont installés à l'étranger. Souvent ça a été dit dans des paradis fiscaux et qui nous le constatons représentent la grande majorité des influenceurs. C'est totalement l'esprit de la proposition de loi et on compte sur le gouvernement pour qu'il suive les choses de près, tous les élus du groupe les indépendants voteront en faveur de la proposition de loi. Merci de votre attention. Nous aussi. Merci la parole est maintenant Anne-Catherine Loisier. Pour le groupe Union centriste. Madame

Madame la présidente, madame la ministre. Madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à un phénomène récent mais dont les caractéristiques et l'ampleur en matière commerciale évolue rapidement. Je salue donc tout particulièrement l'initiative de nos collègues députés et le travail de notre rapporteure Hamel Jacques R. Même si ce texte cible essentiellement les grands influenceurs. Nous sommes aujourd'hui à l'aube de ce que je qualifierais d'une nouvelle ère du marketing digital pour tous qui ne s'appuie pas que sur la notoriété, mais aussi sur les nanos où les micros influenceurs et c'est-à-dire tous ces jeunes appâtés par les facilités de l'outil et des gains et jusque-là peu informés du cadre légal et c'est sur ce point que je voudrais attirer votre attention, mes chers collègues, en effet, depuis quelques années, les marques s'attache les services d'apprentis influenceurs dont les comptes sociaux totalisent seulement quelques centaines, voire quelques milliers d'abonnés sur TikTok ou Instagram inscrit sur des plateformes comme Millau il 26 ou influence You ces apprentis influenceurs sont mis en relation avec des marques souhaitant valoriser leurs produits, certains intermédiaires n'impose aucun seuil de popularité n'importe qui peut donc vanter les produits des marques sur ses réseaux sociaux puis recevoir une commission sur les ventes générées. Ses créateurs de contenus. Non en général aucun contact avec la marque. Certains disent clairement qu'ils sont rémunérés, d'autres présentent les produits comme s'il les avait choisi eux-mêmes et se livrent à de véritables éloges, l'un des objectifs des plateformes de recrutement, je dirais, et de permettre aux entreprises d'enrôler des dizaines voire des centaines d'influenceurs avec le minimum d'efforts des campagnes massifier et. Sont ainsi déployés par certaines marques je cite un professionnel les abonnés des petits influenceurs sont leur entourage Direct ou les personnes qui se considèrent comme proche de. Ils sont très efficaces pour générer des conversations des conversations et les transformer en achat en revanche pour faire découvrir un produit au plus grand nombre rapidement les gros influenceurs demeure préférable. Face au déploiement de ces stratégies commerciales évoque l'utile à l'encadrement des pratiques et donc bel et bien un sujet d'actualité qui ne ne concerne pas pas que les grands influenceurs mais je dirai tout un chacun dans son domicile, dans sa famille dans ses proches. Pour cela, nous le savons, la répression des fraudes, manque de moyens. De fait, les scandales liés aux produits vantés se sont multipliées dropshipping abusif produit s'avérant dangereux placements financiers risqués. Le texte de la Commission prévoit une définition plus précise de l'activité d'influence commerciale, un renforcement des pouvoirs de police administrative de la DGCCRF et une augmentation des montants des amendes. Le point faible restant à ce jour. Madame la Ministre les 10 ETP consacrée à ce contrôle, ce qui est notoirement insuffisant. Vu l'ampleur de la tâche. La présente, proposition de loi érige un cadre plus clair et plus protecteur pour les consommateurs, elle interdit la promotion de certains biens et services, comme, comme les produits financiers elle encadre plus précisément le dropshipping diverses dispositions visent à renforcer la vigilance et la responsabilité des consommateurs sur la nature des annonces promotionnelles. D'autres enfin ont été supprimé par notre commission pour éviter des durcissements qui relancerait des débats sur des sujets déjà stabilisée comme sur les produits alimentaires ou le vin enfin ce texte sera complétée par la prochaine transcription de la directive européenne dite DMA DSA. La commission a ainsi adopté un amendement visant à conditionner l'entrée en vigueur de la présente proposition à la réponse de la Commission européenne attestant de sa conformité au droit de l'Union. Cette proposition de loi que le groupe centriste soutiendra permet donc de renforcer le cadre de pratiques mouvante, sachant que la nature même des réseaux sociaux et de leur usage entraînera sans nul doute la nécessité de revoir encore ces dispositifs à l'avenir, je vous remercie de votre attention. Et la parole est maintenant à Édouard Courtial pour le groupe Red les républicains. Merci madame la présidente, madame la présidente de la commission et Madame la Ministre Madame la rapporteure, chers collègues. Le développement de l'économie numérique et des réseaux sociaux a donné naissance à des phénomènes encore inimaginable il y a quelques années. Parmi ceux-ci, l'émergence de célébrités documentant jour et nuit leur vie et la mettons à disposition du public sur toutes les plateformes inimaginable. Mais entre 2 selfie à la plage et un poste sur une recette de cuisine et le public est également exposées à du contenu bien moins innocents et désintéressé placement de produits concours promotion rémunéré de services et produits et cetera. Pratique constituant le principal moyen de rémunération de ce que l'on appelle désormais des influenceurs ne sont malheureusement pas toujours réalisées dans la plus grande des transparences. Ce flou et certaines pratiques à la légalité ou à la morale douteuse s'explique par la relative nouveauté du secteur et un manque de régulation spécifique. Bien que la régulation générale soit également applicable. Rien qu'au 1er trimestre 2023 sur 50 influenceurs contrôlée par la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, 60% ont fait l'objet de constats d'infraction qui ont conduit à 18 injonction de cesser des pratiques illicites et à 16 procès-verbaux pénaux. lui devenait donc. D'agir avec par exemple des scandales de promotion d'actes médicaux réalisés en dehors de tout cadre médical et présentant des risques énormes pour les victimes. de cette PPL et de rétablir un peu d'or dans ce qui est devenu un véritable Far-West où certains influenceurs s'apparentent à des charlatans vendant remède miracle et autres arnaques en 1er lieu cette PPL donne enfin une définition légale de la notion d'influenceur commerciale par voie électronique afin de lever un flou qui a trop longtemps pu être exploitées par des personnes malentendantes dans un même objectif, de clarté et de transparence. L'obligation faite pour les influenceurs d'afficher clairement le caractère commercial d'une opération permettra d'éviter des dérives et la confusion dans l'esprit du public. La nature particulière de ce public appelle d'ailleurs à une vigilance accrue. En effet, les mineurs représentent une part importante du public des influenceurs voire même majoritaire pour certains et ton père d'un petit Pierre bientôt 10 ans. Je parle d'expérience la naïveté l'insouciance enfantine doivent être protégés face aux personnes tentant d'en abuser pour leur profit personnel. Ce à quoi répond l'article 5 ce dont je me félicite. Cette PPL accompli donc un travail nécessaire de réglementation dans le secteur en ayant. Besoin tout en laissant une liberté d'action assez grande aux acteurs pour ne pas freiner l'activité économique. Les influenceurs violent la loi ne pouvant plus se cacher derrière le flou de cette dernière, la commission a eu raison d'ajouter des sanctions dissuasives pour les influenceurs récidiviste. Enfin, il ne faut se bornant pas oublié un acteur indispensable de l'influence en ligne les plateformes ces relais sans qui les insultent les influenceurs existeraient pas leurs responsabilité sur les contenus qu'elles hébergent devrait faire l'objet d'un examen rigoureux lors de l'examen prochain du projet de loi sur le numérique annoncé par le gouvernement. Pour le meilleur mais trop souvent pour le pire, l'influence sur Internet est un secteur en pleine expansion et qui semble destiné à perdurer une réglementation juste et intelligente et la fondation solide sur laquelle un secteur peut se bâtir et prospérer. Ce texte ne sera sûrement pas la réglementation finale en la matière mais il est une première Pierre robuste et nécessaire qui bénéficient aussi bien aux consommateurs qu'aux influenceurs respectueux de la loi je vous remet. Et dernière orateur de sont général. François Bonhomme. Pour le groupe Les Républicains. Madame le Ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues. En France, à l'air de On connaît une expansion continue de l'activité commerciale d'influenceurs dans tous les domaines. Que ce soit la mode de la beauté et le bien être tourisme l'alimentation encore la technologie ou les jeux vidéo. D'autres assurent la promotion des produits ou de conseils, relatifs entre à l'entreprenariat ou encore la finance à l'éducation. On voit même des influenceurs politique naturellement, ces pratiques sont favorisés par l'appât du gain et suscite une multiplication parfois anarchique des vocations entraînant de très nombreuses dérives Il existe déjà. Un certain nombre de règles du juridique et le législateur se doit naturellement d'imposer une transparence nécessaire et la responsabilité dans la pratique commerciale d'influenceurs ainsi que de mieux protéger les personnes visées. Souvent le jeune par ce type de message. Malheureusement. L'arsenal législatif actuel s'avère bien trop limité et souvent dispersés. L'activité des influenceurs ne ne s'exerce pas certes dans une zone de non-droit. Et des guides ou. Tout simplement la loi sa peine de 2017 sont venus. en quelque sorte rappeler les règles de bonne conduite pourtant. Malgré ses obligations, il apparaît nécessaire aujourd'hui de légiférer. Pour plus de transparence et de responsabilité notamment dans la pratique commerciale des influenceurs. Ce manque de transparence nécessite tout d'abord une définition juridique de celui-ci. Que vient opportunément. Précisé l'article 1er. Plus de transparence est également nécessaire en ce qui concerne les partenaires commerciaux. De manière générale, de nouvelles possibilités technologiques offertes. Ils viennent favoriser un certain nombre de pratiques et de dérives commerciales parfois dangereuses. Cette situation appelle donc. Une réponse rapide et une bien meilleure protection de l'internaute consommateur. De même la. La promotion de certains produits ou services pouvant nuire à la santé ou à la situation financière de certains followers nécessite de nouvelles interdictions limitation. Concernant la santé même si les influenceurs commerciaux ne sont pas exemptés de l'application de la loi Évin encadrant la publicité. Les sénateurs ont. Souhaité inscrire explicitement l'interdiction de toute promotion directe ou indirecte de produits nicotiniques. Au-delà de cigarettes le vapotage et les sachets de nicotine qui sont concernés. Autre mesure qui avait été introduite par article de c'est l'encadrement de la promotion des boissons et aliments trop sucrés. Des informations à caractère sanitaire devait figurer au sein du message promotionnel et faire l'objet de au préalable d'un arrêté interministériel après avis des agences sanitaires concernées. Il est regrettable et même dommageable que la commission ait fait le choix de supprimer toutes dispositions visant les produits alimentaires. Même chose pour l'ancienne article de C. à qui prévoyait que les influenceurs. De moins de 16 ans ne pourrait plus faire de publicité pour des produits alimentaires trop sucré. Ce dispositif visait pourtant à protéger en particulier le jeune public dont on sait qu'ils sont des consommateurs captifs pour une partie de l'industrie agro-alimentaire. À ce sujet, j'aurai l'occasion de défendre 2 amendements. Pour y revenir en matière de santé. La proposition de loi entend aussi interdire la promotion de tout acte de chirurgie ou de médecine esthétique qui n'est pas rare en effet de voir des influenceurs, faire la promotion d'injections de Botox d'actes d'orthodontie. De liposuccion d'implantation capillaire avec tous les risques sanitaires. Que cette démarche peu soucieuse de l'éthique comporte. Et la commission a fort opportunément par amendement. Ajouté. Une interdiction pour toute promotion de la station de thérapeutique ou de pseudo-traitements. En fait la législation actuelle est beaucoup trop dispersée et demande donc une rédaction d'un texte unificateur en matière d'influence commerciale où sont traités l'ensemble des principaux sujets. Je crois que c'est la principale vertu de ce texte. Sans doute à l'usage. Cette proposition de loi laissera-t-elle apparaître des insuffisances juridiques auxquels initiateur de voir à nouveau y répondre. l'article 7 prévoyant la remise par le gouvernement d'un rapport d'information et d'évaluation au Parlement sur la mise en oeuvre de cette proposition de loi permettra, je l'espère d'identifier ces nouvelles failles et si besoin de les combler. La nouvelle rédaction de cet article. Vous voulez Paname la rapporteure. Paraît en ce sens plus précises et opportunes. Et donc, à l'exception de celui concernant les conditions de promotion du groupe du produit alimentaire. Je pense que ce texte mérite tout notre soutien. Merci la discussion générale est donc Close et nous allons passer à l'examen du texte de la commission, avec d'abord 2 amendements en discussion commune et je vais donner la parole à Henri Cabanel pour le 52. Si madame la présidente, madame la ministre, chers collègues. Cet amendement propose de rétablir en partie la version de l'article 1, adopté à l'Assemblée nationale. Le texte issu de la commission des affaires économiques ne mentionne que les communications des influenceurs réalisé à titre onéreux, ce qui peut peut exclure les avantages reçus à nature. Or, ces derniers sont très fréquents et doivent être expressément prise en compte en étant considéré comme participant de l'activité d'influence commerciale à ligne des personnes peuvent faire acte d'plus à se détourner par exemple laver des conseils de beauté dans les magazines de les pages sort en ligne avec citation des produits, un échange d'davantage nature et qui sont sur les radars du E-commerce car pas de contrat ni de rémunération un montant minimal des avantages en nature serait fixé par décret par exemple 150 euros comme c'est le cas actuellement pour les, les parlementaires et les réseaux et les représentants d'intérêts. Il n'est pas proposé de rétablir le critère de notoriété qui apparaît complexe à appréhender. Merci donc le périmètre des activités d'influence est difficile à évaluer dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune régulation à l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, de la commission des des affaires économiques. Le texte que nous examinons aujourd'hui se borne à réguler l'activité d'influence commerciale, c'est-à-dire l'influence réalisé à titre onéreux et lorsqu'elle est encadrée par un contrat. Quid du reste des contenus. Si l'objectif est de lutter contre les dérives de l'influence cette définition même de l'influence est insuffisante. La promotion de biens et de services d'opinion d'idées par les influenceurs suivis par les milliers d'abonnés y compris lorsqu'il exerçait activité sans contrepartie matérielle nécessite d'être régulées. Concernant les médias classiques, la liberté de communication fait l'objet de limitation comme le prévoit l'article 1 de la loi du 19.186. Il est donc légitime de vouloir étendre ces limitations. Des aux aux réseaux sociaux. C'est pourquoi à l'Assemblée nationale, notre collègue Aurélien taché, avait proposé l'instauration d'un seuil de nombres d'abonnés. Une définition qui trouve aussi ses limites pour élargir le périmètre. C'est une nouvelle régulation. Je vous propose donc de compléter, plutôt les améliorations de notre rapporteur en nous appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation afin de distinguer l'influence commerciale de l'influence et de permettre des régulations complémentaires et distinctes dans le cadre légal. Je vous remercie qu'quel est l'avis de la commission, madame la rapporteur sur ces deux amendements. Madame. C'est madame la présidente. Donc ces deux amendements. Visent à modifier la définition de l'activité d'influence commerciale. Adopté en commission. 2 amendements qui visent à supprimer donc la mention à titre onéreux cette mention s'entend au sens du code civil c'est-à-dire qu'il y a une activité d'influence commerciale lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un Avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Cet Avantage peut être une rémunération financière un Avantage en la Thur ou un bénéfice économique pour sa propre activité toutes les pratiques et modalités de rémunération devrait donc être couvertes par la définition actuelle l'amendement de 52 pardon vise également à introduire un seuil. En somme, ou en valeur pour les avantages en as-tu reçu. Un produit de faible valeur dont la promotion est effectué par des influenceurs peut par exemple avoir des conséquences importantes sur la santé des consommateurs. Donc ce serait dommage que la promotion de ce produit soit exempté des règles que nous allons voter aujourd'hui. L'amendement 17 propose de réintroduire un critère d'audience mais l'influence se mesure pas seulement au nombre d'abonnés, mais aussi à la capacité d'influer sur les habitudes de consommation et les pratiques des internautes tous les influenceurs commerciaux doivent être concernés par cette loi. Voilà pourquoi je propose un avis défavorable pour ces deux amendements. 52 et 17. S'il n'y a pas de d'explication de vote. Je vais donc mettre aux voix, ces deux amendements qui ont reçu un double avis défavorable qui est d'abord le 52 qui est pour. Qui est contre ou qui s'abstient n'est pas adopté le 17 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté à l'article. Excusez-moi. Les amendements sont arrivés trop vite

Le texte que nous voterons ce soir a pour objectif de permettre le développement responsable et respectueux de l'activité commerciale. Notamment de l'influence de Par ailleurs, je remercie d'ailleurs les auteurs de de de ce texte qui sont en tribune pour leur présence. Le but est aussi de protéger les utilisateurs et particulièrement. Les les plus fragiles, les jeunes mais également de préserver l'activité des créateurs de contenus vertueux. C'est dans un texte qui responsabilise toute la chaîne de valeur de l'influence commerciale qui régule cette activité et en et en sanctionnant les dérives. Il s'agit pas d'entraver la liberté d'expression ni. D'entraver le développement de cette activité l'influent l'influenceur exprime un point de vue donne des conseils dans un Style et un traitement qui lui sont propres. Et que son audience identifie d'ailleurs. Il est responsable de ses contenus et j'insiste bien sûr il est responsable de ses contenus qu'il diffuse notre abonnement propose d'intégrer cette notion de responsabilité dans la définition de l'activité d'influence d'influence commerciale et ce sans préjudice de dispositions qui figurent à l'article 2 bis de la proposition de loi bien sûr c'est satisfait mais cette loi a une visée pédagogique. Elle doit sensibiliser les influenceurs sur la portée des contenus qu'il diffuse et au regard de leur large audience de leur responsabilité d'ailleurs dans la protection de leur public. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure. Madame la présidente. Donc un ajout rédactionnelle qui est proposé ici mais qui ne semble pas nécessaire. Pourquoi, parce qu'un influenceur qui ait pu bien texte une photo ou une vidéo depuis son compte et de fait, responsable de ce qui publie car son nom son image et sa personnalité y sont associés. Voilà pourquoi je propose un avis défavorable. L'avis du gouvernement. J'aurais le même avis. Madame la présidente. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un double avis défavorable qui pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je me vois l'article 1er qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 1er bis, un amendement de la rapporteure. Il s'agit d'une précision juridique pour assurer la bonne coordination avec la loi relative à l'exploitation commerciale de l'image des enfants. qui est contre qui s'abstient. Il est adopté à l'article 2 Harlequin moment 41 monsieur pardon. Merci madame la présidence là. L'article 2 A est un article chapeau qui rappelle que l'activité d'influence commerciale et soumise aux dispositions relatives à l'encadrement de la promotion des biens et des services. Les influenceurs s'adresse à une communauté d'abonnés qui fédère d'ailleurs les contenus qu'il diffuse peuvent avoir une incidence significative sur le comportement de leurs abonnés. Les dispositions de cet article ont une portée pédagogique notre amendement propose d'aller au bout de la démarche pédagogique en rappelant très clairement que les interdictions et les sanctions encourues sont également applicables et par ailleurs et proposez de rappeler que les manoeuvres pour contourner ces règles sont interdites. On pense par exemple au recours aux messages privés pour. Pour s'adresser aux membres d'une communauté et de contourner ainsi. Une interdiction ou encore à la diffusion de Story dont les contenus éphémères qui empêche toute contestation ou de l'infraction. Merci Des précisions rédactionnelles, qui ne sont pas forcément nécessaire puisqu'elle revient à dire que le contournement de la loi est interdit. Et par ailleurs, les sanctions applicables aux influenceurs différencié selon les infractions commises commises sont bien précisé dans cette proposition de loi donc un avis défavorable. Avis du gouvernement, pour les mêmes raisons, j'aurais le même avis que le rapporteur défavorable. Je vais donc mettre aux voix sa maman. 41 double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté le 72 est un amendement rédactionnel. Si le gouvernement n'y voit pas d'inconvénient. Et le Sénat non plus. Il est adopté. Merci, pardonnez-moi madame mardi art il était c'était c'est rédactionnelle qui vous pose problème à la qui nous amène à commenter. Tout petit problème Pardon, madame la présidente, je demanderai le retrait à défaut sera un avis défavorable formulation pourrait être comprise. Comme visant les conditions techniques de la diffusion des publicités davantage que l'encadrement spécifique des publicités diffusées, c'est pourquoi la vie sera. Du côté du gouvernement défavorable. Qui contre qui s'abstient. Il est adopté 2 amendements identiques, faisant l'objet d'une édition commune. Monsieur Cardot. Merci madame la présidente. Alors que les publicités pour l'alcool sont interdites à la télévision et au cinéma, elle reste autorisée sur Internet sous réserve de respecter un certain nombre de règles. Nous sommes confrontés depuis quelques années à une présence de de plus en plus massive de des jeunes et de la de la publicité pour l'alcool sur les réseaux sociaux. Cela remet en cause l'efficacité des actions de prévention et de lutte contre la consommation excessive d'alcool, particulièrement auprès des jeunes publics. Or ce sont bien les réseaux sociaux qui arrive en tête des médias consommée par les jeunes, l'association France. Alerte sur l'importance de contenus illégaux, créés par les influenceurs pour promouvoir des marques d'alcool et sur les difficultés à contrôler et à faire retirer les contenus illicites et obtenir des sanctions à France. Démontre que plusieurs milliers de contenu de personnes exercent une activité d'influence commerciale promouvant une marque d'alcool. Ont pu justement d'être observés en un an sur les réseaux sociaux. Une partie significative de ces contenus enfreint la loi Évin. Justement, il s'agit de publicité déguisée avec un vérité avec une véritable mise en scène fabriqué pour créer un phénomène d'identification et de proximité chez les jeunes, c'est c'est une incitation à la consommation d'alcool notre amendement propose ainsi de préciser que les influenceurs doivent indiquer le message à caractère sanitaire directement sur l'image ou la vidéo du contenu publicitaire pendant toute sa diffusion. Je vous remercie. Monsieur le Président Ruquier pour le 58 identique. Oui merci. La présidente Madame la Ministre un amendement identique de madame Le Guillotin. Sur les supports autorisés, la diffusion de contenus publicitaires en faveur de l'alcool, tels que l'affichage et la presse. Le message à caractère sanitaire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et directement écrit sur les images et les influenceurs déjà l'obligation d'un guide, indique un message à caractère sanitaire pour accompagner leurs publicité en faveur d'alcool mais sociaux laisse la possibilité d'inclure ce message à la fin d'une inscription qui accompagne les vidéos les images.

le message à caractère sanitaire lorsqu'ils promeuvent l'alcool sur les côtes du SMR le message. Pas indiqué, dans un souci d'harmonisation règles lui sidère les influenceurs doivent directement sur l'image ou la vidéo du contenu publicitaire. Indiqué ce message à caractère sanitaire. Merci qui. De l'avis de la commission. Les amendements donc 25 et sans ça 58 hein porte sur l'affichage du message. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé sur l'image ou la vidéo publiée par influenceurs durant l'intégralité de la promotion. L'objectif de cet article 2 A. Et d'effectuer. On a eu l'occasion de le dire et de le redire, par souci de pédagogie à l'égard des acteurs du secteur, une clarification sur le cadre juridique applicable aux influenceurs. Il est ainsi déjà rappelé qu'ils doivent respecter les dispositions, certaines dispositions du code de la santé publique. Je le rappelle et c'est c'est une ligne que nous tenons vraiment sur tout le texte l'objectif l'enjeu ce n'est pas de durcir le cadre existant, mais déjà de faire respecter ce cadre. C'est pour cela que la commission des affaires économiques a adopté un amendement visant à adopter à doter pardon, les associations de lutte contre l'alcoolisme du statut de signaleurs de confiance afin de faciliter la régulation des contenus publicitaires frauduleux en matière de promotion de l'alcool donc un avis défavorable pour ces deux amendements. 25 et 58. Merci madame la présidente. L'amendement. De la sénatrice Meunier. Nous sommes clarifier les modalités d'application de l'insertion du message sanitaire pour les publicités réalisées par les influenceurs. Et c'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur le. L'amendement de Madame Meunier. Ce sera aussi en amendement favorable pour l'amendement 58 de Madame Guillotin.

Rappeler quand même hein à mon collègue. Car, donc déjà au PLFSS. Votre groupe avait déposé un amendement. Pour augmenter les droits d'assise ce concernant le 20. Je crois qu'à travers votre amendement. Une fois de plus. Vous attaquez. Le le milieu assis et l'alcool il y a le vin et les spiritueux. Je peux en faire attention. Mes chers collègues à mon Maingot le milieu viticole est en danger. Je pense que ce type d'Amman demain ne va pas dans le bon sens. Donc attention au vote. vote. Je vais donc mettre aux voix pardon Monsieur Guey, excusez-moi. Merci madame la présidente, monsieur. C'est dur d'être à l'extrême gauche. C'est pour ça Merci madame la moi. On a un débat. On est face à un phénomène quand même. D'hyper-alcoolisation. De pré-adolescents et préadolescents. Qui. Boivent de plus en plus vite. Avait des alcools de plus en plus fort, non pas pour. Un aspect entre guillemets festif. Mais bien. Pour se mettre extrêmement mal. Nous sommes face à ce phénomène et on ne réglera pas tous par cette PPL et en encadrant évidemment la question mais laissez. Et la question que vous posez laisser. Des influenceurs à des influences se filmer entre. Et penser que l'alcool serait celle de moments festifs et cool. Et qui n'aurait aucun problème de santé publique ne va pas dans le bon sens et si la loi Évin a été créé, c'est parce que je pense que nous avons déjà eu ce débat est déjà le régler. Donc oui un encadrement et personne ici ne veut interdire l'alcool. Personne ne parle de ça et les deux amendements ne reviennent pas sur cette question mais simplement qu'au moment. Où on le fait on puisse indiquer que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que des influenceurs des influenceuses qui ce film ou qui en font la promotion au même titre que la publicité ailleurs en forment. La jeunesse et franchement. Que nous n'ayons pas et que nous ne voulions pas aller vers cela. J'ai un petit débat. Et je pense que nous devrions suivre ces deux amendements et l'avis du gouvernement sur cette question là. Il en va. De la santé publique notamment sur un public extrêmement jeune, extrêmement influençables. Je vous remercie. Merci madame la présidente. Oui je, je rebondis sur ce que vient de dire collègues Fabien Gay. Effectivement il y a un moment, c'est l'intérêt général qui prime et l'intérêt général, c'est de faire attention à la santé de notre de notre jeunesse. Bien entendu, il n'est pas question ici de prohibition de l'alcool mais il s'agit de protéger bien entendu, et bien il y a les facteurs économiques, il faut prendre l'économie en compte mais ça ne doit pas être le facteur dominant et qui doit opérer toutes les autres conditions pour pouvoir faire de la publicité sur un produit, on ne peut pas se permettre de vendre ou d'inciter à consommer n'importe quoi, on le sait bien, on le dit assez souvent sur des drogues. Eh bien l'alcool doit faire partie aussi des produits sur lesquels on doit être très vigilant et moi je soutiens complètement cet amendement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cet amendement. Monsieur cardons et madame la rapporteure parole après. Oui merci madame la présidente. Effectivement c'est juste rappeler à mes collègues. Durant 2 des rangs de de droite que tout simplement ce cet amendement vise à être en. En corrélation avec la mention sanitaire obligatoire qui existe déjà sur la loi Évin, et donc c'est en complément, ça vient appuyer donc je ne comprends pas pourquoi on a ce débat en fait puisque vous avez certainement voter la loi Évin je. Donc je je suis, je suis très surpris qu'on revienne sur des choses comme ça mais bon bref c'est peut-être une une affaire. De d'influence de lobbies en particulier dans le viticole qui qui vous pousse à faire ce genre d'intervention.

madame la rapporteure et Madame Eustache-Brinio ensuite. Merci, merci, Monsieur le Sénateur cardons de rappeler ce que nous soutenons en fait hein. Dans le texte c'est qu'il existe déjà un cadre cadre légal qu'on le mette en place et qu'on le fasse respecter, donc vous l'avez dit très clairement, je ne l'aurais pas dit mieux. Donc merci beaucoup et puis je le redis la l'objet de cette PPL. L'objet de cette PPL. Ce n'est pas de d'évoquer en tout cas ce sujet qui est bien sûr un sujet que nous partageons une préoccupation que nous partageons la protection de notre jeunesse face encore une fois aux ravages de l'alcool et ce n'est pas le sujet, je le redis cette PPL voilà c'est ce que je voulais ajouter merci. Madame le stage Bruno. Oui merci madame la présidente. Je suis désolée madame Brochard mais moi je vais voter cet amendement parce que cet amendement de bon sens. Sincèrement, je pense que on parle aujourd'hui de dérive des influenceurs on parle c'est le texte écrit donc la dérive elle existe et rappeler des choses rappeler des règles parce que c'est un domaine que nous ne maîtrisons plus ces influenceurs quand vous demande aux petites filles à l'école ce qu'elles veulent faire va tout influenceuse parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc si un texte qui doit commencer à mettre des limites partout, je pense qu'il est bien de le faire et moi, je voterai cet amendement. Madame la présidente Prima. Merci madame la présidence je voudrais comme l'a fait madame la rapporteure rappelé la position de la commission. La position de la Commission. C'est-à-dire que ceux qui s'applique partout et la loi Évin s'applique partout s'applique aussi pour les influenceurs Tout ce qui est marqué dans la loi Évin s'applique ici pour les influenceurs. Il y a donc pas de surenchère ou de sous-enchère ou de. d'une droite sénatoriale de de de ne pas lutter contre l'alcoolisme des jeunes c'est vraiment des accusations qui sont pas tout, pas du tout fondé je voudrais pas qu'on soit dans la caricature ici l'article cet article dit de faire de, d'appliquer la loi Evin. Donc, cet amendement est superfétatoire. C'est tout. Et ce qu'il n'y a plus d'explications de vote tiré quatre du code de la santé publique indique que toute publicité pour une boisson alcoolisée à l'obligation de comporter un message sanitaire sans spécification dans Pérès ment dans un objectif d'uniformité de stabilité juridique,

Bien je vais donc mettre aux voix, ces deux amendements identiques, qui ont reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement qui est pour.

Je. Défendu. Il est défendu. Très bien. Et le second n'est pas soutenu, bien. Non il y en a aucune qui là OK. Hé ben écoutez madame la rapporteur, vous allez nous dire ce qu'il avait dans cet amendement. La clarification des règles applicables en matière de retransmission illicite des manifestations sportives et bienvenue. Cela s'inscrit donc dans la continuité des travaux de la commission des affaires économiques sur l'interdiction des promotions pour des abonnements à des paris sportifs. L'objectif poursuivi est donc le même mieux protéger les consommateurs dans la perspective des grands événements sportifs à venir. Voilà pourquoi je propose un avis favorable pour ces 2 amendements trois Merci madame la présidente. L'alinéa 1 de l'article 2 a clarifie dans une disposition chapeau que les réglementations applicables à la promotion et à la publicité des biens et services s'applique aux influenceurs comme vient d'ailleurs de le rappeler, la président de la commission des affaires économiques. Cette liste. Non exhaustive de dispositions applicables à l'influence commerciale, elle doit être courte notamment vous le savez, par respect du principe constitutionnel de la portée normative de la loi. J'ajoute que l'amendement ajoute dans cette liste, l'interdiction des retranchements illicite de compétitions sportives. Qui sont déjà prévues aux articles L. 333 du code du sport. Il ne s'agit donc pas pour nous de dispositions portant sur la promotion de ces retransmissions. Ils ne sont pas en rapport Direct avec l'objet de cette loi. C'est pourquoi nous demanderons le retrait, le cas échéant, ce sera. Un avis défavorable. Alors je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 3 qui a reçu un avis favorable de la commission un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Je me vois l'article 2 A qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté un amendement 18 de Madame de Marco. Cet amendement est un amendement de coordination Abella l'amendement 17, il vise à étendre les dispositions du présent article à l'ensemble des d'utilisateur du réseau exerçant une forme d'influence afin de préserver la santé publique mais aussi l'environnement ou le droit d'auteur, comme nous allons en débattre. Quel est l'avis de la commission. Un amendement qui porte sur l'élargissement du régime d'interdiction à l'ensemble du secteur de l'influence commerciale et non commercial, je le rappelle, l'objet de cette proposition et bien d'encadrer le secteur de l'influence commerciale. Voilà pourquoi je propose un avis défavorable.

monsieur Cabanel. Merci madame la présidente. L'article 2 B de la proposition de loi interdit aux influenceurs toute promotion directe ou indirecte de le soin, c'est qui que portant atteinte à la protection protection de la santé publique, la violation de cette interdiction est désormais puni de 2 ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. Des des interdictions portant sur d'autres domaines ont été introduites en commission promotion de sachets de nicotine abonnement aux pronostics sportifs encadrement des jeux de hasard cet amendement propose d'éteindre les interdictions et donc les sanctions applicables en cas de violation de ces dernières aux personnes physiques ou morales qui sollicitent les services des influenceurs. Marc entreprises individus en effet pour être efficace les sanctions doivent s'appliquer à tous les acteurs bénéficiant de l'influence commerciale qui enfreindraient la loi. Madame la Ministre pour l'amendement 65. justement pour le recentrer sur les obligations nouvelles qui ne concerne que l'influence commerciale, et pour en exclure le rappel d'interdiction déjà existantes. Les alinéas qui ne font que rappeler les dispositions déjà applicable à droit constant aux influenceurs ont leur place à l'article de ah les réinscrire une seconde fois à l'article 2 B en prévoyant. Une sanction spécial introduit comme vous l'imaginez un risque constitutionnel de non bis in idem in idem. Il est en revanche absolument nécessaire de préciser le régime de sanctions qui sera applicable en cas de manquement aux dispositions nouvelles prévues par l'article 2 qui concerne la l'interdiction de faire la promotion des actifs numériques. Le présent amendement prévoit que le régime de sanctions qui sera applicable. Sera celui prévu par l'article L 222 Tiret 16 Tiret 1 du code de la consommation pour des manquements du même type. Je vous remercie.

Cet amendement a pour objectif d'interdire aux influenceurs d'interagir ou de se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec des animaux non domestiques dont la détention comme animal de compagnie est interdite en France. C'est cohérent avec ce que nous avons déjà voté dans le cadre de la loi du 30 novembre 2021, puisque le prévoyait cette loi, l'interdiction de l'exploitation de ces animaux non domestiques dans les spectacles itinérants ainsi que leur présentation en discothèque. De même elle avait très fortement restreint et encadré leur présentation lors d'émissions de variétés ou jeter Élysée. Pourquoi est-ce qu'on fait cette proposition parce que ces interactions et mise en scène impulsée par des influenceurs alimente un trafic important d'espèce non domestique et participe évidemment au mal-être de ces animaux. Je pense qu'il n'est pas utile d'y insister un influenceur, qui s'expose sur ses réseaux avec des animaux sauvages le fait à pur dessin lucratif personnel cherchant à faire le buz puisque c'est le nombre de ses abonnés qui détermine le montant perçu à chaque poste et qui lui permettra de nouer des partenariats publicitaires à titre informatif. Ce montant peut d'ailleurs atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros pour un seul poste. C'est donc une promotion, c'est bel et bien une action, d'influence qui a une contrepartie financière se mettre en scène avec un animal sauvage est devenue un gage de succès qui se monnayent cher, on assiste à des surenchères pour des shooting photo avec des ours, des serpents, d'autres animaux. C'est un business juteux qui se développe au détriment des animaux. Interdire aux influenceurs de poster des photos ou des vidéos, les mettant en scène avec des animaux non domestiques permettra d'enrayer cette escalade qui favorise les activités illégales en France et contribue au trafic d'animaux non domestiques. Dans le 1er amendement d'interdire. Toute promotion de copies Trading promotion du bitcoin autres crypto-LFT ou placements hasardeux et dans le 2ème mouture ne proposant juste les placements les plus à risques, pourquoi. Aujourd'hui 14%. Des 15 24 ans disent détenir des cryptomonnaies ou envisager d'investir dans l'année. L'an dernier sur Instagram, c'est plus 30% de publicité pour dire venez investir, même si vous ne connaissait pas. Le but est de suivre celles et ceux qui vous donne des conseils et avec cela vous deviendrez immensément riche. Et la réalité. C'est comme au casino. Pour un gagnant ou une gagnante, c'est des dizaines, des centaines de milliers de gens qui perd toutes leurs économies, et à chaque fois. C'est en réalité la banque qui ramasse par exemple l'an dernier. Hein des influenceurs les plus connues crypto gouv. Arnaqué 300 personnes pour près de 404 millions d'euros. Donc on voit qu'y compris. On peut avoir des jeunes extrêmement vulnérables qui ne rêve qu'une chose de la gloire et beaucoup de fortune et qui pensent qu'en suivant des influenceurs. Ils vont pouvoir devenir des traders de haut vol et qui en réalité perd toutes leurs économies, c'est exactement la même question et je pense qu'on devrait avoir le débat avec le gouvernement. Sur la question des paris sportifs, je pense qu'il faut l'encadrer plus sévèrement sur les paris sportifs en ligne, y compris dans la perspective de la Coupe du monde et des Jeux olympiques qui se dérouleront en France donc nous proposons dans le premier, d'interdire tout cela et dans le deuxième c'est un amendement de repli au moins ce qui est. Les placements à très haut risque et qui font perdre beaucoup d'argent. Madame Boulay-Espéronnier pour le 28. Madame la présidente. Dans la foulée de l'amendement de mon collègue Arnaud Bazin. Le 18 novembre 2021. Le Sénat a adopté la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. La mesure phare de cette loi. Les animaux sauvages plus particulièrement l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants cet amendement s'inscrit donc dans la continuité de ce texte. Au cours des dernières années. Nombreux sont les influenceurs avoir fait le Buzz en postant avait. En poste posant avec des animaux sauvages captifs au 1er rang desquels le Serval poser avec ces animaux et la garantie d'une certaine audience l'animal sauvage fascine pouvoir se prendre en photo est perçu comme un privilège que beaucoup sont prêts à monnayer très cher le trafic d'animaux sauvages est particulièrement lucratif à l'échelle mondiale et représentent un marché estimé par le WWF à 19 milliards de dollars par an, selon l'Office français de la biodiversité cité. Il s'agit de la 3ème activité criminelle la plus lucrative, au monde après les trafics de drogue et d'armes. On pourrait penser que cette activité n'est possible que dans les pays du monde ou le bien-être des animaux et des droits humains sont bafoués sur l'autel du profit. Pourtant cette mode lancée par des influenceurs a rapidement été imité en France. Ses activités en plus de porter préjudice aux animaux encourage à multiplication des naissances en captivité puisque le petit sont plus docile. Plus facile à manipuler, potentiellement moins dangereux et surtout extrêmement apprécié sur les réseaux sociaux. Ce sont des machines à l'AX qui pour la plupart sont font vivre une une vie entière en captivité. Après avoir été exploité pendant quelques mois. Cet amendement a donc pour objectif de limiter les contenus à des fins commerciales. Est-il besoin de le préciser, mettant en scène des interactions entre des femmes ou des hommes et des espèces non domestique. qu'est l'avis de la commission sur ces amendements. proposée par l'amendement 53 elles sont de bon sens. Sans toutefois être nécessaire cette proposition de loi responsabilise. C'est un des objectifs, l'ensemble des parties prenantes à un contrat d'influence commerciale dont les agents d'influenceurs et les annonceurs qui sont solidairement donc responsable en cas de dommages causés aux tiers, donc si à l'annonceur ou un agent d'influenceur propose un influenceur de faire la promotion d'un bien ou d'un service interdit par cette proposition de loi sa responsabilité sera donc engagé donc ce sera une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable pour cet amendement. 53. En ce qui concerne l'interdiction de la promotion de certains produits et services financiers. La commission des affaires économiques à adopter. Une rédaction de compromis. Qui permet à la fois de clarifier le cadre légal existant sans contraindre de façon excessive, le développement de la filière française des crypto-actifs. En particulier, il s'agit d'éviter de contraindre les prestataires de services actifs numériques enregistré mais dont aucun n'a encore été agréée par l'AMF. L'Autorité des marchés financiers. La réglementation européenne. Ah de toute façon rendu obligatoire un tel agréments à compter de 2024 ou de mi-2026. Il n'est donc pas souhaitable d'adopter un régime transitoire pour des raisons de souveraineté. Donc ici, nous sommes particulièrement sensibles où nous devons nous assurer que les retombées économiques de cette filière naissante bénéficie avant tout à nos territoires et éviter une fuite supplémentaire des influenceurs vers l'étranger. Ce sera donc un avis défavorable pour les amendements. 65 42. Qui reviennent au risque, je le redis, de revenir sur le compromis trouvé. Ce sera également un avis défavorable sur l'amendement 44 car tout investissement financier comporte un risque de perte. La question est toutefois de savoir jusqu'à quel point cette perte est taxé acceptable. C'est pourquoi il est déjà prévu d'interdire la promotion des contrats financiers les plus risqués. Notamment ceux pour lesquels les risques de pertes sont les plus importants. Difficile à évaluer et volatile. Enfin, sur l'interdiction des publications avec des interactions ou des mises en scène d'animaux sauvages non domestique. L'objectif de lutte contre la maltraitance animale et bien évidemment un sujet important. Mais j'attire votre attention sur le fait que les rédactions proposées dans le texte sont trop la rage car visant toutes les interactions avec des animaux sauvages non domestique. De plus, il n'est pas précisé si ces interactions ont lieu dans un but commercial ou non. Ne nous trompons pas, il s'agit pas ici de faire le débat sur cette cause qui nous tient tous à coeur, mais véritablement de nous concentrer sur le cadre encore une fois de cette où l'objectif de cette PPL. Qui est bien donc de réguler les publications commerciales des influenceurs et non pas de modérer l'ensemble des contenus qu'ils publient le risque serait aujourd'hui de contraindre. Une personne qui serait en vacances à l'étranger qui publierait un contenu avec un, un, un animal dans, dans le cadre de de ces loisirs donc je le redis, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le fond. Encore une fois que nous partageons. J'attire encore une fois l'attention sur le périmètre qui n'est pas définie en tout cas dans cette dans ce texte. Et donc, en résumé, ce sera un avis défavorable pour l'ensemble de ces amendements. Je vous remercie. Merci madame la présidente, je, je prends deux minutes. Que je ne reprendrai pas je n'abuserait pas de montant mais. J'ai vraiment à coeur de partager avec vous la la logique. De la position du gouvernement sur chacune des interdictions. Qui sont proposés, ici au au sein de cet article 2 B. Avec. Bruno Lemaire. Mais je dirais surtout avec les députés Vojetta et l'apport Que tout le monde regarde et qui sont haut et c'est assez républicains d'être présent. On a eu à coeur surtout de. De faire attention à respecter. De faire en sorte que les obligations. Posées aux influenceurs commerciaux soient strictement du même acabit. De la même qualité que celles qui existent sur d'autres canaux de communication là encore je reprendrai les mots de la rapporteure. Il ne s'agit pas, et je pense notamment monsieur le sénateur Gay à votre intervention sur l'alcool et la présidente Prima la rappeler. Il ne s'agit pas d'une position de fond sur l'alcool ou sur les animaux non domestiques. Pour autant, il s'agit du fait que nous sommes en train, enfin que vous êtes en train d'écrire le droit, la loi et que nous nous exposons les députés, les sénateurs s'expose avec ce texte, à des risques de rupture d'égalité injustifié, je vous le dis d'autant plus que j'en ai et je j'en ai fait les frais récemment sur certains textes. Ça n'est pas un mythe et ça existe. Donc si nous légiférons plus. Et si nous créons plus d'interdiction pour les influenceurs commerciaux qu'il n'en existe en droit pour les autres types de canaux de publicité ce risque de rupture d'égalité est vraiment important, il y a aujourd'hui une réalité, c'est que les influenceurs sont des créateurs, des acteurs économiques. Vous avez tout se rappeler et ils n'ont pas vocation à supporter plus de contraintes que les autres acteurs ça justifie d'ailleurs de rappeler dans l'Arctique chapeau de ah les grandes dispositions existantes et c'est bien pour ça que le deux a et décrit ainsi rappelons toutes les obligations et interdictions en matière de publicité et de communication. C'est pourquoi. Je le redis, le gouvernement aura un avis défavorable. Sans remettre en sur les les propositions d'interdiction supplémentaires sans jamais remettre en en cause les fondements et l'importance de chacun des sujets. Ça me semble important de le dire. Les seules exceptions sont celles où il n'existe pas à date de cadre tout court ou de Khadr suffisant. Comme nous en parlerons pour la chirurgie et la médecine esthétique au de le législateur pourra se saisir d'interdiction d'encadrement généraux qui ne s'applique pas uniquement aux influenceurs commerciaux et le gouvernement va proposer. Très prochainement, c'est-à-dire demain en conseil des ministres un projet de loi numérique qui précisera encore les choses. Pardon, madame la présidente pour cette. Insertion mais qui me semble important en termes de philosophie des interdictions oui strictement. Les mêmes que celles qui existent pour d'autres canaux. Pourquoi, parce que sinon nous nous exposons tout ça un vrai risque de rupture d'égalité et au fait que ce texte travailler portée par les députés et les sénateurs soit retoqué ce qui serait dommage. C'est pourquoi vous comprendrez qu'à l'exception de l'amendement 65 que j'ai porté au nom du gouvernement, j'aurai dans cette droite ligne exactement les mêmes avis sur l'ensemble des amendements, c'est-à-dire le 53, le Le 44 le 42 le 28, ce sera une demande de retrait et à défaut un avis défavorable je vous remercie. je comprends le scrupule en matière de solidité logistique exprimé par la rapporteure et quand nous sommes dans la même situation. Nous avons les mêmes préoccupations. Mais je ne peux pas la suite dans ses arguments. On nous dit que on interdirait de par ce cet amendement à un particulier de se prendre en photo quelque part avec un animal et ensuite de le poster sur le réseau mais c'est pas du tout ce qui est écrit deux et dit clairement est interdit pour les personnes exerçant l'activité d'influence commerciale de c'est à ça qu'on se rattache donc on est bien uniquement dans ce cadre-là on atteint pas, on n'attend pas. Aurait aux libertés individuelles puisqu'on cible précisément sur les personnes qui ont cette activité d'influence commerciale et le 2ème argument qui consiste à dire que l'on n'est pas dans d'un si dans une situation de promotion commerciale je pense y avoir répondu tout à l'heure dans l'exposé des motifs en rappelant que c'est ah traverse l'usage de ces animaux qu'on multiplie le nombre de clics et d'abonnés et que c'est ça qui est générateur donc en fait de ressources, donc en fait c'est une auto promotion. Donc on est dans une forme de promotion qui en plus entraînent directement la valorisation de la promotion commerciale qui est faite par la suite puisque c'est le nombre d'abonnés qui compte donc il me semble que tant du point de vue de la précision de qui on s'adresse et du respect des libertés individuelles que du sujet qu'on soit bien dans le le dans une question de promotion commerciale nous répondant donc à travers cet amendement à ces 2 préoccupations et vous avez dit pour terminer madame la rapporteure tout à l'heure qui avait promotion commerciale. Vous avez cité les éléments du code en disons que notamment quand il y a un bénéfice économique pour sa propre activité. Ben là c'est exactement le sujet il y a un bénéfice économique pour la propre activité de l'influence. Merci madame la présidente, je souscris évidemment à ce que vient de dire mon collègue dans la première rédaction de l'amendement. Vous disiez qu'il fallait spécifié que c'était pour des besoins commerciaux. Il s'agit bien évidemment de cela et il s'agit d'éviter. Alors d'abord que le Sénat soit logique à ce qu'il avait voté en novembre dernier par rapport à la condition animale par rapport à la d'intention d'animaux sauvages à la promotion de ceux-ci à des fins commerciales. Deuxièmement il s'agit d'éviter évidemment la banalisation et on est bien dans le cas d'un texte bien précises sur les influenceurs qui eux-mêmes affluence créer des effets de mode et influence dans le sens pour faire effectivement des lacs et suscité des succès commerciaux. Donc c'est bien. Dans le cas d'un d'un d'un texte qui est bien spécifique et qui va évidemment à l'encontre de ce qu'on souhaite pour la protection des animaux et surtout il faut quand même qu'il a une certaine cohérence politique dans ce que nous avions voté et on a pris en compte ce que vous disiez madame la rapporteure en re rédigeant les amendements dans le sens de ce que vous disiez. Et pour nous c'est tout à fait précis et dans un cadre bien précis. Je remercie. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Bon j'entends un argument développé par vous et par Madame la rapporteure. Sur le fait qu'il ne faudrait pas être plus dur avait les influenceurs que ce que nous permet. Dans le reste de la loi. Moi je pense que par exemple sur la question des 2 amendements sur les animaux. Il faut faire évoluer la loi et que ce que nous demandons et ce qui est demandé ici moi je les voterai. Nous le fassions dans tout l'espace public parce que je pense que c'est. Une question autour de la condition animale, nous avons déjà eu le débat ici sur lequel il nous faut faire beaucoup de progrès. Sur l'amendement de de monsieur Cabanel, moi je pense qu'il est extrêmement intéressant. Et là aussi. Pour l'instant. Il n'y a que chez les influenceurs ou les marques seraient elle. Se laverait les mains de ce qui se passerait dans la promotion de leur propre marque. Donc pareil je l'adopterai et puis pour finir sur les cryptomonnaies. Un désaccord leur profond avec. Madame la rapporteur. Loin de moi l'idée de vouloir interdire les cryptomonnaies, les NFT d'ailleurs tout ça et n'est pas égale. Ce que le copie Trading par exemple moi je pense que c'est une arnaque profonde et qu'il nous faudrait l'interdire. Faire croire à des gens qu'on va le leur apprendre à traîner en 30 secondes et qui vont se faire un porte-monnaie c'est faux. Une illusion mais sur les cryptomonnaies. Le NFT. Loin de moi l'idée de vouloir les interdire à loin de moi l'idée que nous voulions qu'ils partent tous que ça ne ruisselle pas dans leur dans notre économie et nos territoires. Je vous rassure, madame la rapporteure celles et ceux qui font ça sont déjà bien loin de la France et ne payent pas d'impôts mais. Sur la question de la cryptomonnaie. Et de NFT, par exemple, il ne se pose la question, que chez les influenceurs et de l'espace numérique parce que c'est là où se développe cette activité et donc c'est là en premier le où il faut l'encadrer. C'est pour ça j'appelle à voter ces deux amendements. Je vous remercie madame la présidente. Merci madame la présidente. Donc une nouvelle fois sans vouloir alourdir le débat, je pense que tous les débats qui sont menés ici sont justes mais qu'il ne faut pas les mener que sur les influenceurs et donc l'argument de Madame la ministre qui dit que nous risquons une rupture d'égalité devant la loi. Ivo sur tous les sujets que nous venons d'évoquer, il vaut sur les animaux il vaut sur l'alcool il va il va être valide tout à l'heure sur, sur les médicaments sur la chirurgie et il va y avoir un problème de rupture d'égalité devant la loi et cette rupture d'égalité devant la loi, elle met en péril le texte d'un point de vue constitutionnel. Monsieur Cabanel. Oui je, j'entends bien les les arguments de de madame. La présidente de la commission mais bon et effectivement j'ai j'ai j'ai du mal à comprendre parce que les frères et soeurs. Il y a un commanditaire qui. Appelle à ses services et donc je je je comprends pas vraiment pourquoi on sanctionnerait uniquement l'influenceur et pas le commanditaire. Donc c'est pour ça que je je comprends pas pourquoi le le le sept demain donc à a essuyé de 2 avis défavorables, même si j'entends ce que je viens d'entendre. Très bien, il n'y a plus de demandes d'explications de vote sur ces amendements. Je ne vois plus, je vais donc les mettre au vote. On va commencer par l'amendement 53 de monsieur Cabanel double avis défavorable qui est pour. Qui est contre. il n'est pas adopté le 65 du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour.

Qui est contre. Il est adopté.

Il n'est pas adopté et je pense que le 28 de Madame Boulay-Espéronnier tombe du fait de l'adoption de ce monsieur Bazin. Mais vous êtes satisfaite néanmoins Madame Boulay-Espéronnier.

Merci madame la présidente. Cet amendement concerne effectivement un sujet important. Nous sommes extrêmement inquiets. Certains d'entre nous sommes inquiets sur ces influenceurs qui prennent. une espèce de forme de médecins pour la jeunesse et donc effectivement, nous pensons que la santé physique et mentale de certains français. Est aujourd'hui menacée par la promotion de traitements médicaux de médicamenteux ou chirurgicaux sur les réseaux sociaux et on en voit les effets catastrophiques des personnes et notamment des jeunes parce que si on parle aujourd'hui d'influenceurs c'est parce que beaucoup de jeunes subissent ces influenceurs et ces jeunes en situation de mal-être sont la proie facile des influenceurs qui leur sujet à des traitements hors contexte médical qui ne leur conviennent pas nécessairement ils peuvent avoir des conséquences désastreuses, et parfois irréversibles sur leur santé, en particulier les influenceurs proposent toutes sortes de solutions miracle à des victimes fragiles et en souffrance qui espèrent ainsi résoudre leurs problèmes au guérir de leur maladie sans contrôle médical, je le précise. Cet amendement vise donc à interdire toute promotion sur les réseaux sociaux des actes procédés techniques méthode traitement médicamenteux et chirurgie pour lutter contre ces pratiques dangereuses. Les influenceurs n'ont aucune légitimité à pouvoir ces soins ou ses médicaments. Madame monsieur Salmon. Dans le lit. Le quatre. Merci madame la présidente. Cet amendement prévoit une interdiction de la promotion des produits de santé, dispositifs médicaux, ainsi que des compléments alimentaires, il ne vise pas à contraindre la liberté d'entreprendre, mais à protéger les consommateurs et à préserver la santé publique. Il s'agit de contrecarrer des pratiques problématiques créent le DVD sur les réseaux sociaux de conseils de santé inapproprié donné par certains influenceurs à destination du public et dont les conséquences peuvent être particulièrement dramatique, comme l'ont démontré les dérives de l'influenceur Dylan Thierry qui avait vanté des pilules aux propriétés miraculeuses prétendument en capable de remplacer la chimiothérapie. En effet une partie importante de la promotion effectuée sur les réseaux sociaux concernent des produits de santé. Si les influenceurs sont soumis aux dispositions du code de la santé publique concernant la publicité relative aux médicaments et aux dispositifs médicaux qui ne doit être ni trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique, il nous paraît nécessaire d'encadrer strictement la promotion de certaines typologies de produits lorsqu'elle contient des allégations de santé de bien-être et de performances physiques. Dans l'intérêt de la protection des consommateurs et de la santé publique. monsieur Bonhomme pour le deux. Merci madame la présidente. Comme ça a été dit l'obtention d'une autorisation de mise. Sur le marché de médicaments. Pour cela il faut que les indications d'utilisation de prescription soit strictement notifié par le laboratoire. La procureure demande ainsi que les conditions de création et les performances suisses spots sont ainsi impérativement détaillé par le fabricant malgré cet encadrement certains influenceurs se livrent sur des plateformes numériques à une promotion d'usage détourné de médicaments et de dispositifs médicaux. La conséquence, c'est que certains médicaments servant à traiter des pathologies graves comme par exemple le diabète peuvent se retrouver aujourd'hui hein de tensions dans le monde entier car leur usage est ainsi détournés de leur fonction première ne c'est notamment le cas de l'antidiabétique visait à réguler la glycémie qui est habituellement prescrit aux adultes souffrant de diabète de diabète de type 2. Parmi les effets secondaires notables. Il y a la perte de poids. Ainsi sur les réseaux sociaux ce midi quand même présenté par certains influenceurs comme une solution miracle pour maigrir. Ce phénomène. Venant des États-Unis a gagné évidemment la France et commence à être préjudiciable pour l'approvisionnement de ces traitements personnes réellement malade de plus en plus de pharmacies françaises également signal et déclare que des personnes non diabétiques se présente avec une ordonnance pour ce médicament. La conséquence directe de ce détournement et de la promotion qui en effet tu réseaux sociaux c'est que cet antidiabétique est considéré par l'Agence nationale de sécurité du médicament comme en tension et elle a sonné l'alerte il y a 2 mois. Il s'agit donc d'une prise et dévoyée de médicaments qui peut costume danger pour la santé de celui qui l'utilise à mauvais escient. J'ai une autre exemple aussi combien cernant la promotion de capteurs de glucose en continu qui sont utilisés à des fins. Esthétiques ou en cours pour améliorer les performances sportives. Je propose donc de mettre fin à ses usages détournés de certaines influences par certains influenceurs de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux sur les réseaux sociaux. Monsieur gardons. l'antidiabétique. Est hein. Je tiens à rappeler que c'était un médicament injectable qui permet de réguler la glycine. Il est presque il aux adultes souffrant de diabète de type 2, médicament dont l'un des effets secondaires notables et la perte de poids depuis plusieurs mois en France des influenceurs. On fait la promotion sur les réseaux sociaux et vante la vertu de l'amaigrissement de ce médicament. La Fédération française des diabétiques alerte sur ce phénomène qui s'intensifie. De plus en plus. Prendre ce médicament sans suivi médical est évidemment très dangereux pour la santé. Autre conséquence, certains médicaments Servent à traiter le diabète ils sont aujourd'hui en tension d'approvisionnement, ça a été dit tout à l'heure, la promotion de médicaments détournés de leur usage principal et donc un usage récréatif esthétique ou encore d'amélioration des performances est désormais courante sur les réseaux sociaux et d'ailleurs on peut citer d'autres exemples comme la promotion de la codéine, pour faire des cocktails, l'éducation non médical de certains médicament est très C'est la raison pour laquelle il faudra faire attention aux effets nocifs sur la santé et ça peut aussi générer de la dépendance, l'interdiction stricte de la promotion de l'usage détourné de médicaments. Nous sommes donc de voir tête préciser de manière très explicite dans la loi sur l'influence commerciale a donc pour objectif de lutter contre la promotion de l'usage détourné de médicaments et de l'interdire explicitement, je vous remercie. Merci madame la rapporteure qu'est l'avis de la commission sur ces amendements. Alors évidemment nous partageons votre constat. La vulnérabilité la crédulité ne devrait pas être un Business l'objet de cette PPL et justement de mieux protéger les consommateurs et d'identifier clairement ce qui est autorisé, ce qui est interdit en matière de santé publique. L'amendement hein et partiellement satisfait. Car de façon inédite. Cette proposition de loi prévoit une interdiction de la promotion de la chirurgie esthétique par les influenceurs, ce qu'il y ait une belle avancée, une grande avancée sur lesquels nous sommes unanimes. En tout cas sur ces dispositions. Mais le Champ d'application de l'interdiction proposée est beaucoup trop large. J'insiste, nous ne sommes pas dans les. Nous ne souhaitons pas faire que du symbole véritablement dans ce que nous votons aujourd'hui il s'agit surtout aujourd'hui de faire en sorte de ne pas proposer de dispositions dangereuses. Ou risque de créer une rupture d'égalité majeure avec ce qu'il est aujourd'hui possible et autorisé sur les autres canaux publicitaires. Je le redis. L'idée, ce n'est pas de de ne faire que du symbole en l'état actuel du droit, il existe déjà de nombreuses règles encadrant la promotion de produits de santé de médicaments. Elles sont rappelés à l'article 2. Ah de cette proposition de loi. Pour les mêmes raisons. Une interdiction générale et indifférenciée de la promotion de produits de santé, de médicaments et de compléments alimentaires, tels que prévu à l'amendement IV n'est pas souhaitable. N'oublions pas que cette proposition de loi est une première étape et qu'il s'agira de la faire vivre, de tirer un bilan de la mise en application de cette loi et pourquoi pas en effet d'aller plus loin dans un second temps les amendements de et 32 aborde également un sujet important. L'usage détourné des médicaments et des dispositifs médicaux. C'est un véritable enjeu de santé publique. Vous avez cité l'exemple d'anti-diabétiques utilisé à des fins détournées pour perdre du poids sur les réseaux sociaux on ne pouvant aller plus loin. On évoque d'ailleurs une nouvelle tendance à l'utilisation détournée d'anti-allergiques pour prendre du poids et tenter de ressembler à ces Stars complètement transformé surtout par la chirurgie esthétique d'ailleurs mais ce que vous proposez d'Inter 18 dire pardon est déjà interdit par le code de la santé publique et vous le savez et l'article de à rappel justement aux influenceurs les règles à respecter en la matière. La proposition, la publicité pardon des médicaments et dispositifs médicaux ne doit pas être trompeuses ni porter atteinte à la santé publique cette publicité doit notamment présenter le produit de façon objective et favoriser son bon usage, implique de respecter les dispositions de l'autorité de mise sur le marché, surtout les prescriptions thérapeutiques recommandées par la Haute Autorité de santé, autrement dit de ne pas faire la promotion d'un usage détourné. Par ailleurs il me semble que l'adoption en commission d'un nombre Visant à interdire, je le rappelle, la promotion de l'abstention thérapeutique par les influenceurs répond également à nos préoccupations à vos préoccupations en matière de santé publique. Ainsi l'exemple évoqué d'un influenceur incitant à l'abandon de la chimiothérapie pour faire la promotion de compléments alimentaires et couvert par cette nouvelle interdiction. Nous avons fait déjà de grands pas je vous propose, nous vous proposons un avis défavorable pour l'ensemble de ces amendements. Qui de l'avis du gouvernement. Je n'aurai qu'une référence vous rappeler à toutes et tous. Que l'intégralité de l'article 2

Tout ce que vient de dire la rapporteure cette exactement. Je n'ai pas une virgule à retirer l'avis du gouvernement. L'intégralité des publicités détournées. Usage détourné ou trompeurs. Tout ça est déjà puni par les 2 articles du code de la santé publique, je viens de mentionner, j'aurais donc strictement les mêmes avis que la rapporteur sur les amendements un quatre de 32 défavorable. Je vous remercie.

Merci madame la présidente. Moi je ne comprends pas bien à quoi sert ce texte Madame la Madame le rapporteur. On a un sujet de fond pour notre société avec les influenceurs. Voilà et ce texte concerne les influenceurs. On voit très bien que même s'il a des règles qui s'appliquent dans le code de santé et caetera, personne ne respecte parmi les influenceurs, ils font ce qu'ils veulent. Personne ne les contrôle personne finalement ne saisit une quelconque autorité sur des sujets de santé et les quatre amendements qui sont là dans ce sont des sujets de santé. Moi je voterai les quatres clairement donc sincèrement je ne comprends pas comment dans un texte qui concerne la limite que vous voulez donnez-vous Madame la Ministre aux influenceurs et les dérives qui qui en découlent. Comment ne peut-on pas écrire dans un texte que tous ces sujets liés à la santé. Alors excusez-moi la chirurgie esthétique. Je veux bien le Botox est jolie ma il y a pas que ça et c'est certainement pas le plus grave dans ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc la chirurgie esthétique. Oui pourquoi pas, mais il y a tout le reste tout le reste. Donc moi je suis désolé, je persiste à dire qu'il faut aussi que dans ce texte, on mette des limites sur tout ce qui est lié à la santé et en particulier pour protéger la jeunesse. Monsieur. Merci madame la présidente. Je je vous avoue que que je découvre en partie le texte j'ai travaillé quelques heures avant. Et donc j'ai je remercie d'ailleurs à la fois la ministre rapporteur de nous expliquer qu'il était la nuance entre la portée du texte et qui a passé à vivre et toutes les limites, et quelque part tout ce qui est déjà satisfait finalement à la fois par le droit existant et par la rédaction. J'ai entendu le débat concernant les médicaments, et je comprends tout à fait l'intervention. Je ne peux que soutenir les interventions de notre rapporteur et Madame le Ministre sur ce Champ là simplement la lecture, il y a un trou dans la raquette.

ça concerne la prudence psychologique d'un certain nombre de de de de de patients qui, dans leurs mesures de prises en charge sont reconnus par la chaise comme étant de bonne pratique. Mais le fait de le faire par Internet ou par le hé bien peut entraîner des contre-indications directe sur la prise en charge. Autrement dit vous êtes suivi par un psychologue. C'est un certain nombre d'actions, notamment en matière de handicap. Il y a pas difficulté, le fait de le faire à distance de l'non contrôlée. Eh bien ce n'est plus reconnu que maintenant un élément de sécurité HS, donc vous avez un trou dans la raquette.

Madame la ministre. ce que j'apprécie d'ailleurs. C'est un plaisir mais je voudrais juste dire que nous discutons un un texte d'origine parlementaire, porté par des députés, dans le cas d'une démarche transpartisane. Ce texte et je trouve les articles notamment un très important, il a vocation et on l'a dit toutes et tout je crois. Réguler une action économique. Il a aussi vocation à. Préciser les droits mais aussi les devoirs on arrivera sur le sujet des sanctions. Il a aussi vocation. À définir enfin ce qui est un influenceur commercial et ce quelle influence commerciale. Je voulais juste préciser parce que j'étais sensible à votre prise de parole, que ça n'est pas parce que en droit et effectivement j'ai émis la position du gouvernement et je n'y reviendrai pas. J'ai à coeur d'essayer de faire en sorte que ce texte puisse. Avancer le mieux possible, et faire en sorte qu'il ne soit pas retoqué. Je je pense que il faut aussi considérer ce texte dans ce qu'il apporte au domaine de l'influence commerciale et ne pas le regarder uniquement sous la houlette de l'interdiction. Je comprends votre sensibilité mais je n'adhère pas au fait qu'il y a sur ces dispositions. Des trous dans la raquette. Il y a 2 que je viens de vous romancier né du code de la santé publique et je pense que ce texte il est utile et je ne doute pas que vous rendrez toutes et tous, peu importe, nos divergences d'ailleurs encore plus utile, mais c'est un texte utile.

Du médicament de l'Autorité nationale de sud de la sécurité du médicament qui nous dit que par exemple l'Ozempic qui est un produit amaigrissant et totalement détournée de ses usages. Et si vous allez sur TikTok. Je sais bien qu'ici ce pas n'est peut-être pas les spécialistes de TikTok mais ça fait fureur. Et quand vous connaissez la CAF. Le caractère influençable. Des jeunes qui sont soumis à ces influenceurs et les effets sur notamment les stéréotypes de taille. Je pense que ça intéresse certains ici, on voit bien que tout ça passe en dehors des radars, alors Madame la Ministre vous vous contentez de dire. C'est punissable c'est puni. Oui c'est puni mais ce n'est pas puni c'est punissable. Mais ce n'est pas puni. Parce que la sanction elle elle y est pas. Donc il y a au moins un sujet de cet ordre-là que vous devriez. Ajouter au au sujet de savoir si c'est efficient si c'est opérationnel et si ça existe dans le code de santé publique, c'est quand même peut-être de donner des indications au toutes les autorités publiques pour que il y a des poursuites dans ce domaine parce que je peux vous dire que vu l'évolution technologique et vu la la diffusion de cette une technologie par TikTok et compagnie ça risque de se, de s'aggraver. Au point que on arrive à des tensions sur un médicament majeur qui concerne. Excusez du peu. La première main dit chronique en France que le diabète. Très bien. Madame la rapporteur. J'aimerais juste. Certainement pas synthétiser mais. Dire que. Là nous nous sommes en train de nous éloigner de l'esprit de cette PPL l'esprit de cette PPL ce n'était pas de. Renforcer pas renforcer pardon de la transformer en PPL basé sur uniquement des interdictions mais essentiellement dans un 1er temps, il s'agissait d'une première étape pour pour encadrer. Rappeler le cadre légal aujourd'hui qui doit être appliqué. Et certainement pas de contraindre à l'excès. Encore une fois toutes les activités qui se pose à nous mais on n'est pas en train de. Mais il ne transformez pas le débat, nous ne sommes pas en train de dire qu'aujourd'hui toutes les dispositions qui porte sur la santé publique ne sont pas importantes que nous tous les sujets ne sont pas importants. C'est pas du tout seul sujet c'est aujourd'hui de faire on l'a dit acte de pédagogie aujourd'hui il existe des dispositions qui ne sont pas connus par les influenceurs dont vous savez là le bâton. Ce n'est pas la principale. Réponse au contraire et donc ne transformez pas, s'il vous plaît. Le débat, il s'agit pas là aujourd'hui de dire que nous sommes contre les sujets de fond mais de dire qu'il y a un cadre et que notre rôle de législateur, c'est de façon réaliste de le rappeler et de le faire respecter. Merci. Très bien. Madame Benbassa. Je voudrais dire que je suis d'accord avec ma collègue. Puisque vous, vous l'avez pas insisté sur le fait que. OZEMPIC est en rupture de stock. Et les malades qui. Utilisent ce médicament n'arrive plus à se fournir puisque beaucoup de gens achètent ce médicament sans ordonnance également les, les pharmacies ont reçu un avertissement mais pour le moment les malades du diabète n'arrive pas à. Acheter ce médicament en pharmacie avec ordonnance, je crois que ce n'est pas en faisant appliquer tel texte ou tel texte qu'on va mettre fin à ces ruptures de stock liées à la promotion faite par les influenceuses et influenceurs merci. merci madame la présidente, madame la ministre madame la rapporteure. L'exercice de la médecine est très encadrée. L'exercice de la pharmacie est très encadré là dans le cadre des influenceurs. Il y a des achats sur Internet de médicaments. En plus, on s'adresse à des patients qui sont influençables car en situation de souffrance justement par ceux qui sont en situation de souffrance il vous s'engouffrer dans ces propositions qui leur paraissent miraculeuses pour essayer de les sauver en dehors d'un cadre thérapeutique légal donc il me semble que, en plus de l'abus de faiblesse. Il y a cet exercice illégal. Certes nous ne sommes pas là pour donner des interdictions. Mais tout de même nous sommes peut-être là pour essayer de protéger en particulier ses jeunes. Très bien je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 1 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

tout ça. Je crois que l'amendement est adopté. Et qui. Probablement, il fait tomber tous les suivants. Il va probablement c'est certainement et donc il est 20h 6 nous allons suspendre la séance elle sera reprise à 21h 35 pour la suite de l'examen de ce texte et la séance est donc suspendu.